La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation. Il y en a-t-il en séance. Je ne vois pas. Le procès-verbal est donc adopté sous les réserves d'usage. Madame, la Première ministre. Mesdames, et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance et retransmise en Direct sur Public Sénat et notre site Internet. Chacun sera attentif au respect de valeurs qui sont pour nous essentielles. Le respect des uns et des autres et le respect du temps de parole. Et. Je vais donner la parole à. Autre collègue Jérémy Bacchi pour le groupe communiste, républicain, citoyen Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous ne minimisons pas ce qui se passe à Mayotte depuis quelques temps les violences, les agressions au contraire la détresse de la population et l'insécurité qui règne sont insoutenables, notamment pour les plus faibles pour nous la seule solution envisageable pour résoudre cette spirale infernale est une réponse républicaine. Or, aujourd'hui, votre réponse est uniquement répressive, elle n'a pas digne des valeurs républicaines, détruire des bidonvilles. Expulser des sans-papiers ne permettront pas de rétablir la paix cela permet un vice-président du conseil départemental de Mayotte de dire tranquillement sur une chaîne de télévision que peut être il faut en tuer quelques-uns sur le fond, cet élu s'attaque violemment à nos valeurs républicaines et l'absence de réaction plus au niveau de l'État nous laisse un goût amer. L'opération Wambushu que vous avez déclenché est une atteinte à ses droits. On attendait la France de la France une réponse respectueuse du droit et de nos valeurs et non qu'elle se comporte comme chef de bande en effet vous démolissez des bidonvilles où vivent des Comoriens et des Mahorais, parfois très jeunes sans leur proposer de solution de logement digne, ne pas comprendre que les Comores sont à la fois plusieurs île avec des statuts différents, mais en même temps avec un seul et unique peuple c'est conduire dans une impasse toute tentative de résolution d'ailleurs le droit international et clair sur le sujet pour l'ONU c'est un archipel constitue même pays des enfants grandissent sans leurs familles au nom du droit du sol et se retrouve à survivre au quotidien la République doit s'incarner dans ce cas-là de meilleur à Mayotte et pas seulement sur le volet répressif alors que les droits les plus essentiels comme l'accès à l'éducation à la santé à l'alimentation un logement digne, ne sont pas assurés. Monsieur le Ministre, la détresse sociale est grande quand en dehors des réponses répressives à vous apporter des réponses sociales à la hauteur des attentes des mahoraises et des Maoris. Je vous remercie. Pour vous répondre. La parole est au ministre de l'Intérieur les bien. Monsieur Gérald Darmanin. Vous avez la parole. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, permettez-moi de vous dire que tout est scandale dans les propos que vous venez de tenir. Vous venez de vous asseoir sur la constitution de la République. Je vous rappelle que ces ces assemblées le président Chirac qui a inscrit Mayotte dans la Constitution. Vous venez de dire que Mayotte n'était pas française mais qu'elle était comorienne, c'est-à-dire que pour un représentant du peuple français au siège ici des représentants de Mayotte. Vous partez du principe que la France n'est pas chez elle à Mayotte. Alors que les Maoris ont choisi par de référendums dans les années 70. Monsieur le sénateur, et alors même que vous participiez à d'autres gouvernements de parti des années après, ils ont choisi librement de rester français. Vous venez de dire. Que la France se comporte en chef demandent qu'on nous interpellons au péril des policiers, des gendarmes, tous les jours et toutes les nuits justement des bandes criminelles et c'est le premier objectif de cette opération on ou que nous lançons à la demande de tous les élus mahorais et même du responsable et les filles de Mayotte, ça mérite quand même d'être soulignée, je peux vous envoyer son communiqué de presse que vous n'avez manifestement pas eu l'occasion de dire dans votre question d'actualité. Oui, monsieur le sénateur. Ce que veut le gouvernement fait ici à Mayotte. C'est ce qu'il aurait dû faire depuis très longtemps. Interpellé les bandes cassé et la spirale incroyable des bangas sert des habitats. Illégaux où vivent des enfants, des vieillards, des personnes handicapées qui n'ont ni eau ni électricité, ni gaz. Et oui, oui, monsieur le sénateur, l'immigration irrégulière est inacceptable dans notre département comme à Mayotte, c'est-à-dire dans toute la France. Monsieur le Ministre, je ne dis pas que la France ne doit pas agir, ce que je dis c'est qu'il y a des conditions aujourd'hui qui aggrave la situation le VISA Balladur par exemple en est un parfait exemple aujourd'hui qui ne fait qu'aggraver pour le coup ce fossé qui existe entre les différentes z'île comorienne et je crois qu'il est grande tentes de l'abroger. Merci. La parole est à d'autres collègues. Thani Mohamed Soilihi, ni pour le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Il avait la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer depuis quelques jours l'Hexagone découvre avec effroi les immenses difficultés auxquelles le département de Mayotte est confrontée, immigration, gestion de l'eau, assainissement, logements insalubres, la liste est longue. Les chiffres les plus difficiles à accepter. À mon sens sont ceux qui touchent notre jeunesse. Laquelle représente plus de la moitié de la population. Un système de rotation. Il n'a inédits et inacceptables liés à un manque crucial d'infrastructures hein traîne 75% de décrochage scolaire. Quand le niveau national et de 10% les problèmes s'accumulent et s'amplifie depuis des décennies. C'est le cas de l'insécurité alimentée par la multiplication des gangs et l'immigration illégale et massive. Une situation, je le répète avec force ici sans égal dans le reste du territoire français. L'opération Bouchoux que vous avez eu le courage d'engager. Monsieur le Ministre et une réponse forte, très attendue par la population, elle n'est ni honteuse ni glorieuse et les nécessaires pour réaffirmer l'autorité de l'État et protéger nos compatriotes de Mayotte elle tranche avec l'inertie de ces dernières années. Je veux ici, rendre hommage à nos forces de l'ordre à leur engagement sans faille ou en Bouchoux, qui signifie reprise hein shimaoré se fixe comme objectif de restaurer le droit à la sécurité, mais demain il faudra aussi envisager et Wambushu de l'éducation de la santé, de l'Aménagement et du logement. Monsieur le Ministre, alors que cette opération vient à peine de débuter les Mahorais sont inquiets. Pas la suspension des reconduites à la frontière vers les Comores ainsi que par certaines décisions judiciaires qui ne sont pas toujours. Comprise. Quelles mesures supplémentaires attendez-vous déployés pour que cette promesse de retour à l'ordre républicain soit un succès. On vous répondre. La parole est à. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, madame c'est 7h. Monsieur le sénateur, d'abord je veux dire que c'est à votre initiative et à celle des élus mahorais que l'État, sous l'autorité de la Première ministre a décidé d'engager à Mayotte. Des moyens sans précédent des moyens sans précédent. Pourquoi d'abord pour maîtriser la démographie. Le problème de cette magnifique île de Mayotte qui pourraient être plus belle encore que sont les Bahamas ou les Seychelles, vous le savez mieux que personne. Avec ce lagon incroyable c'est qu'il est ce ce ce territoire déstabilisé par une population qui malheureusement fait dériver des services publics, quel qu'il soit ça explique de la sécurité. Le service public de l'éducation. Je rappelle qu'à Mayotte, vous le savez, les enfants quand ils vont à l'école, vont à l'école qu'une demi-journée par jour parce qu'il n'y a pas assez d'établissements scolaires poursuivent la démographie qui arrive. Déstabilisé en santé, 80% des enfants qui naissent à l'hôpital de Mamoudzou ne sont pas nés de Mahorais et 900 parturientes chaque année sont accoucher par les sapeurs-pompiers de l'île de Mayotte, ce qui montre une difficulté bien sûr de sanitaire pour notre pays. Difficultés sociales de manière générale, du fait de cette démographie donc d'abord il s'agit de la reprise de la sécurité. Je l'ai dit, vous savez sur les 60, objectif de la police judiciaire, 22 ont déjà été interpellées, présenté en 15 jours au service de monsieur le garde des Sceaux et nous espérons qu'ils vont appliquer des décisions de justice qui sont prononcés qui sont fermes. Entre 7 et 10 ans de prison pour la plupart des personnes que nous avons interpellé ensuite la destruction des Mangas. Le ministre du Logement nous a mis à disposition tous les relogements possibles et contrairement à ce que j'entends évidemment que tous les mineurs non seulement ne sont pas reconduits à la frontière mais en plus sont logés et accueilli dans les services de l'enfance. Merci le département et la secrétaire d'État à l'enfance et oui nous luttons contre l'immigration irrégulière Sri Lanka Madagascar Afrique des Grands Lacs certes tous déstabilisé pour de réseau pour une autre et bien évidemment les Comores avec lequel nous continuons à discuter. Nous continuerons notre travail et je laisserai ce actualité la Premier Ministre les policiers, les gendarmes autant d'autant qu'il le faudra à Mayotte pour que Mayotte se sentent comme n'importe quel département français. La parole est à notre collègue Rémi Féraud. Pour le groupe socialiste écologique. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, quelques jours après votre passage en force pour imposer la réforme des retraites et sa promulgation par le président de la République. Même l'agence de notation Fitch a sorti sa casserole en abaissant la note de la France. Certes. Et même si leurs appréciations ont des conséquences. Pour notre part nous ne reverrons pas les agences de notation mais toute votre action, elle est faite pour satisfaire leurs exigences reconnaissait ainsi que votre politique n'est pas seulement injuste elle manque aussi d'efficacité et elle crée de l'inquiétude. Or vos annonces en matière budgétaire ne sont pas rassurantes non plus parce que derrière le flou et les contradictions de votre programme de stabilité se cachent à l'évidence des mesures d'austérité sur la solidarité et les services publics parce que vous parlez de revue des dépenses mais vous refusez obstinément toute mesure de justice fiscale. Votre méthode brutale conduit à une telle crise sociale et démocratique qu'inquiète même les marchés financiers. Alors il vous faut aujourd'hui changer de gouvernance pour redonner une perspective au pays est un espoir aux Français. Monsieur le Ministre, allez-vous vraiment attendre 100 jours pour prendre acte de l'impasse dans laquelle et le gouvernement. Allez-vous vraiment attendre 100 jours pour changer radicalement de méthode et donner à votre action un nouveau cap qui soit plus juste mais qui soit aussi plus claires et plus efficaces.

Je vois que vous lisez des bons auteurs madame la sénatrice. Il y a un peu d'inconséquences. je vois votre sourire. Il y a un peu d'inconséquences. Dans votre question, monsieur le sénateur, à la fois vous regretter la décision de l'agence de notation Fitch dont nous prenons acte avec la Première ministre hein et dans le même temps vous nous dites qu'il ne faudrait pas réduire les dépenses publiques réduire la dette et rétablir les finances publiques de la France. Nous nous sommes conséquent. Nous avons en 2017 et 2018 rétabli les finances publiques de notre pays, nous sommes revenus sous les 3% de déficit et nous sommes sortis de la procédure pour déficit excessif. Ensuite nous avons eu à faire face à 3 crises successives. La crise des gilets jaunes. La crise du Covid et la crise de l'inflation et à chaque fois, nous avons pris les mesures de protection nécessaires pour éviter les conséquences à nos compatriotes sur les salariés sur l'emploi, sur l'industrie sur les entreprises de notre pays. Maintenant que nous sortons de cette période de crise et j'ai bon espoir que nous sortions de la crise inflationniste dans le courant de cet été. Nous revenons à la normale. Il est temps de rétablir les finances publiques de la France, nous avons engagé avec la Première ministre une revue des dépenses publiques. Je tiendrai des assises des finances publiques au début du mois de juin pour regarder comment aller plus loin dans la réduction à dépenser le rétablissement de nos finances publiques, nous allons accélérer le désendettement de la France et nous ne faisons pas ça pour quelques agences de notation, que ce soit nous le faisons pour les Français pour l'indépendance de la France et pour la souveraineté nationale. Monsieur le Ministre, j'ai pas lu tous les derniers romans mais j'ai lu l'appréciation de Fitch et elle conteste votre méthode sans forcément contester vos objectifs. Moi je vois que vous risquez d'aggraver encore votre politique et de maîtriser les dépenses publiques en sacrifiant encore davantage la solidarité les services publics, les investissements d'avenir et encore une fois sans prélever leur juste contribution sur les plus riches sur les grandes entreprises sur les multinationales comme le demandent les Français, après cette période si douloureuse et si injuste. Voilà ce que j'avais à vous répondre, et j'espère que nous pourrons avancer. Monsieur le Merci monsieur le président, ma question s'adresse à monsieur le ministre dans l'agriculture et de la souveraine. La souveraineté alimentaire. Depuis plusieurs mois la filière noir traverse une crise sans précédent avec des cours qui s'effondre de près de trois zéro le kilo nécessaires pour couvrir les frais de production les noix partent actuellement quand elles partent au prix de 50 centimes à l'euro le kilo. Pourquoi cette crise. Elle est liée à la conjonction d'une surproduction mondiale et en France d'une chute de 30% de la consommation de loi magasin là non. N'étant pas considéré en période d'Elfassi ont comme un produit essentiel, malgré ses qualités nutritionnelles reconnues. gagne les producteurs qui soient du loft de la Dordogne ou de la Corrèze avec la noix du Périgord. La de la vallée de la, de l'Isère avec la noix de Grenoble ou d'ailleurs avec des problèmes de trésorerie, de stockage et de conservation des lois un frigo pour qu'elle n'aura ainsi ce pas alors que faire. Une réflexion est en cours pour déterminer une stratégie globale de commercialisation et de communication de la filière française sur plusieurs années dans le Lot un travail a débuté avec la MSA, la culture DDT. Pour un ciblage face avec une prise en charge des cotisations sociales pour les exploitations en grande difficulté. Mais cela ne sera pas suffisant. En attendant, la profession demande le déblocage d'un fonds d'urgence gérés localement au plus près des besoins pour répondre à la crise. Il vous est également envisagé un retrait du marché des noix de qualité moyenne et une campagne d'arrachage. Monsieur le Ministre, quelles mesures envisagez-vous de prendre pour venir en aide à c'était si hier qui pèsent lourd dans l'économie de nombreux départements.

Sur une fille. Alors c'est assez paradoxal au fond parce que. On est dans une filière qui est plutôt en crise de croissance. Ce que vous avez décrit, c'est plutôt une filière sur lequel la demande mondiale est plutôt croissante du fait d'ailleurs de ce qu'on appelle le phénomène du snacking. Et en disant plus plus 50% de surface. En noix et donc c'est ça aussi qu'on a sous les yeux, c'est une crise de croissance dans un contexte d'une surproduction cette année de conditions climatiques et d'une condition de marché qui crée ces conditions là, je rappelle que la France est le premier exportateur européen le 4ème exportateur mondial et c'est bien là dessus qu'il faut qu'on essaye aussi de travailler pour conforter cette souveraineté qu'on a sur cette filière sur cette filière de noix. Alors vous me demander les réponses qu'on peut apporter. Vous en avez cité un certain nombre. La première c'est sans doute un, un travail que nous devons faire en terme de communication, y compris avec la grande distribution. Ça c'est à l'intérieur de nos frontières pour mieux valoriser la noix et faire en sorte qu'on puisse déstocker ce qu'on a en trop cette année. Deuxièmement, c'est un travail que nous devons faire à l'extérieur de nos frontières européennes et mondiales pour valoriser encore vous avez indiqué les signes de qualité qui sont les nôtres, pour faire en sorte que là aussi on puisse développer les choses, de on a des outils de régulation je l'ai dit aux acteurs de la filière que j'ai rencontrés il y a un peu plus d'un mois. De se saisir des programmes opérationnels puisqu'à leur demande, ils peuvent intégrer ces programmes opérationnels et ça permet d'intégrer des mesures de retrait, donc des mesures de régulation de marché, il a une semble que c'est un élément important et donc je je l'ai recontacterai aussi pour leur dire qu'ils peut se rapprocher de France AgriMer il me semble être un élément important,

C'est le travail que nous faisons sur le plan de souveraine très fruits et légumes, la filière fait partie de cette grande famille des fruits et légumes, même si ça là c'est plutôt les coqs pourrait-on dire, et donc on va travailler avec eux, à la fois sur les questions phytosanitaires comment on arrive à réduire les produits en même temps, garder de la compétitivité et par ailleurs comme on fait en sorte d'ouvrir de nouveaux marchés. Donc la communication les outils de régulation sur les stocks, la vocation exportatrice qui font conforter et deuxièmement, le plan de filière fruits et légumes.

Monsieur le ministre. L'eau est un bien commun et sa gestion durable une nécessité vitale. Aujourd'hui, les sécheresses sont redoutables et de plus en plus brutale des dérèglements climatiques s'accélère et notre adaptation n'est pas à la hauteur parce qu'elle n'intègre pas suffisamment l'articulation entre les interventions d'urgence nécessaire et les interventions structurelles qui sont-elles indispensables. C'est pourquoi je m'adresse à vous Monsieur le Ministre Bruno Lemaire depuis plusieurs jours, le maire de la ville de Grigny dans l'Essonne discute avec l'usine locale de Coca-Cola pour que l'entreprise arrête de puiser de l'eau dans la nappe phréatique en Isère STMicroelectronics. Qui a bénéficié de 2 3 milliards d'euros d'argent public va consommer près de 29.000 mètres m3 jour l'équivalent de la consommation d'une ville de 100.000 habitants en Bretagne, l'installation de l'usine bride or fait l'objet de contestations par sa consommation de Terres agricoles et le manque de ressources en eau pour chacun de ces exemples des solutions de réutilisation et de recyclage de l'eau existe les procédés sont coûteux et sans volonté exigence politique sans conditionnalité des aides à la gestion de l'eau, la gestion de l'eau passera toujours au second plan. Monsieur le Ministre, vous supprimez la CVAE et renforcer les aides fiscales mais quelle contrepartie exigées vous pour que les projets de réindustrialisation soient économes en eau et en ressources naturelles. Monsieur le Ministre, nous soutenons la réindustrialisation utile de notre pays car on peut être écologiste et pour l'industrie. Mais peut-on être libéral et soucieux de l'écologie. Combien de milliards consacrés-vous à cette exigence de réindustrialisation compatible avec le dérèglement climatique. Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur. Vous-même dans votre intervention. Expliquait qu'on pouvait être écologiste et en faveur de la réindustrialisation. Je vous prends au mot et je vous réponds. Pendant trop d'années. Ce n'est pas une critique et ciblées contre qui que ce soit parce que malheureusement elle pourrait concerner beaucoup au cours de ces dernières décennies pendant trop d'années, on a fait de l'écologie grâce à la désindustrialisation. C'est-à-dire qu'on a baissé nos émissions puisqu'on a fermé des usines. Et que dans le même temps, au moment du diminuons nos émissions nationales on augmenter notre empreinte puisqu'on s'est retrouvés à importer des produits qui venaient de l'extérieur Que la réindustrialisation permet de retrouver des circuits courts et de s'inscrire dans cette logique. C'est non seulement quelque chose de souhaitable, mais c'est exactement le chemin que nous devons suivre et ce sera au coeur du projet de loi industrie verte qui sera présentée par Bruno Lemaire et qui évidemment accompagné par le ministère de la transition écologique Bien sûr il y a des défis dans cette réindustrialisation et dans ces défis. Il y a la gestion des ressources naturelles. Il y a celles qui concernent le foncier disponible. Il y a celles qui concernent la formation et les hommes et les femmes qu'il faudra faire en sorte d'orienter et il y a bien entendu la question de l'eau. Sur l'eau. La trajectoire globale, elle est simple, c'est celle de la sobriété, quelles que soient les usages, ce que disent les rapports du GIEC, c'est que l'eau dont nous disposons ça moins nombreuses puisque l'augmentation des températures augmentera l'évapotranspiration, et que parallèlement la végétation absorbera une part plus élevée. Et c'est exactement ce qui explique que, au-delà de cette trajectoire de sobriété. Nous devons optimiser les usages dans les optimisations d'usage. Vous citez Grigny. Une usine Coca Cola pompent dans la nappe phréatique. Il y a des alternatives technologiques qui permettent aujourd'hui avec des procédés de réutilisation avec des dispositifs sur place de pouvoir éviter ce type de choses, je ne peux pas croire. Que vous disiez terminez votre intervention en disant que vous étiez favorable à la réindustrialisation et que dans le même temps. Confronté à la réalité de certains projets qui permettent de créer des emplois en proximité et d'éviter une empreinte carbone désastreuse. Vous vous abrite lui et ensuite derrière forcément les difficultés mais les chemins que nous avons à construire pour rendre possible cette réindustrialisation verte de notre pays. Monsieur le Ministre, en l'absence de réponse du ministre de l'industrie. Je voudrais vous dire que nous prônons la relocalisation depuis longtemps car c'est une condition de la transition de la transition écologique indispensable mais l'industrie ne doit pas seulement être décarboné. Comme vous le revendiquez. Elle doit être réellement verte c'est-à-dire socialement utiles soutenable et économe en eau les arbitrages sur les prélèvements d'eau doivent être transparents décider démocratiquement et exigeant en termes de modération des prélèvements pour préserver les milieux. La parole est au président Claude Malhuret, pour le groupe les indépendants République. Après Après l'incendie d'écart de gendarmerie il y a un mois à Sainte-, Soline le 1er mai à Paris, ce sont les policiers eux-mêmes qui ont été transformée en torche vivante. Semaine après semaine, l'ultra gauche et les Black blocs programme l'escalade. Avec pour objectif l'insurrection. Balayé la réforme des retraites. Le guide suprême de la France soumise à Poutine, vêtu d'un manteau de cuir qui aurait fait fureur dans les années 30 nous a expliqué lundi avec les gestes de la main et du menton en vogue à l'époque qu'il fallait je cite. Mettre à bas la mauvaise République ce n'est pas un énième et de dérapage verbal, hier à l'Assemblée un de ses sous-fifres s'est chargé de l'exégèse lors des questions au gouvernement, il commence à s'adressant à vous madame, la Première ministre policier brûlé les coupables chez vous il continue la Ve République permet d'agir sans le peuple et contre lui. Elle n'est plus légitime. À bas Macron et la mauvaise République vive la Constituante et la VIe République, le 14 juillet, vous aurez votre prise de la Bastille. Cette névrose obsessionnelle de se croire chaque jour le 13 juillet 89. Comme d'autres se prenne pour Napoléon pourrait sembler le mériter qu'une consultation à Sainte-Anne. Mais méfions-nous. Les émeutes et parfois même les insurrections ont souvent été déclenchée par des dingues et je conseille à ceux qui ne l'ont pas encore fait de se documenter sur la VIe République que nous propose la France irrécupérable la cinquième serait vite regretté comme un modèle de démocratie. Cette tenaille entre les violences dans la rue et la zadisation de l'Assemblée nationale qui dure depuis des mois est en train peu à peu de saper la confiance des Français dans leurs institutions et de dissoudre lentement le respect pour l'ordre républicain. Dans ce contexte, je veux rendre hommage au jeune policier de 27 ans brûlée avant-hier est toujours hospitalisé, mais aussi aux 405 membres des forces de l'ordre blessés depuis ce jour-là et oh 1083 blessés depuis le début de l'année en accomplissant leur mission et vous poser ma question, comment adapter notre Cenal juridique pour mieux protéger nos forces de l'ordre face aux voyous organisés parasitant désormais toutes les manifestations avec pour seul but de casser du flic.

Lundi à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans notre pays. Dans la très grande majorité des villes grâce à la responsabilité des organisations syndicales et à l'engagement des préfets et des forces de l'ordre. Les cortèges ont pu défiler sans heurts et les idées s'exprimer pacifiquement. Malheureusement, vous l'avez souligné, Monsieur le Président. Une fois de plus, dans plusieurs villes comme Paris, Lyon, Nantes ou Rennes. Des casseurs, décidé à en découdre avec les forces de l'ordre se sont infiltrés dans les cortèges et ont provoqué des violences parfois très graves. Et en disant ces mots je pense aux commerçants, aux élus, aux habitants qui ont découvert hier matin leur vitrine leur mobilier urbain ou leur voiture. Avec de lourds dégâts. Je pense aux manifestants que ces casseurs mettent en danger, sans hésiter, je pense aux parlementaires, dont les domiciles ont été visés aux militants dont certains ont été pris à partie. Je pense enfin et bien sûr à nos forces, nos forces de l'ordre attaqués dans plusieurs villes dans un déchaînement de violence. Plus de 400 policiers et gendarmes ont été blessés lundi certains gravement et la France entière a été choquée par les images du policier grièvement blessé par un cocktail Molotov. Alors je veux dire aux policiers et aux gendarmes ma solidarité et mon soutien. Celui de mon gouvernement et je n'en doute pas celui de tous les élus dans cet hémicycle. Et je le répète devant vous. Les auteurs de ces exactions doivent être identifiés et traduits en justice. Aujourd'hui, certains continuent à mettre en cause les forces de l'ordre excusez les casseurs occulter les violences, c'est l'honneur de nos policiers et de nos gendarmes de protéger la liberté d'expression, la liberté de manifester. Nous sommes et nous resterons à leurs côtés. Toutes les mesures susceptibles de renforcer leur protection dans le respect des libertés publiques seront étudiés. Monsieur le Président, vous évoquez également les nouvelles outrances du leader de la France insoumise. Elles s'inscrivent dans une remise en cause permanente de nos institutions, elles sont une nouvelle étape pour Seif sapé la confiance de nos concitoyens dans notre démocratie. Ah bah la mauvaise République dit-il, chacun le sait bien. Pour Jean Luc Mélenchon Mélenchon. La seule bonne République c'est lui. Pour notre part nous sommes et nous resterons du côté de la République et de l'Ordre républicain je vous remercie. La parole est à notre collègue. Le président François Noël Buffet pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, Merci monsieur le président, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. J'ai le Ministre vous portez depuis quelques jours une opération d'envergure à Mayotte de lutte contre l'immigration irrégulière. Dans ce territoire un peu particulier. Ont-ils été rappelé tout à l'heure par notre collègue Thani Mohamed Soilihi. Les circonstances de vie de l'ensemble de nos concitoyens. 50% de la population est étrangère et 50% de cette population est en situation irrégulière depuis de nombreuses années, nous nous constatons constatons pardon. Une augmentation des actes de violences de toute nature. Aujourd'hui dans votre opération, vous vous heurtez à la non-réadmission d'une partie de ces gens en situation irrégulière à Anjouan ou en comment Où en êtes-vous aujourd'hui des accords de réadmission. De la part de ce pays de ce que nous tentons d'expulsés de Mayotte. Car sans réussite et sans obtention de ces fameux laissez-passer consulaires devenue aujourd'hui beaucoup trop célèbres, je pense que l'opération se rate en difficulté. Nous avons besoin de comprendre et de savoir l'état de la situation et l'état des discussions avec les dirigeants des Comores. Pour vous répondre. La parole est au ministre de l'Intérieur, des outre-mer. aurait pu. Largement répondre à cette question. Mais bien sûr. Vous rassurer sur le fait que nous avons avec les Comores une coopération efficace depuis 4 ans puisque, chaque année je prends l'exemple de l'année dernière 25.000 reconduites à la frontière, dont 100% des personnes comorienne qui ont été condamnés par la justice française ont été renvoyés aux Comores avouer, vous qui connaissez très bien ces questions que ses résultats. On aimerait les avoir avec d'autres pays, donc nous avons avec les Comores évidemment une bonne coopération, dans la circonstance dans lequel nous sommes rappeler d'ailleurs par le sénateur du groupe communiste, il y a une revendication, vous le savez historique des Comores a récupérer je mets évidemment des guillemets, l'île de Mayotte et dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, aujourd'hui, je pense bien évidemment aux circonstances électorales qui touchent la partie comorienne. Nous avons des discussions qui pour l'instant font que il n'y a plus d'échanges, pas simplement entre étrangers en situation irrégulière et laissez-passer consulaires mais entre personnes qui viennent de Mayotte pour aller vers les Comores et des Comores pour aller vers Mayotte et si j'étais encore plus précis d'Anjouan surtout pour venir à Mayotte qui n'a pas toujours, vous le savez bien la même position que Moroni et donc aujourd'hui. Depuis 5 jours. Il n'y a plus d'échanges de bateau, officiellement pour des raisons techniques au port d'Anjouan entre Mayotte et les Comores qu'il s'agisse des étrangers en situation irrégulière ou qu'il s'agisse de simples voyageurs. Tout à fait réveillé des 2 côtés de la frontière et de la mer. Nous utilisons tous les moyens diplomatiques pour renouer le contact, j'ai eu moi-même 3 fois cette semaine. Le ministre de l'Intérieur, je l'ai d'ailleurs invité à venir me rejoindre. À Paris, il a accepté cette invitation dans quelques heures, dans quelques jours, je le recevrai pour reprendre la coopération avec les Comores. Si nous continuons les 25.000 reconduites à la frontière. Chaque année, nous arriverons à tenir notre objectif de lutte contre immigration irrégulière à Mayotte, puisque vous savez que le problème particulier n'est pas tellement la reconduite à Mayotte. Mais l'arrivée des kwassa-kwassa et je veux ici constater que la mobilisation de la Légion étrangère, la mobilisation des policiers, des gendarmes en non mais il y a 1500 policiers gendarmes à Mayotte en ce moment faut qu'il y a quasiment pas d'arriver de kwassa-kwassa et donc si nous reprenons les reconduites classique en lien avec nos amis des Comores tout en empêchant l'arrivée des kwassa-kwassa nous aurons limiter fortement l'immigration irrégulière à Mayotte. Je précise pour dire qu'il faut aussi changer le droit à Mayotte. On a eu l'occasion de faire des propositions, nous en parlerons peut-être dans un texte immigration discuteront bientôt nous l'espérons tous, monsieur le président de la commission des lois, mais aussi dans le débat constitutionnel que nous pourrons va avoir demain ou après-demain allemand du président de la République, j'ai déjà dit que j'étais favorable, la modification du droit du sol à Mayotte pour limiter notamment cet appel d'air sur le territoire mahorais. Avec impatience le texte immigration pour essayer d'apporter effectivement une réponse. Nous l'attendons. Et comme soeur Anne, pour l'instant, nous ne voyons rien venir, mais peut-être que cela viendra et, et en tous les cas nous ils passeront le temps qu'il faut cependant. C'est vrai qu'il eut été utile que nous l'ayons car je pense qu'il reste, je suis convaincu qu'il faut maintenir dans le texte l'idée qu'il ne peut pas y avoir de VISA s'il n'y a pas de laissez-passer consulaires on mettra pas en place. Un rapport de force puissant avec les les pays sources nous aurons beaucoup de mal et la situation risquera de se continuer telle qu'elle est aujourd'hui mais je crois que pour Mayotte. La solution n'est pas seulement celle-ci elle est évidemment substantielle mais il faut donner un avenir à Mayotte, lui donner un projet, un projet économique et un investissement de long terme qui seule sera à terme le garant d'une vie normale de nos concitoyens mahorais. Merci. La parole est notre collègue Stéphane Demilly. Pour le groupe de l'Union centriste. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre de l'économie. Cela a été dit vendredi dernier, l'agence de notation Fitch a dégradé la note de du crédit de la France, la faisant passer de double à à double à moins. Pour justifier sa décision. L'Agence évoque notamment je cite des déficits budgétaires importants et des progrès modestes. Concernant la réduction des déséquilibres cela après 3 ans d'abondantes dépenses publiques destinées à amortir le choc du Covid et de l'inflation. Comme les 2 autres agences de notation très connu. Et ça ne et Moody's. La principale activité de Fitch consiste à évaluer la capacité des États à rembourser leurs dettes en leur attribuant une note matérialisée par des lettres. La meilleure note et triple A pour signifier un crédit de qualité optimale. Ce que nous avions d'ailleurs avant 2012. La pire et C ou D où on se rapproche du défaut de paiement. La note de la France a donc été dégradé d'un cran vendredi dernier. Cette décision, comme l'a constaté l'OFCE va à contre-courant du signal envoyé au marché par le gouvernement avec l'adoption de la réforme des retraites, une réforme censée attester d'une volonté de maîtrise des équilibres budgétaires à long terme. Mais avec cette note. La réalité est aujourd'hui tout autre. S'il y a une perte de crédibilité de notre pays sur sa capacité à rembourser sa dette. Nous serons hypothétiquement amenés à emprunter plus cher sur les marchés donc à payer plus d'intérêt. Cela grèvera les finances publiques et nos marges de manoeuvre budgétaires qui sont nous le savons tous, déjà très contraintes. Rappelons que la charge de la dette publique est passée en quelques mois, de 37 à 50 milliards d'euros. Alors concrètement, Monsieur le Ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour que nous retrouvions sur les places financières internationales. Un Label de confiance et de crédibilité rassurant pour nos prêteurs. Et pour le dire autrement, Monsieur le Ministre, comment comptez-vous enrayer cette dégradation de la notation de la France.

à la bonne tenue des comptes publics. Et je sais pouvoir compter sur vous pour adopter dans quelques semaines à la loi de programmation des finances publiques qui nous permettra de donner le cadre de ce rétablissement. Première remarque. La France n'a pas de difficulté à lever de la dette sur les marchés. 2 agents se sont prononcés il y a eu une dégradation de Fitch Moodys en revanche, le rappel n'a pas jugé bon de modifier la notation de la France et nous attendons la 3ème décision qui soit celle de l'agence Standard dinde au début du mois de juin. Je constate également que sur les marchés, vous m'interrogez sur la précision des chiffres. Le spread avec l'Allemagne a peu évolué de 50 à 59 points de base. Preuve que il y a une véritable solidité de la France ce qu'elle émet de la dette sur les marchés. Je rappelle que pour l'Italie ce spread est de l'ordre de plus de 180 points de base. Donc gardons notre sang-froid sur la crédibilité de la dette française et de la signature française, ensuite je vous rejoins à 1000%. Bien sûr que nous devons avoir une stratégie cohérente, stable, déterminé de rétablissement des finances publiques elles passent tout de suite par 3 décisions immédiates. La revue des dépenses publiques qui a été engagé par la Première ministre et qui aura lieu, je tiens à le dire, pas l'année 2023 mais toutes les années, à partir de l'année 2023, ce qui veut dire que chacune des dépenses publiques, sera examiné pour vérifier que véritablement elle remplit le service que nos compatriotes sont en droit d'attendre. 2ème rendez-vous les assises des finances publiques pour nous engager sur la trajectoire que j'ai indiqué troisième rendez-vous de la loi de programmation des finances publiques qui gravas dans le marbre la trajectoire financière de la France et l'accélération du désendettement qui est marqué dans le programme de stabilité 4 points de désendettement supérieure à ce que nous avions envisagé. que tous ceux qui ici croit dans la nécessité d'avoir des finances publiques bien tenues nous rejoignent dans sa détermination à accélérer le désendettement de la France. La parole est maintenant. Aux. Jean-François Husson, rapporteur général pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Ministre des Finances dans une France en proie malheureusement à des tensions sociales persistantes. La récente dégradation de la note de la France à double A négatif par une agence de notation confirme, s'il en était besoin nos inquiétudes au regard de l'incapacité à réduire notre endettement qui atteint des sommets. On pourrait et, bien sûr, espérer bénéficier d'une croissance soutenue. Mais les prévisions fournies par les économistes, pour la période 2023 2027 sont bien moins favorable que celle du gouvernement. Cela aura donc nécessairement des effets sur l'évolution des recettes publiques et par suite sur les déficits. Pour vous, Monsieur le Ministre confirmé que ce camouflet financier à tout le moins cette alerte adressé au gouvernement ne vous. Ne vous inspire pas d'inquiétude particulière et que nos comptes publics ne dérive pas dangereusement. Quelles conséquences enfin en tirez-vous sur l'évolution des conditions de financement de la France et sur l'évolution de la charge de la dette. Oui monsieur le le sénateur Husson, là aussi je connais votre engagement sur le sujet des finances publiques. Je ne suis pas là pour être inquiet, je suis là pour être déterminée. Et déterminé dans le rétablissement des finances publiques avec des décisions très structurante qui d'ailleurs ont été votées pour certaines à votre groupe dont je salue l'esprit de responsabilité. Les premières décisions structurantes. Ça a été la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites que vous avez voté et dont je rappelle que Fitch contrairement à ce que j'entends dire trop souvent a salué l'efficacité pour le rétablissement des finances publiques, la 2ème décision très concrète. Vous savez que la sortie du bouclier tarifaire. La fin du gel sur les prix du gaz puisque les prix du gaz sont revenues à la normale et la sortie progressive du plafonnement sur les prix d'électricité. Nous voulons que d'ici la fin 2024 début 2025, nous soyons sortis définitivement et totalement des boucliers tarifaires qui était utile pour protéger nos compatriotes quand c'était nécessaire, mais qui ne sont plus utiles, dès lors que les prix reviennent à la baisse. J'espère que vous nous soutiendrez aussi dans cette décision, enfin 3ème, remarque la loi de programmation des finances publiques. Une fois encore, j'en ai parlé à plusieurs à plusieurs reprises avec le président de votre groupe, je reste ouvert à toute amélioration qui permettra d'adopter cette loi de programmation des finances publiques et de graver dans le marbre cet engagement. Pourquoi c'est important. Mais pas pour faire plaisir aux agences de notation. Mais une fois encore pour rétablir totalement et pleinement notre indépendance et notre souveraineté financière et tout simplement aussi parce qu'en période d'augmentation des taux d'intérêt laisser filer la dette, comme le proposent certains, c'est jeter l'argent par les fenêtre 1 point de taux d'intérêt supplémentaire c'est horizon 2027 15 milliards d'euros de charges supplémentaires sur la charge de la dette. C'est plus que le budget du garde des Sceaux, je pense que le garde des Sceaux et surtout tous nos compatriotes préfèrent qu'on dépense de l'argent pour les policiers pour la sécurité pour les gendarmes pour la justice pour l'école pour l'hôpital pour les services publics plutôt que pour le service de la dette. C'est pour cela que vous pouvez compter monsieur le sénateur sur ma détermination totale à rétablir les finances publiques et accélérer le désendettement. Monsieur rapporteur général. Oui, vous dites, Monsieur le Ministre, déterminer si j'en juge par les 6 années qui sont passées et le résultat qui est celui qu'on constate aujourd'hui au moins je fais un constat, c'est que vous avez singulièrement manqué de détermination. 2ème élément qui me paraît. Inquiétant puisque je, je suis également inquiet. Ce sont les chiffres qui sont dans le programme de stabilité que nous allons examiner ce soir que nous avons mis à Bruxelles où je dois vous dire que les dépenses par rapport à la loi de programmation que nous avons étudié à la fin de l'année en décembre. Elles ont augmenté de 30 milliards d'euros. Dérive supplémentaire. Alors Monsieur le Ministre, oui nous sommes déterminés et nous sommes déterminés pour un temps de vérité et non pas pour du camouflage, parce que ce, ce qui est en train de se passer, vous nous demandez de travailler sur la loi de programmation des finances publiques. Mais alors pourquoi avez-vous continuer à dépenser de l'argent que nous n'avons pas qu'il faut aller emprunter quand nous vous avons proposé. Au mois de décembre des pistes d'économies. Vous avez balayé d'art vers demain. C'est regrettable. Donc je vais vous dire comme je l'ai dit il y a pas très longtemps. Monsieur le ministre, il faut vraiment se mettre au travail. La parole est à votre collègue Nicole Bonnefoy, pour le groupe socialiste écologiste. Thierry Philippe. Merci monsieur le président. Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues. On ne compte plus les fermetures temporaires de services d'urgence ou hospitaliers aux 4 coins du pays. Le Sénat par sa connaissance du quotidien de nos compatriotes vous interpelle depuis des mois. Oh j'oserais-je même dire depuis des années sur la désertification médicale à l'oeuvre qui se déporte à présent vers l'hôpital et les urgences je vous questionner moi même encore récemment sur le risque de fermeture de l'hôpital de Ruffec ou de Confolens. Dans mon département en Charente. C'est ainsi en cascade, qu'arrivent les nouvelles fermetures de services que par euphémisme. Vous appelez suspension temporaire pas un territoire bien souvent rurales n'est épargné par l'avalanche de défections de médecins épuisés par la charge de travail de nuit comme de jour, les maternités ferme en pagaille, par manque de médecins et mettent en danger la vie des femmes. Monsieur le Ministre, je vous prie d'écouter les territoires. Attention à ne pas considérer un service fermé comme un service désengorger. À ce stade, la promesse d'Emmanuel Macron d'améliorer l'offre de soin d'ici la fin de l'année est un mirage. Vous devez ce mercredi faire un 1er bilan du CNR santé. Nous avons eu ce matin un aperçu peu convaincant sur France Inter de votre boîte à outils. La situation n'est pas acceptable, vous le savez et les Français comme les élus locaux ont besoin de clarté sur les données du ministère en matière de fermeture le recours massif aux 15 est-il l'Alpha et l'oméga de vos moyens d'action. L'urgence des urgences. Monsieur le Ministre, c'est l'accès à la santé et non les retraites où sont vos propositions de régulation de l'accès aux soins, où est votre vision de moyen terme pour assurer la continuité du service public de santé. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les les sénateurs, madame la sénatrice bonne foi. Ce qui serait surtout un mirage, c'est de vouloir faire croire aux Français que nous pourrons demain à voir 5000 ou 10.000 médecins de plus ce n'est pas vrai, il faut le dire et c'est bien notre organisation globale qui doit être repensée Dans ce cette réorganisation. Nous sommes en train nous tous ensemble de gagner le combat contre les dérives de l'intérim médical. Je dis nous parce que c'est le gouvernement sous l'autorité de la Première ministre. Les professionnels de santé et les élus, territoire par territoire qui nous permettent de gagner ce combat indispensable pour la survie de notre hôpital public. Cette dérive de l'intérim médical amenait la fuite des médecins hospitaliers, de l'hôpital public, Qu'elles ont été les solutions mises en place et y compris dans votre département de Charente et et pour l'hôpital de de Confolens qui assure réouvrir entre guillemets son service des urgences. Eh bien c'est la solidarité territoriale qui est porté par les ARS. C'est la possibilité de travailler de façon plus intelligente à l'échelle d'un territoire pour que les parcours de soins ne soit pas interrompu ne soit pas rompu et qu'on continue à garantir la sécurité et la qualité des soins pour nous tous nos concitoyens. D'une façon plus structurelle et pour répondent au à l'engagement du président de la République sur les services d'urgence. Bien entendu, un service d'urgence de fermer, n'est pas un service d'urgence désengorger ça semble une évidence, mais par contre nous avons les outils pour aboutir à ce désengorgement ça passe d'abord par une meilleure gestion de de la Manche. Je dois rappeler que le sas dont vous parlez, qui est une des solutions c'est la première fois que l'été dernier, grâce à la mise en application du numéro 15 et en demandant à nos concitoyens d'appeler le SAMU, que nous avons pu faire diminuer la fréquentation de nos services d'urgence, et cela perdure dans les départements qui ont mis en place ce ça s'il y a également d'autres solutions. L'aval des urgences la gestion des lits là aussi à l'échelle territoriale avec le public et avec le privé et puis enfin quelques éléments de réorganisation de nos services pour qu'ils soient plus fluide. Mirage comme vous dites n'est loin d'être inatteignable et là aussi nous l'atteindrons territoire par territoire, et tous ensemble. Je vous remercie. Ah la bonne foi. Oui j'ai le regret de de vous dire Monsieur le Ministre que avec le gouvernement. Vous gérez la crise de l'hôpital. À la petite semaine, sans vision d'ensemble, sans mesurer les conséquences de vos propres lois, comme celle sur l'intérim vous éradiquer la médecine de proximité et vous condamnez des territoires entiers à la rupture de soins. La parole est à notre collègue. Dominique Estrosi Sassone pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à Madame, la Première ministre. Les titres de presse se sont multipliées ces derniers jours pour parler de bombe sociale de catastrophe des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour alerter sur les dangers de cette crise du logement qui cause une fatigue quotidienne pour tous les personnes qui sont obligés d'habitude d'habiter loin de leur lieu de travail, qui crée une angoisse pour toutes celles qui arrive à la fin de leur vie active sans possibilité d'acheter un toi qui provoque la colère de ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas habiter dans leur région près de leur famille victime de prix dissuasif 100.000 mal logés de plus 10% de personnes à la rue de plus 100.000 demandeurs de logements sociaux de plus que l'année dernière hausse des taux d'intérêt constructions neuves en berne gigantesque chantier de la rénovation énergétique. Marché de la location grippé parcours résidentiel bloqué tous les voyants sont au rouge et votre gouvernement jusqu'il y a peu encore été dans un déni total voire pire encore aux abonnés absents. Alors madame, la Première ministre. Pourquoi avoir autant négligé la politique du logement qui est au coeur de la vie quotidienne de tous les Français.

Évidemment que le logement est une priorité de ce gouvernement et nous y travaillons depuis de nombreux mois et c'est une priorité du président de la République depuis 2017. le plan logement d'abord qui a permis à 440.000 familles de quitter la rue pour obtenir un toit est un plan qui a fonctionné la lancement de ma prime Rénov'malgré les difficultés que je n'ai pas est un plan qui fonctionne plus d'un million cinq de chantier ont été réussis. Oui il y a une crise aujourd'hui du logement. Nous n'avons pas découvert au, au détour d'articles d'être. Nous y travaillons depuis plusieurs mois et, et le mot bombe sociale est un mot que j'ai employé moi-même dès le mois de novembre dernier. Parce que cette crise d'où nous la pressentions elle n'est pas le fait du précédent gouvernement et l'effet d'une politique du logement insuffisantes depuis de nombreuses années et et nous allons-y répond nous allons-y répondre comme madame, la Première ministre, il a dit dans sa feuille de route avec un certain nombre d'initiatives immédiates, une action avec la Caisse des dépôts comme elle avait déjà été ne me mener à la fin de la crise Covid d'acquisition de logement pour sortir un certain nombre de projets qui sont aujourd'hui bloqués notre priorité, c'est de loger tous les Français de manière digne et abordable. Donc et des et des, la promotion immobilière cédée toute la filière de la, de l'habitat et à la fois l'habitat privé mais aussi l'habitat social et nous le ferons, nous travaillons avec. Le le ministre. De l'Économie et des Finances avec les banques pour à faciliter l'accès au crédit car vous le savez aujourd'hui avec l'augmentation des taux l'accès au crédit et est difficile et avec Bruno Lemaire, nous y travaillons et Christophe Béchu. Nous y travaillons d'arrache-pied. Enfin comme la Première ministre, il a annoncé, nous travaillons au maintien. Du PTZ, qui est un moyen pour nos concitoyens d'accéder au logement d'avoir. Une possibilité d'avoir un apport personnel puisque le PTZ est souvent considéré de la sorte. Et je peux vous assurer et vous y êtes invités lors du Conseil national de refondation du logement qui sera présenté le 9 mec. Nous continuerons à travailler tous ensemble à l'union sacrée du logement. Madame Estrosi Sassone. Monsieur le Ministre, madame la la Première ministre, effectivement je pense que vous avez dressé une fois de plus un constat aborder avec quelques mesures conjoncturelles dans la feuille de route des 100 jours de madame, la Première ministre. On parle simplement de faciliter l'accès au logement et de favoriser le mieux-vivre mais on a besoin. Au-delà des réformes et de problème conjoncturel d'apporter des remèdes à des problèmes structurels. Il faut une véritable remise à plat de la politique du logement, ainsi qu'un inventaire de la réglementation. C'est du bon sens mais aussi de l'urgence parce que sinon cette crise du logement derrière elle se profile une crise sociale une crise sociétale hautement inflammable dans un pays qui est déjà à fleur de peau. La parole est au président. Jean-François Longeot pour le groupe de l'Union centriste. La parole. Ma question à laquelle ça se lit j'associe mon excellent collègue Philippe Tabarot s'adresse à monsieur le ministre des Transports. Monsieur le ministre. Le conseil d'orientation des infrastructures a remis son rapport à la Première ministre il y a plus de 2 mois. Les principales annonces du gouvernement sont conformes à ce que la commission d'aménagement du territoire et du développement durable préconisait. Un effort massif sur le ferroviaire, 100 milliards d'euros à l'horizon 2040, dont la moitié sur le réseau. Le lancement des CPER très attendu par les élus et un mandat donné à la Société du Grand Paris pour instruire les projets de RER métropolitains. L'annonce de ce plan suscite néanmoins plusieurs interrogations. La régénération du réseau est effectivement urgente. L'âge moyen de ce dernier de 30 ans en France contre 17 chez nos voisins allemands. Il nous faudra donc dans les prochaines années stabiliser et l'âge moyen de ces derniers, avant de le faire redescendre, via une augmentation des opérations de régénération. La décarbonation des transports nécessitera un report modal massif de véhicules individuels vers le train. La stratégie annoncée par le président de la République de développer des réseaux de RER métropolitains et la bonne ces derniers permettront à l'échelle du pays, de supprimer des millions de trajets en voiture et d'offrir aux habitants des grandes métropoles des réseaux de transport en commun performant qui ne seront plus l'apanage de la seule région parisienne, à titre personnel, je me réjouis du mandat donné à la Société du Grand Paris, d'instruire les projets de RER métropolitains en combinant son expertise avec celle de la SNCF réseau je crois que la France a tous les atouts permettant de mener à bien cette grande entreprise. Monsieur le Ministre, pourriez-vous préciser la position du gouvernement sur ce texte est partagé à la représentation nationale les projets du gouvernement en matière de RER des développements. Plus largement, je souhaite vous interroger, Monsieur le Ministre, sur les modalités de financement du CO. Oui, ma question est simple, quelles sont les méthodes de financement 20 envisagée par le gouvernement. Je vous remercie. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Longeau le 10 mars dernier, la Première ministre a en effet présenté un ambitieux plan d'avenir pour les transports qui doit beaucoup aux travaux et aux priorités de votre commission et aux travaux qu'a porté au sein du conseil d'orientation des infrastructures notamment votre excellent collègue Philippe Tabarot en effet. Nous aurons l'occasion de discuter de ces Budgets quelques orientations en réponse aux questions que vous soulignez, d'abord la priorité que nous partageons que j'ai indiqué dans cet hémicycle à plusieurs reprises au réseau ferroviaire, nous avons en effet malgré les réinvestissements récent réseau ferroviaire. bien plus vieux que le réseau ferroviaire de nos voisins allemands et nos principaux voisins européens, nous allons la Première ministre a indiqué augmenter progressivement d'ici la fin de législature de 50 pour %, cela n'a jamais été fait de 50% les crédits annuels investis dans le réseau ferroviaire français. C'est la condition pour restaurer un certain nombre de lignes parfois sinistrés. Qui traverse notre territoire Bordeaux Marseille Paris Limoges Paris-Clermont-Ferrand ou dont vous connaissez la vétusté la nécessité du réinvestissement. C'est aussi une priorité donnée au service Express métropolitain qui je le rappelle, ne sont pas des projets au service des centre-ville mais des projets qui vise à développer une alternative à la voiture individuelle dans les périphéries à 30 40 50 80 kilomètres des centre-ville, et la proposition de loi présentée à l'Assemblée nationale par le président Zulesi. Pour être très clair, nous la soutiendrons nous la soutiendrons parce qu'elle met en oeuvre l'outil juridique notamment par l'évolution du statut de la Société du Grand Paris qui permettra de créer pour les collectivités qui le souhaitent, les sociétés de projets qui porteront la mise en oeuvre de ces projets. Il faut financer en effet cet effort important, c'est 100 milliards d'euros collectivement avec les collectivités locales dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques des crédits qui se déploieront les années qui suivent et il faudra aussi mettre à contribution la Première ministre a indiqué d'autres secteurs et d'autres modes de transport, le secteur des routes. Les sociétés autoroutières, en particulier le secteur aérien, nous le ferons en débattant ici même lors des prochains Budgets et puis je veux insister sur un projet qui tient à coeur au Sénat en particulier, c'est la question du Lyon-Turin. Nous avons bien sûr cette priorité à coeur j'aurai l'occasion d'échanger avec le prendre région Auvergne Auvergne-Rhône-Alpes dans quelques jours parce que nous devons porter cet effort budgétaire l'État s'y engage mais nous aurons besoin d'être soutenus et accompagnés. Je vous remercie. Monsieur le Président Madame la Ministre j'ai participé la semaine dernière. La conférence nationale du handicap, réunion à laquelle d'ailleurs je représenter notre président du Sénat. Cette 6ème édition de la CNH s'est tenu dans des circonstances particulières. Alors que ces conférences ont été jusqu'à présent des moments de partage d'objectifs avec les acteurs du monde du handicap. Cela n'a pas été le cas cette année. Après avoir fait connaître leur insatisfaction en amont et demander un report de plusieurs semaines en fin d'engager un viré un véritable travail de concertation, de nombreuses associations dont le Collectif handicap n'ont pas participé à cette CNH. Cette situation est dommageable, d'autant qu'un consensus pouvait être trouvé au regard des thématiques de travail retenus. Au cours de cette CNH le prends de la République a énuméré un certain nombre de propositions concernant l'accessibilité, la scolarisation, l'emploi, l'accès aux soins et nous ne pouvons que saluer un certain nombre de mesures, je pense notamment, ou 1,5 milliards d'euros annoncés pour l'accessibilité le remboursement à 100% des fauteuils roulants ou la création de 50.000 solutions en établissements et dans les services sur 5 ans. Mais en écoutant le discours du prendre public les 70 engagement et de nombreuses mesures afférentes. Nous nous posons tous cette question comment financer ce programme qui se chiffre à plus de 4 milliards d'euros. Je vous remercie pour votre réponse. Pour vous répondre. La parole est à la ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Vous avez la parole. Merci monsieur le président, mesdames les sénatrices. Monsieur le. Le sénateur Moulier. D'abord je vous remercie pour cette question qui permet de mettre le focus sur cette conférence nationale du handicap qui était un moment important pour le monde du handicap pour les personnes handicapées pour les associations pour les familles qui était un, un moment attendu, vous l'avez dit ou certaines associations ont grincé un petit peu des dents sans que je comprenne véritablement quel était le sujet parce que la préparation de cette conférence nationale du handicap. Ça a été 8 groupes de travail 40 réunions 500 personnes mobilisées. Beaucoup de contributions écrites que nous avons intégré à la réflexion. En fait c'est une vraie co-construction qui a été réalisé avec des comités de pilotage également qui ont donné les conclusions au fur et à mesure de l'évolution des travaux donc cette mauvaise humeur. Moi je la prends pour ce qu'elle est. Je constate quand même que la majorité des associations de ce collectif handicap était présente. Lors de cette CNH et je crois que les associations sont exigeantes et qu'elles ont raison d'être exigeante. Parce que elle elle souhaite simplement que les handicapés et les personnes handicapées accède pleinement à leurs droits et accéder pleinement à leurs droits notamment par exemple sur les sujets d'accessibilité dont vous avez parlé, du président de la République, c'est un milliard 5 sur l'accessibilité des fonds pour les collectivités afin qu'elles accélèrent leurs programmes d'accessibilité et des fonds pour les petits propriétaires ou pour les les commerces du quotidien et les cabinets médicaux par exemple afin qu'ils accélèrent cette. Cette mise en accessibilité. Eh bien nous sommes très en retard et je crois que cette déclaration, cette volonté de mettre notre pays en marche vers une accessibilité totale hé bien fera plaisir aux associations et fera en sorte bien qu'elles reviendront toujours dans la co-construction que nous avons réalisé pour cette CNH et je n'ai pas le temps de répondre à votre autre question mais un, un investissement pluriannuel est prévue et bien sûr, tout cela sera mis à disposition. Du Sénat est à votre disposition compte tous les tableaux d'investissement pluriannuel seront établies.

qui est importante. Concernant le financement. Les sommes sont élevés. Vous avez dit, l'objectif est aussi à un et visite élevé mais ici où ça nous serons vigilants sur 2 choses, d'abord au moment du PLF et du PLFSS 2024 nous serons vigilants pour voir la traduction des engagements du président de la République dans les comptes qui nous seront proposés mais surtout nous serons vigilants qu'il n'ait pas de transfert de charges sur les collectivités car le principe à la fois de l'utilisation de la DETR d'être de la difficile de ne pas être transférés sur le fond de l'incivilité et les départements également ont également de vigilance sur le les politiques médico-social. Le grand principe quand l'État s'engage l'État épais. La parole est notre collègue Jean-Jacques Michaux. Pour le groupe socialiste, écologiste, RFI. Dans ce contexte, plus de 2 millions de personnes seront effectivement affectés par l'extinction des tarifs réglementés du gaz prévue le 30 juin et en vérité, plus de 7 millions de ménages si on tient compte de ceux qui ont basculé en offrent de marché mais dans les contrats sont indexés sur le tarif réglementé. Certes, vous avez annoncé la prolongation du bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année. Mais si la volatilité à la hausse des prix énergétiques demeure face aux dysfonctionnements du marché de l'énergie, la perte de la maîtrise publique tarifaire garantis par des tarifs réglementés auquel se raccrochent le bouclier tarifaire est évidente. Qu'adviendra-t-il alors pour les consommateurs. En 2024, il y a là une grande inconnue et à tu vois mesure d'assurer que le basculement sur l'offre passerelles ou d'autres contrats n'est pas d'incidence sur les tarifs à court ou moyen terme car de toute évidence la piste évoquée par le gouvernement, visant à mettre en place un prix de référence déterminé par la Commission de régulation de l'énergie qui servirait de base à la poursuite du bouclier tarifaire n'offre aucune garantie, et sûrement pas celle de tarif réglementé qui étaient fixé par les pouvoirs publics, on le voit bien, le débat n'est pas nouveau, il resurgit aujourd'hui quelle est notre capacité à retrouver une maîtrise publique tarifaires sur les biens de première nécessité que sans l'électricité ou le gaz. Alors Madame la Ministre voici ma question, alors que l'inflation et les dérèglements du marché sont toujours en action. Entendez-vous reporter la fin des tarifs réglementés et plus largement au delà des dispositifs conjoncturel par ailleurs bienvenue. Quelles sont les mesures que le gouvernement prend au sein de l'Union européenne pour que le prix du gaz et, en conséquence de l'électricité n'atteignent pas des niveaux exorbitants 5 convenu ne sans commune mesure avec les coûts de production de l'électricité dans notre pays. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Michaud merci pour cette question qui va me permettre de rassurer ceux qui nous écoutent. Tout d'abord et je pense que c'est important de le préciser et peut-être contrairement à ce que vous laissez entendre le tarif réglementé du gaz est un tarif de marché c'est un tarif qui évolue chaque mois sur la base d'une formule et qui a augmenté de 200% entre octobre 2021 et octobre 2022. Et vous l'avez bien compris, c'est pas ça qui protège les Français. Vous l'avez d'ailleurs mentionné ce qui protègent les Français c'est c'est le bouclier énergétique quand les prix du gaz se sont affolés, comme l'année dernière et le ministre de l'économie le disait un instant ses tarifs de ce ce prix du gaz est désormais rerentrer grossièrement dans l'ordre. Ce bouclier, il sera prolongé jusqu'à la fin de l'année. Il concerne tous les ménages qui se chauffent et qui cuisine au gaz qu'ils soient au TRV gaz ou pas. Alors qu'est ce que change. Cette évolution du TRV gaz. Vous savez que c'est une décision de justice qui a. Tenu à supprimer cette référence et donc nous accompagnons les Français et au fond ça va pas changer grand chose pour les Français, les 2 millions de Français qui aujourd'hui. Ont un contrat sur la base du TRV gaz. Pourquoi. Soit ils font le choix de conclure un contrat avec un fournisseur de gaz qui leur convient. Soit ils ne font rien et automatiquement, ils bénéficieront de leur fournisseur de gaz, un contrat qui sera effectivement sur la base d'un tarif qui est calculé par l'creux, c'est au fond exactement la même chose que par le passé sauf que au lieu d'imposer à Engie de suivre ce tarif Engie s'engage à suivre ce tarif, il n'y aura évidemment aucun coup de changement de contrat, aucun changement de compteur, cela se fait automatiquement et je veux dire ici. Je crois que la Première ministre de l'art l'a répété à de nombreuses reprises. Aucun pays n'a comme ce gouvernement autant protéger les Français contre l'évolution des coûts de l'électricité et du gaz et vous pouvez compter sur nous pour continuer à accompagner les Français. Ces tensions. La parole est à notre collègue Muriel Jourda pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, mes chers collègues, ma question et pour Monsieur le le ministre de l'Intérieur et je voulais à mon tour évoquer les les violences d'une brutalité inouïe et dont les forces de l'ordre ont fait l'objet lors des manifestations du 1er mai dernier chacun je crois à garder en tête l'image de de ce policier en feu qui. Je l'espère, je le pense, a ému et horrifié la quasi-totalité des Français et il s'agissait d'un policier parmi les plus de 400 membres des forces de l'ordre qui ont été blessés à cette occasion et et vers lesquelles vont tous nos voeux de rétablissement à cette occasion, Monsieur le Ministre, vous avez déclaré que ces violences étaient inacceptables. Vous l'avez déclaré le jour même où vous l'a déclaré le lendemain lors de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Vous l'aviez dans des conditions similaires. Déclaré le 25 mars 2023 à Sainte-, Soline le 23 mars 2023 à Lorient le 29 octobre 2022 dans les Deux-Sèvres, le 1er mai 2022, déjà à Paris le 14 avril 2022 à Rennes, le 20 mars 2021 Verdun j'arrête là parce que je ne pourrais pas remonter jusqu'à la date de votre entrée en fonctions qui était au mois de juillet 2020. Je n'en ai pas le temps. Ces violences sont inacceptables. Nous en sommes d'accord et nous pouvons être à vos côtés pour vous le dire. Et après, que faisons-nous. Ou plutôt, que faites-vous. Merci monsieur le le président, madame la sénatrice. Merci de soutien des policiers, des gendarmes je j'applique la loi de la République, madame la sénatrice, c'est-à-dire la loi votée par deux chambres et d'ailleurs. Je suis tout à fait dans le regret de vous dire que le gouvernement était à l'écoute de la proposition de loi de monsieur Retailleau. Qui a été adopté par la haute comme la Basse. Assemblée et, pour autant, cela a été censurée par le Conseil constitutionnel si vous attendez du ministre de l'Intérieur qui outrepasse ses lois de la République pour appliquer sa loi personnelle. Nous ne serions pas en démocratie. Donc la question que je vous pose madame la sénatrice. La question, je veux ça c'est. Que proposez-vous. Le gouvernement a fait des propositions. Le gouvernement a fait des propositions mais le après-ministre a répété. Une question de monsieur le Président Maluret. Le garde des sceaux l'a dit ce matin à une chaîne de grande écoute. Nous sommes favorables à remettre l'ouvrage sur le métier d'une proposition de loi d'un projet de loi, qu'importe le père du moment qu'le portent des beaux enfants, Madame la sénatrice, pour que nous luttions contre ces casseurs qui non seulement attaque et veulent tuer des policiers, des gendarmes mais empêche les manifestants de manifester. Je vous renvoie d'ailleurs à ce titre et je dis pour le groupe du Parti communiste que je salue ici au communiqué du parti communiste français qui évoquait ce que les blacks blocs ont agressé des élus et des membres du Parti communiste et je me réjouis que le parti communiste comme la plupart des grands partis républicains se sont même position que vous. On peut donc se retrouver pour que nous puissions avoir l'équivalent de ce que nous avons dans les stades de football que des hooligans n'avait pu dans des stades pour aller voir des matchs de football parce qu'on a pas voir un match de football avec des cocktails Molotov dans la poche, on ne va pas dans des manifestations, avec des cocktails moto. Dans la poche et quand on est très connu des services de police et très violent. Le ministre de l'Intérieur et comme vous il aimerait pouvoir leur interdire à aller dans des manifestations. Simplement, la loi Madame. La sénatrice. Vous l'aurez constaté, et j'ai pas loin de la commission des lois ne permet pas au ministre de l'Intérieur donc votons ensemble un texte qui permettra d'être au rendez-vous de ce rendez-vous. Madame Jourdain. Je vous remercie monsieur le ministre de rappeler que effectivement le dernière loi qui a voulu agir sur le sujet émanait du groupe les républicains au Sénat, et peut-être n'aurait-elle pas été censurée par le Conseil constitutionnel si nous l'avions voté telle quel et non pas modifié par votre prédécesseur. Mais la réalité c'est que je ne souhaite pas polémiquer sur ces sujets. Je souhaite juste que nous prenions ensemble la mesure de l'enjeu qui est celui de ces violences. L'enjeu c'est l'état de droit. L'État de droit, c'est la fin de la loi du plus fort. C'est une loi qui est votée par le Parlement qui est appliqué par une justice efficace et qui est respecté, parce que les forces de l'ordre ont elles aussi respecter. Or le Parlement. Il est mise à mal et sa légitimité est mise à mal par tous les conventions citoyennes que vous décidez, la justice elle est considérée comme si peu efficace par nos citoyens que les exemples de justice se multiplient dans le pays et les forces de l'ordre et bien ces 2 derniers pans qu'ici il va, elle va vacille est bien feront vaciller aussi les doigts de droits. L'état de droit. Alors, agissez. Et tu as d'autres collègues. Nathalie Goulet, pour le groupe de l'Union centriste. Oui, monsieur le président, mesdames, messieurs le visites, mes chers collègues, je voudrais d'abord à ce moment précis assuré au nom de mon groupe. Le soutien évidemment aux forces de police, de gendarmerie et aux forces de maintien de la paix. J'ai une, une question pour le ministre de l'Intérieur qui pourrait paraître anecdotique, mais enfin c'est peut-être un détail pour vous mais peu Nour ça pour nous ça veut dire beaucoup. Il s'agit de la les 40 pages de circulaire. Pour l'élection des grands électeurs aux élections sénatoriales. En effet, d'abord il faut saluer la date du 9 juin qui est une date assez proche d'habitude on avait les listes électorales beaucoup plus tardivement. Donc je vais d'abord vous remercier, mais en plus vous indiquer la clé, l'inquiétude d'un certain nombre d'élus quant à la complexité de cette circulaire, notamment en ce qui concerne les communes nouvelles pour lesquels il n'y a pas pas beaucoup d'indications ou plus exactement trop d'indications pour que ce soit vraiment claire, sans que les préfets puissent nous donner à l'heure actuelle, le nombre exact de grands électeurs pour les comme une nouvelle comme je l'ai dit c'est peut-être un détail pour vous mais pas pour les sénateurs renouvelables par ailleurs la date du 9 juin pose aussi un problème car c'est une date fixe et il y a un certain nombre d'élus qui ne pourront pas être et cette date et pose pose problème car elle est aussi la date du congrès de la fédération des centres de gestion de la fonction publique territoriale qui se passe à Ajaccio et qui va devoir évidemment comprendre un certain nombre d'élus. Donc Monsieur le Ministre, je voulais vous poser la question, que pensez-vous faire pour simplifier les dispositifs qui sont actuellement en place. Oui, bonjour madame la sénatrice. Monsieur le Président ce les les sénateurs, madame la sénatrice. Je suis un peu étonné de votre question parce que d'abord si l'élu n'est pas là c'est pas à vous que je pense qu'il peut faire une procuration malheureusement puisque les élections s'adresse sont convoqués pour le mois de septembre. On n'a pas convoqué les conseils municipaux en juillet et en août qu'il me semble que les sénateurs aient envie de parler également aux électeurs qui ne connaissent pas encore, c'est-à-dire ceux désignés

on prévient je crois assez tôt. Je crois qu'on a prévenu 2 mois avant la date pour les l'ensemble des des des maires pour convoquer ses conseils municipaux et il est prévu d'ailleurs que si le quorum n'est pas atteint. Parce que là nous parlons bien des conseils municipaux qui désigne des électeurs. Donc il s'agit de quand même de villes en général. Plutôt conséquente, on va dire cela comme ça en tout cas qui désigne des grands électeurs. S'il n'y a pas de quorum. Ils peuvent convoquer un conseil municipal, là franchement, je crois même. Que sur la question de, de la date, vous avez largement la possibilité de convoquer ses conseils municipaux sur la question des des villes nouvelles, vous avez raison, il y a une multiplicité de villes nouvelles, et notamment des villes nouvelles qui sont de taille de plus en plus importante et ces villes nouvelles refont faire le calcul puisque ce n'est pas le cas dans les précédentes élections sénatoriales du nombre de grands électeurs chaque préfet. Je suis étonné mais je me je me renseigner dès cet après-midi auprès de votre préfet le département s'il n'a pas si vous l'expliquer. On va donc re-expliqué monsieur le préfet département que peut être il s'est mal exprimé envers vous. Chaque préfet connaît le nombre de grands électeurs qui sont disponibles si j'ose dire, dans les villes qui ne désigne des grands acteurs, à Tourcoing je connais déjà les grands électeurs que mon conseil municipal pourra désigner pour la grande le grand plaisir des sénateurs du Nord qui se présentent aux suffrages des grands électeurs de de tours Donc nous pouvons si vous le souhaitez, madame la sénatrice. Refaire passer un message aux préfets, mais je crois que ceci désormais ont tous les moyens pour pouvoir désigner les grands électeurs pour qu'elles sont cette âge se tiennent le mieux possible.

dont je vous ai annoncé que c'était évidemment un, un sujet qui était évidemment pas majeur par rapport à tous les sujets que vous avez à traiter, et vous avez traité aujourd'hui mais il faut quand même le le traité, c'était Monsieur le Ministre, par rapport à une circulaire de 40 pages envisager une différenciation entre les départements qui avaient conclure un scrutin de liste Je vais donner la parole à notre collègue Hechter Benbassa pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre. Olivier Dussopt, Monsieur le Ministre, attendez-vous comme le président de la République, que les Français se lassent ou prennent peur. Violences et blessés de part et d'autre ne se comptent plus. Cela permet de remettre la sécurité au centre, protéger les Français et certes un devoir n'il en est autre que vous oubliez toujours les entendent et leur répondent. C'est pourtant simple, ils ne veulent pas travailler 2 ans de plus. Mais leur colère à d'autres raisons encore plus profonde plus ancienne je connais les gilets jaunes pour les avoir longtemps côtoyé dans les rues de Paris. Or ils sont là avec les autres. Syndiqués ou pas, jeunes et vieux, le dépit en bandoulière. La rancune de leurs blessés déjà oublié dans la tête tous avec ou sans gilet ont une seule exigence, vive le mieux or vivent le mieux c'est aussi partir à la retraite à un âge qui permettent d'en profiter vraiment et plus longtemps mais vivre mieux c'est aussi être traités autrement par ceux qui vous gouvernent monsieur Macron peut se promènent. Dans nos régions si lui, si le gouvernement ne change pas. La colère ne retombera pas suffit-il de dire dans un tweet. Merci aux travailleurs pour se rapprocher de la Ve République est à l'agonie votre exercice ultra verticale du pouvoir la tu le RN lui vous remercie Monsieur le Ministre, quand admettrez-vous qu'il faut négocier et que négocier quand la colère est si grande. C'est aussi savoir céder quand céderait vous sur un texte inutile et injuste CD n'est pas forcément perdre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Benbassa. Vous dites madame la sénatrice qu'il faut négocier, qu'il faut discuter. La réforme des retraites sur laquelle vous revenez a fait l'objet d'une concertation de quatre mois, qui n'a pas permis trancher tous les différents, nous le savons mais 4 mois elle a fait l'objet d'un débat parlementaire, ici même, c'est une centaine d'heures de débat et à la fin, un texte qui a été adopté avec une large majorité du Sénat une première fois, une seconde fois en commission mixte paritaire à nouveau dans l'hémicycle ce texte il est légitime et il a été adopté de manière démocratique. Vous dites il faut négocier, il faut continuer à discuter, c'est une réalité, c'est ce que nous allons faire, nous allons faire puisque le président de la République l'a dit la première miss là dit aussi il a un certain nombre de sujets qui relèvent de l'agenda social sur les conditions de travail sur l'emploi des seniors sur le déroulement des carrières qui à nos yeux relève très directement la négociation entre les partenaires sociaux il y a des sujets qui ont déjà fait l'objet de négociations, le partage de la valeur. Notamment et nous allons transposer de manière fidèle et intégrale l'intégralité de de l'accord passé par 4 des 5 organisations syndicales et 3 organisations professionnelles. Il y a des sujets sur lesquels nous allons continuer à ouvrir des discussions et les sujets qui, par la loi de réforme des retraites relève du dialogue social, je pense notamment. À la nécessité même l'obligation désormais pour les branches professionnelles de négocier des accords de prévention de l'usure professionnelle qui permettront aussi d'améliorer les conditions de travail des des hommes et et vous dites madame la sénatrice dans votre question, qu'il y a des manifestations qui sont violentes, qu'il y a des blessés et qu'il y a finalement une forme. De grande violence du débat public et de ces troubles, je note 2 choses, madame la sénatrice. La première c'est que j'ai en tête des images de vous-même manifestants il y a quelques mois et parodiant le passage à tabac du président de la République, en donnant des coups sur une effigie à son image. J'ai aussi en tête la question, vous venez de poser, Il y a deux minutes, pas une fois, madame la sénatrice, pas une fois vous avez apportez votre soutien aux forces de l'ordre qui sont mis à dure épreuve et par vos encouragements aux désordres par vos encouragements aux bouleversement par vos encouragements aux actes qui relèvent d'une forme d'outrance, c'est vous madame la sénatrice qu'est un marchepied pour le Front national.

Je vais suspendre la séance qu'elle sera reprise à 16h 30 pour l'examen de la proposition de loi visant à renforcer l'accessibilité et l'inclusion bancaire. La séance est suspendue.

La séance. Prise. Mes chers collègues par lettre en date de ce jour, la commission des finances monde au Sénat en application de l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires de lui conférer des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour une durée de 3 mois afin de mener sa mission d'information sur la création du fonds Marianne la sélection des projets et l'attribution des subventions. Le contrôle de leur exécution et les résultats obtenus au regard des objectifs du fond. La conférence des présidents examinera cette demande lors de sa réunion du mardi 9 mai prochain. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à renforcer l'accessibilité et l'inclusion bancaire présenté par messieurs Rémi Féraud Jean-Claude Tissot Patrick Kanner Rémi Cardon Mesdames Rémi Cardon Mesdames Florence Blétry ce compta Laurence Rossignol et plusieurs de leurs collègues de monde donc du groupe socialiste, écologiste et républicain. Dans la discussion générale. La parole est à monsieur Rémi Féraud, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur. Chers collègues avec Jean-Claude Tissot et le groupe socialiste, écologiste et républicain. Nous présentons aujourd'hui une proposition de loi de progrès social. Elle s'inscrit dans la lignée d'autres travaux menés au Sénat sur l'accessibilité bancaire notamment sur proposition de notre groupe. Le travail parlementaire a déjà récemment participé à l'obtention de réels progrès par exemple en matière d'accession à l'assurance emprunteur et l'examen de cette proposition intervient alors que nous sortons de la crise sanitaire, que nous sommes entrés dans une période inflationniste dont les conséquences économiques et sociales dramatiques se font sentir durement chez nos concitoyens les plus modestes. Nous souhaitons donc poursuivre le travail entrepris ici au Sénat. Cette proposition, elle intervient alors qu'en parallèle, le secteur bancaire a affiché des bénéfices record ces 2 dernières années et que la remontée des taux d'intérêt décidée par la Banque centrale européenne le conforte. Elle intervient alors que l'association de consommateurs, UFC, que choisir tire la sonnette d'alarme régulièrement sur les montants des frais bancaires appliqués en France un prélèvement. Coûte par exemple 20 euros à la personne concernée à titre comparatif, c'est 17 fois plus qu'en Allemagne et 8 fois plus qu'en Italie. Notre proposition intervient alors que le bouclier bancaire voulue par Bruno Lemaire pour l'année 2023 s'il permet de limiter à 2% la hausse des frais des globalement ne suffira pas à protéger vraiment les personnes les plus fragiles qui sont aussi celles qui se voient infliger le plus de pénalités en raison de leurs difficultés financières récurrentes. Notre proposition intervient enfin alors que le phénomène de désertification rurale en général s'intensifie dans nos territoires et que la question de l'accès aux liquidités en fait partie et en fera de plus en plus parties. C'est pourquoi notre proposition de loi vise à répondre d'une part aux enjeux de renforcement de l'égalité territoriale dans notre pays et d'autre part à améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens en situation de fragilité de fragilité financière durement touchée en ces temps d'inflation. Pour remplir ses objectifs. Notre texte repose sur deux volets, l'accessibilité bancaire alors que nombre de nos concitoyens ont aujourd'hui un rapport dégradée avec l'institution bancaire, que ce soit pour des raisons territorial, social ou l'addition des deux, l'un des objectifs principaux est ainsi d'assurer un maintien sur l'ensemble du territoire de systèmes de retraits d'argent qui permettent à toutes et tous d'effectuer ses achats de la vie quotidienne en liquide s'ils le souhaitent. Le 2ème volet et l'inclusion bancaire en apportant des modifications législatives. Qui améliore les dispositifs actuels à destination des personnes les plus fragiles car ce public fragile représente aujourd'hui une part beaucoup trop importante des recettes générées par les frais bancaires, des établissements de l'ensemble des établissements. C'est une injustice que nous devons corriger. S'agissant de l'accessibilité territoriale. Les deux premières articles de notre texte vise à inclure une composante territoriale dans la mission de service public de la Poste face à la tendance à la fermeture de distributeurs automatiques de billets et surtout face au risque bien réel que ce phénomène s'accélère, nous pensons qu'il faut agir maintenant. Il devient aujourd'hui de plus en plus difficile dans certains territoires notamment ruraux de retirer de l'argent liquide, ce qui pose des difficultés pour les achats du quotidien et nous le constatons à travers le de nombreux témoignages d'élus locaux. Nous pensons que. Les méthodes de retraits d'argent. Qui sont aujourd'hui initiée notamment chez les commerçants ne suffisent pas à répondre à cet enjeu. Certes, notre proposition pourrait paraître pour l'instant inutile puisque 99% des Français se trouverait à moins de 15 minutes en voiture d'un distributeur automatique de billets, d'après la Banque de France. Cela étant, tout le monde n'a pas de voiture, il faut compter le coût de l'essence et il faut surtout à notre envie anticiper sur la disparition programmée de distributeurs automatiques de billets, car avec la très forte diminution de la circulation d'espèces, il apparaît que nous sommes. Probablement proches d'un point de bascule. Nous cherchons donc avec notre proposition à maintenir un accès aisé et égale aux espèces sur tout le territoire avec une nouvelle mission de service public confiées à la Poste et un financement qui s'il n'est sans doute pas parfait à la vertu de ne pas reposer sur l'état et d'être et de partis équitablement entre tous les établissements bancaires. Cette logique de prévention face à la fermeture d'un trop grand nombre de distributeurs et leur mauvaise répartition sur le territoire présente donc un véritable intérêt tout comme d'ailleurs l'article 7 de notre texte, qui rend obligatoire les sanctions pécuniaires. En cas de non respect de la législation en matière de droit au compte et d'offres spécifique, le monde bancaire se dit toujours prêt à faire des efforts mais ils n'acceptent jamais aucune sanction pécuniaires automatique, il faut donc à notre avis renforcer le principe de responsabilité. S'agissant de l'accessibilité sociale nous proposons dans les articles 3 et 4 de renforcer l'information que les établissements bancaires sont dans l'obligation de fournir, d'une part et de rendre proportionnelle aux revenus les plafonds spécifiques, correspondant aux offres de crédit pour les personnes les plus fragiles. D'autre part, dans le même sens, l'article 5 de notre texte porte sur les montants de sur des et serait donc une autre façon de limiter les frais bancaires pour les personnes en fragilité financière. Car comment accepter encore aujourd'hui que ces frais bancaires viennent eux-mêmes contribué à aggraver la situation des personnes modestes qui parfois se retrouvent même pour de faibles montants en découverts et sanctionnés pour cela. Ainsi l'objectif poursuivi par l'article 6 de notre texte et de réduire le niveau à hauteur duquel les Français les plus fragiles, participent à l'ensemble des frais bancaires perçu ce qui n'est pas le cas dans la législation actuelle nous intègre Riom dans l'autre dans l'offre spécifique visé des tarifs adaptés de frais bancaires qui ont tendance aujourd'hui à entraîner les personnes dans une spirale infernale. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, nos propositions, nous semble de nature à apporter plus de protection et plus d'équité en matière de frais bancaires et nous pensons intéressant que le Sénat permettent à la législation d'avancer sur ce point. Je tiens enfin à saluer l'esprit constructif du rapporteur dans son travail préparatoire. Nous souhaitons pour notre part comme auteur de la proposition de loi travailler dans le même état d'esprit tout ce qui permettra d'améliorer l'accessibilité bancaire territoriales ou sociales nous paraît utile nous sourds donc bien sûr ouvert aux propositions de la commission, dès lors qu'elle poursuivre le même objectif. Et en espérant aussi que notre proposition puisse être ensuite adoptée par le Sénat sans être ni trop dénaturé ni trop réduite dans sa portée. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Stéphane Sautarel. Porteur de la commission des finances pour 10 minutes. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues. Dans un contexte marqué par l'inflation et par la tentation d'une renonciation aux espèces qui près d'abord les ménages les plus pauvres. Il nous revient cet après-midi d'examiner la proposition de loi de nos collègues Rémi Féraud et Jean-Claude Tissot et de l'ensemble des membres de leur groupe visant à renforcer l'accessibilité et l'inclusion bancaire. Déposés dans le cadre de l'ordre du jour réservé au groupe socialiste, écologiste et républicain. Ce texte, qui propose notamment de faciliter l'accès aux distributeurs automatiques de billets et de redéfinir les modalités de plafonnement de certains frais bancaires pour les plus fragiles a été examiné dans les conditions du gentleman agreements. Avec les auteurs. Nous avons acté que les points de divergence entre nous était trop important. Ce qui a amené au rejet du texte en commission. Nous examinons donc la proposition de loi dans sa version initiale et à mon tour je veux saluer l'esprit dans lequel nous avons pu travailler avec les auteurs de la loi et en particulier avec Rémi Féraud, membre également de la commission des finances. Cette proposition vise d'abord comme cela a été rappelé à confier à la Poste. Une nouvelle mission de couverture territoriale en distributeur automatique de billets C'est l'article 1er, financée par un fonds chargé de garantir leur accès en moins de 15 minutes, c'est l'article de. La commission des finances propose de supprimer ces articles et ce pour plusieurs raisons. D'abord on n'observe pas de dégradation de l'accessibilité Audab puisque plus de 99% de la population vit à moins de 15 minutes en voiture d'un DAB. L'objectif visé est donc largement satisfait. Au contraire. La nouvelle mission attribuée à la Poste par l'article 1er pourraient être porteuses d'un effet d'aubaine conduisant au désengagement des banques avant l'entrée en vigueur de la loi. Le rapport sénatorial de mars 2021 pour l'avenir des missions de service public de la Poste de nos collègues chaises. Cardon avait d'ailleurs exclu toute nouvelle obligation légale de service public visant à garantir l'accès de la population DAB sur l'ensemble du territoire. J'y reviendrai au moment de présenter mes amendements mais ce rapport miser sur d'autres solutions d'accès aux espèces qu'il s'agit de privilégiés et en particulier le casting choc qui compte déjà plus de 25.000 points d'entrée dans notre pays mais qui gagnerait à être opérables entre les établissements bancaires. L'article de créer un fonds de garantie de la présence bancaire territoriale pour financer la nouvelle mission de la Poste. La commission propose logiquement sa suppression, d'une part parce qu'ayant supprimé l'article 1er, il n'aurait plus d'objets et d'autre part en raison de modalités de financement critiquable. Outre les contributions volontaires des collectivités, les recettes de ce fonds qu'on prendrait un effet, une taxe sur les bénéfices des établissements bancaires et une contribution des établissements à l'occasion de la fermeture des DAB. Concernant la taxation des bénéfices des établissements bancaires pour laquelle aucun taux n'est prévue, celles-ci ne concernerait pas les néobanques et risquerait de conduire à un renchérissement des services bancaires. C'est toutefois la contribution des banques à l'occasion de la fermeture d'un DAB qui est la plus problématique. Elle frapperait les banques de façon indifférenciée selon l'endroit de fermeture. De même, faire contribuer aujourd'hui les banques qui ont maintenu une présence sans impliquer celles qui ont quitté les territoires depuis longtemps serait injuste. Au total, le financement de ce nouveau fonds paraît inéquitable mal répartis trop mal définis pour soutenir de façon pérenne un élargissement des missions de la Poste qui au demeurant vise à remplir un objectif aujourd'hui largement satisfait. J'en viens maintenant au dernier point de divergence entre la Commission et les auteurs, l'article 7 qui vise à imposer à la commission des sanctions. De l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'ACPR le prononcé d'une sanction pécuniaires à l'encontre de l'établissement de crédit qui ne respecterait pas ses obligations en matière de droit au compte, ou qui n'appliqueraient pas la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement. Cette disposition nous semble excessive. La commission des sanctions de la CPR, qui est une autorité indépendante doit pouvoir rester souveraine dans le choix de la sanction la plus adaptée dans un cadre contradictoires bien établies. Elle aussi superfétatoire puisque la commission des sanctions dispose, y compris sur les sujets liés au droit au compte d'un pouvoir de sanction pécuniaires dont elle a d'ailleurs déjà fait usage. Les articles 3 à six vise à enrichir l'information sur le droit au compte et l'offre spécifique ainsi qu'à réduire les frais bancaires des publics les plus fragiles. la commission pardon propose de les modifier. L'article 3 prévoit que la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement défini les conditions d'affichage au sein des agences bancaires de l'information relative au droit au compte et à l'existence de l'offre spécifique. Cet article a pour objectif d'améliorer l'information des clientèles fragiles et du public. J'ai souscrit pleinement l'information à disposition des clientèles fragiles présente en effet des lacunes et nombreux sont nos compatriotes qui n'ont pas accès à des services adaptés à leurs besoins. Faute de les connaître. Je proposerai donc de prolonger la réflexion de nos collègues, auteur de la proposition de loi sans en altérer l'esprit l'amendement de la commission prévoit ainsi d'élargir le Champ des informations que les banques sont tenues de fournir au public et aux personnes fragiles pour inclure outre les informations sur le droit au compte et l'offre spécifique des informations sur la procédure de traitement du surendettement. Le microcrédit, l'exercice du droit d'accès aux fichiers gérés par la Banque de France et les moyens de la contacter sur l'ensemble de ces sujets. La charte préciserai également les modalités de diffusion de cette information par leur affichage à l'agence bancaire ou d'autres moyens, selon ce qui paraît le plus pertinent, enfin cette charte devrait aussi définir les conditions de formation de certains professionnels sociaux les publics relais afin de leur permettre d'orienter et d'accompagner au mieux les potentiels bénéficiaires du droit au compte et de l'offre spécifique. L'article IV prévoit que les plafonds spécifiques sur les frais d'incident réservé aux bénéficiaires de l'offre spécifique et du droit au compte soit proportionnelle au revenu ce qui paraît trop complexe à mettre en oeuvre et supposerait par ailleurs la connaissance par la banque de l'ensemble des revenus de la personne portant ainsi atteinte à la confidentialité des données fiscales. La commission propose donc la mise en place de sous plafond pour les bénéficiaires de l'offre spécifique et du droit au compte. Dans la situation financière et la plus délicate. L'article 5 vise à introduire dans l'offre spécifique, une autorisation de découvert sans frais là encore proportionnelle aux revenus. Outre le problème de la proportionnalité. Cette disposition est contestable, non seulement en ce qu'elle pourrait faire courir le risque d'une spirale d'endettement, mais aussi en ce elle introduirait un droit au crédit encore inexistant dans le droit français. L'établissement de crédit est un effet libre d'accorder ou non un crédit à une autorisation et ou une autorisation de découvert en revanche. Nombre de clients craignent de perdre leur autorisation de découvert au moment de souscrire l'offre spécifique. Un amendement de la commission propose donc de préciser dans la loi de manière explicite que ces deux phénomènes sont indépendants. Enfin, afin d'éviter un report vers d'autres frais. Entraînés par les articles 4 et 5, l'article 6 prévoit que les frais bancaires soumis à la dénomination réglementaires existantes sont limitées pour les bénéficiaires du droit au compte de l'offre spécifique au tiers des facturations appliqués par l'établissement de crédit et sont plafonnées par mois et par par mois et par opération en fonction du revenu des personnes. La limitation des frais proposée par est porté une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle des établissements de crédit et semble redondante avec les plafonds par mois et par opération proposée par ailleurs. Le plafonnement par mois semble lui aussi excessif dans la mesure où les frais bancaires mentionnés ici inclurait les frais de gestion. Au-delà des frais d'incident. Néanmoins, l'introduction de d'un simple plafonnement des frais par opération dont le niveau serait fixé par le pouvoir réglementaire et qui serait réservé aux seuls bénéficiaires de l'offre spécifique et du droit au compte ne me paraît pas excessive la commission présente un amendement en ce sens. Au total, le texte poursuit des objectifs louables, au niveau de l'inclusion bancaire et contient des orientations intéressantes mais mérite donc vous l'avez compris, d'être modifiée pour le rendre opérante. Si les propositions de la commission ont été retenus. Elle appellerait bien sûr à son adoption. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jean-Noël Barrot Ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Madame la présidente, monsieur le président de la commission. Monsieur le. Rapporteur le gouvernement partage évidemment l'objectif d'assurer à l'ensemble de la population à l'ensemble de nos concitoyens. L'accès à des services bancaires de qualité à des tarifs appropriés. Cependant, nous pensons que les mesures proposées par cette proposition de loi ne permettent pas d'atteindre en tant que telle. Cet objectif. Fondamentalement, la proposition de loi prévoit 2 grands types de mesures, d'une part un renforcement de l'accessibilité bancaire territoriale en confiant une mission additionnel à la Banque Postale qui serait appuyé par la création d'un fonds de garantie de la présence bancaire territoriale. D'autre part une évolution des plafonnement des frais bancaires appliqués aux personnes bénéficiaires de la procédure de droit au compte et à celles en situation de fragilité financière ayant souscrit l'offre spécifique ainsi qu'une évolution du contenu de cette oeuvre. Si vous me le permettez je répondrai point par point aux propositions formulées. Par l'auteur de cette proposition, monsieur sénateur Ferrero pour exposer les raisons qui amènent le gouvernement lui y être défavorable. Sur l'accessibilité bancaire territoriale tout d'abord nos concitoyens, quels qu'ils soient sont particulièrement attachés au service de proximité et à la vitalité du territoire dans lequel ils vivent. Nous partageons collectivement la nécessité de lutter contre l'enclavement et de préserver l'attractivité de l'ensemble de nos villages et de nos économies locales qui sont le visage de notre pays et ce, notamment, à l'heure où la. Touche l'ensemble du territoire et où nous assistons à la désertification des services de proximité accessible à nos concitoyens, parfois les plus vient vulnérables. Cette attractivité passe notamment par la garantie de pouvoir avoir accès à notre monnaie commune, l'euro sous forme d'espèces moyen de paiement inclusifs par excellence, permettant les achats. De la vie quotidienne en toute liberté. Il est le sel de nos marchés de l'économie de proximité sociale et solidaire, ou encore de notre lien collectif avec les plus démunis. Aussi le gouvernement et la Banque de France sont très attentifs à préserver l'accès de chacun de nos concitoyens aux espèces, force est de constater que le maillage du territoire pour l'accès aux billets est très bon. Et qu'il est globalement inchangé d'une année sur l'autre. C'est surtout dans les territoires très urbain sur lequel il y a un équipement qui est massif que se concentre la légère diminution du nombre de distributeurs, l'optimisation des installations existantes dans les zones les mieux équipées, se fait au bénéfice du maintien de distributeurs automatiques de billets dans les zones les plus isolées. Ce qui est positif, la robustesse de la filière fiduciaire est en permanence garantie en temps de crise, comme récemment durant les périodes de confinement. L'émission et la distribution des espèces a été maintenue pour répondre au plus près aux besoins de nos compatriotes. Ce maillage garanti par l'action volontariste des établissements bancaires de proximité permet à plus de 99% de la population métropolitaine âgés de 15 ans et plus de se situer à moins de 15 minutes en voiture d'un distributeur automatique de billets. Le rapporteur, l'a rappelé cette dynamique permet notamment de placer la France comme le second pays de l'Union européenne en terme de densité des réseaux d'agences bancaires bien au-delà de la moyenne européenne, avec 549, agence par million d'habitants en France pour une moyenne européenne de 255 agents, c'est-à-dire à peu près 2 fois moins. En complément, commerçants de proximité viennent de renforcer de manière opportune ce maillage. Le nombre de points de distribution dans les commerces est en augmentation et permet de maintenir un accès de proximité, notamment dans des territoires isolés avec bientôt 30.000 points de retrait privatifs. La possibilité de retirer des espèces lors d'un achat chez un commerçant et simple sans complexité administrative. Et permet en. Plus de renforcer l'attractivité des services de commerces locaux. Le retrait d'espèces effectués sans achat associé est en plein développement et s'installe durablement dans le paysage de nos territoires en permettant notamment un lien social et rapproché entre consommateurs et commerçants. Par ailleurs, la Poste. Chargé par la loi du 2 juillet 90 d'une mission d'accès aux espèces maintient déjà au-delà de ses besoins commerciaux, un réseau de 17.000 points de contact, notamment dans les zones rurales et de montagne, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les départements d'outre-mer. Aussi en perspective alors que les transporteurs de fonds par le rachat de certains distributeurs automatiques de billets viennent maintenir le maillage existant alors que les commerçants complètent le dispositif d'accessibilité. L'objectif de garantir l'accès aux espaces à tous nos concitoyens y compris dans les territoires enclavés ou isolées nous semble être préservés pour les années à venir. J'en viens maintenant à la question des frais bancaires et à la question de l'inclusion bancaire. À titre liminaire, je souhaiterais partager avec vous quelques grands constats. Premièrement il est économiquement justifié que les banques facturent leurs prestations de service ainsi que certains frais en cas d'incident. Ces incidents qui correspondent à un fonctionnement anormal du compte induisent des coûts de gestion pour les établissements bancaires il génère d'ailleurs également des coûts pour le bénéficiaire du paiement qui n'est pas payé en cas d'incident et qui n'est dans l'écrasante majorité des cas, pas une banque. Deuxièmement, les Français bénéficient en moyenne d'un niveau de facturation. Des services bancaires qui est satisfaisant. Depuis 2017, les frais bancaires sont globalement orientés à la baisse en raison principalement de la digitalisation et de l'augmentation de la concurrence sur le marché des services bancaires. Troisièmement le secteur fait déjà l'objet de diverses réglementations ambitieuse pour limiter les abus, notamment pour tous les Français. Certains services bancaires sont gratuits. C'est le cas par exemple du relevé mensuel ou de la clôture du compte. Et certains types de frais sont plafonnées pour l'ensemble de la population comme le rejet de chèque 30 euros ou 50 euros selon le montant ou le rejet de prélèvement 20 euros ou bien encore les commissions d'intervention, 8 euros par opération. Euros par mois. Dans ce cas, de la proposition de loi vise en 1er lieu à diviser par 2 ses plafonds par opération actuellement applicables aux principaux frais d'incident et à introduire un plafond annuel pour chacun de ces frais. Ces plafonds bénéficierait à l'ensemble de la population et des plafonds spécifiques plus bas s'appliquerait à la clientèle fragile. Nous pensons que la volonté d'abaisser les plafonds des différents frais d'incident pour toutes les clientèles n'est pas pertinente. La baisse des plafonds qui s'appliquerait également aux clientèles les plus aisés enverrait un signal négatif. Ce qui importe n'est pas de rétablir la police administrative des prix en matière de tarifs bancaires mais de protéger celles et ceux qui en ont besoin. Nous croyons que le dispose actifs actuel, qui prévoit un plafonnement global des frais d'incident concentrée sur les populations les plus fragiles qui en ont le plus besoin. Demeure la meilleure réponse pour arrêter le plus rapidement possible les effets de sur sur accumulation de frais car il est vrai que dans certains cas, ces frais sont largement subi et peuvent créer une spirale d'endettement aggravant la situation des clients fragiles. Le gouvernement a travaillé sans relâche au cours des années passées pour mettre en place ce dispositif qui a aujourd'hui fait ses preuves. Ce nouveau cadre a été élaboré depuis 2018 selon une méthode inédite et qui a fonctionné, qui est celle d'une approche partenariale avec les établissements bancaires, suite aux engagements pris par les établissements bancaires en 2018 devant le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Lemaire et le président de la République Emmanuel Macron les personnes fragiles bénéficient désormais d'un plafonnement global de leurs frais d'incident bancaire. 25 euros par mois pour les clientèles fragiles et 20 euros par mois 200 euros par an pour les clients fragiles bénéficiaire de l'offre spécifique ses engagements dont la mise en neuve re-contrôlée par l'ACPR et l'observatoire. De l'inclusion bancaire. Ont porté leurs fruits. Cette stratégie a été payante. L'Observatoire de l'inclusion dedans. Qui a requis l'instance publique de suivi des politiques d'inclusion bancaire en effet dressé un bilan positif des actions engagées par le gouvernement. Je me période donner quelques chiffres des résultats obtenus. 4 millions de clients sont considérés comme fragiles financièrement fin 2021 et donc bénéficiaires des disques. Positif de plafonnement des frais, c'est 20% de plus par rapport à 2018. Le montant moyen des frais facturés par les banques à leurs clients considérés comme fragiles est en diminution, 221 euros en 2021, soit 10% de moins qu'en 2020 et enfin l'offre spécifique se diffuse presque 700.000 bénéficiaires de l'offre spécifique à la fin 2021, c'est-à-dire une progression de. 56% par rapport à 2018. Mesdames, et messieurs les sénateurs, les Français ménage comme entreprises ont la chance de pouvoir compter sur un système bancaire robuste qui finance efficacement l'économie comme il l'a démontré encore durant cette crise et qui applique des frais globalement raisonnables ces dernières années, le gouvernement a agi de manière résolue pour renforcer l'accessibilité l'inclusion bancaire. L'encadrement en matière de frais bancaires avec pour objectifs et priorités de mieux protéger ceux pour qui une intervention de l'État. Nécessaire, c'est-à-dire les personnes en situation de fragilité financière. C'est chose faite avec des résultats que je vous ai évoqué et cela été con a con. Puis, à la faveur d'une approche partenariale avec le secteur bancaire, qui je crois est un gage de succès dans la durée, le gouvernement continuera d'être vigilants et exigeants dans son dialogue avec les banques et de conduire certaines réformes lorsque cela sera nécessaire. Mais les réformes conduites jusqu'ici ont d'ores et déjà permis d'atteindre un point d'équilibre et c'est la raison pour laquelle le gouvernement sur un certain nombre de propositions d'amendements. Tout au long de nos débats et et s'opposera à. La proposition à. La proposition de loi. Qui est examiné aujourd'hui. Merci. Dans la suite de disques. Plus en général. La parole est à monsieur Bernard buis pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants pour 4 minutes. Madame la présidente. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Monsieur le président de la commission des finances. Mes chers collègues. La proposition de loi que nous étudions cet après-midi vise à renforcer l'accessibilité et l'inclusion bancaire. Aujourd'hui nous sommes dans une situation où un peu plus de 4 millions de titulaires de comptes bancaires sont considérés comme fragiles par l'observation par par l'Observatoire de l'inclusion bancaire, selon un rapport publié en 2021. Cela étant, quels sont les éléments qui permettent d'attester de la fragilité bancaire d'une personne. Pour être considérés comme en situation financière fragile. Il faut remplir 3 conditions précisées par le code monétaire et financier. La première, avoir effectué le dépôt de dossier de surendettement recevable la seconde avoir été inscrit pendant 3 mois consécutifs au fichier central des chèques et enfin avoir été identifiés par la banque comme étant en situation de fragilité financière. Au titre des revenus et des instits dans constatés sur le compte. Autant d'éléments qui nous rappelle qu'une part non négligeable de nos compris triote sans dans une série de sécurité financière quotidiennement angoissante insécurité face à laquelle nous ne pouvons rester impassible, cela est en fait si le groupe RDPI partage également la volonté de renforcer l'accessibilité et l'inclusion bancaire, force est de constater que les mesures proposées par notre collègue nous semble inefficiente et disproportionnée. D'une part certains dispositifs présentés dans le texte ne permettent pas d'apporter des réponses convaincantes et pertinente aux enjeux d'accessibilité et d'inclusion bancaire par exemple, la mission de couverture territoriale. À la Banque Postale engendrerait une charge supplémentaire non compensée par les dispositifs de financement établit à l'article de. Outre le fait que cette mesure pourrait entraîner un désengagement des autres banques sur l'établissement de nouveaux distributeurs automatiques. Nous ne pouvons pas légitimement imposer à la Banque Postale. Cette pression financière injustifiée. L'article 3, qui impose des obligations d'information en matière de droit au compte et doivent. Spécifique ne représente à mes yeux qu'une redondance de la législation actuellement. Par Par la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement adoptée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. L'article IV qui impose un plafonnement des commissions proportionnelles aux revenus commissions perçues par les établissements de crédit pour les irrégularités de fonctionnement du compte bancaire entraînera inexorablement des difficultés d'application elles seront notamment provoqué par la complexité de collecte des informations nécessaires et par le potentiel, problème de lisibilité des nouveaux plafonds. Les dispositions établies à l'article IV hein durée définitivement un risque de surendettement pour les plus précaires à cause de cette volonté d'instaurer une autorisation de découvert sans frais et proportionné aux revenus. D'autre part, certaines mesures de la proposition de loi sont à mes yeux, totalement disproportionnée. Je pense notamment à l'article 6 contraire à la liberté d'entreprendre lorsqu'il prévoit une double-plafonnement des frais de services bancaires. Mais je pense surtout à l'article 7 qui impose à la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le fait d'adopter une sanction pécuniaires à l'encontre de tout établissement de crédit qui ne respecterait pas ses obligations en matière de droit au compte ou n'appliquerait pas la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement. J'estime qu'on ne le rapporteur qu'une telle disposition obligatoire est excessive, la possibilité d'imposer des sanctions pécuniaires sans qu'un juge puisse se prononcer pose nécessairement un problème dans d'autres États de droit. Pour toutes ces raisons, notre groupe ajustera sa position sur cette proposition de loi en fonction des amendements adoptés. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jean-Claude Tissot pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour six minutes.

Madame la présidente, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Comme l'a présenté. Mon collègue Rémi Féraud, avec lequel j'ai eu le plaisir de m'associer pour rédiger cette proposition de loi. Ce texte est une réponse cohérente à des inégalités territoriales et sociales qui fracture de nombreux départements territoires ruraux il zones urbaines défavorisées. Le point de départ de notre réflexion ce cette proposition de loi fut le constat partagé, que ce soit à Paris ou dans nos départements en particulier le mien la Loire du profond détachement de nos concitoyens avec les institutions bancaires. C'est donc dans une volonté de répondre aux enjeux sociaux et économiques par des mesures concrètes que notre groupe a inscrit ce texte dans cette niche aux côtés d'une proposition de loi pour résorber la précarité énergétique. Le premier axe de la de la présente, proposition de loi. Qui me tient à partir de Marrakech et la question de l'accessibilité bancaire. Je m'étonne que sur ce point, la droite sénatoriale qui se positionne souvent comme la grande défenseure des territoires ruraux ne soit pas plus intéressée par les propositions que nous formulons car oui et je pense que les collègues de tous les bancs pourrait aisément le confirmer, il existe une désertification bancaire qui se traduit par la fermeture des agences point de contact essentielle pour les clients, mais aussi par l'abandon progressif de certains distributeurs automatiques. Et une nouvelle fois ses désertification bien cibler les mêmes qui subissent déjà l'absence d'offre de soins de proximité, la fermeture des commerces communaux et le terribles recul des services publics dans les territoires. En toute logique ce cumul d'inégalités d'accès crée un profond sentiment de déclassement et d'abandon chez nos concitoyens. Je pense donc sincèrement qu'en tant que membres représentant des territoires. Il est de notre devoir d'anticiper et de répondre à cette problématique. À ce sujet monsieur le rapporteur. Lors de nos échanges qui ont été courtois. Vous avez évoqué qu'une grande majorité des Français se trouve à moins de 15 minutes d'un distributeur Matic de billets nos départements respectifs n'étant pas très éloigné, je pense que vous reconnaîtrez facilement que ses déplacements peuvent facilement varier en fonction des territoires et qui peut également être parfois rendues difficiles à certaines périodes de l'année. Je pense aussi qu'il faut ne pas oublier l'ensemble des publics qui n'ont pas les moyens de se déplacer, que ce soit pour des raisons de santé ou d'impossibilité d'accès à des moyens de transport. C'est la raison pour laquelle le dispositif que nous proposons en intégrant une composante territoriale dans l'émission du groupe La Poste 10 à anticiper et à garantir cette présence bancaire sur l'ensemble du territoire. Parler du maintien des distributeurs automatiques c'est logiquement aborder la question du liquide de l'espèce et de sa place dans notre société, c'est un sujet paradoxal avec une demande sociale mais aussi une réglementation qui s'est accentuée pour empêcher certaines dérives toutefois la réalité de nos territoires doit également guider notre action et il est certain que les paiements en liquide sont au coeur de nombreuses interactions au niveau local et je pense particulièrement à l'ensemble des événements associatif ainsi par ce texte nous avons réellement souhaité poser la question du maintien d'un système de paiement à la fois inclusifs et qui permettent en toute liberté le paiement en liquide d'achat de la vie quotidienne. Dans le travail de réflexion sur ce texte nous avons logiquement analyser l'ensemble des dispositifs qui permettent l'accès à l'eau de l'espèce des points relais, commerçants et le dispositif allô facteurs sont intéressants à ce titre mais ils sont, de l'aveu même des représentants de la Banque Postale très peu connue et donc très peu utilisé très peu utilisé, garantir le maintien des dates dans les territoires reste donc pleinement pertinents aux côtés d'une démocratisation de ses autres dispositifs d'accès pour financer cette nouvelle mission. Nous proposons la création d'un fonds dédié alimenté en partie par une contribution des établissements bancaires en cas de fermeture d'un. Ici, le principe est clair, vous faites le choix de quitter un territoire défavorisés. Très bien, c'est votre choix. Mais vous allez devoir participer pour que l'offre de service seront maintenus pour les habitants du territoire concerné. Alors que les nouvelles missions. Au groupe La Poste sont en permanence sous compenser dans une logique purement libérale nous proposons ici ah si un dispositif cohérent et sur le 2ème axe de cette proposition de loi, nous avons souhaité proposer des solutions concrètes pour renforcer l'accompagnement et la protection des plus précaires dans ses relations toujours particulière avec les établissements bancaires sur ces articles. Je salue les échanges avec le rapporteur qui permettront je l'espère d'avoir et d'obtenir des avancées lors des débats que nous aurons dans quelques instants et face à la complexité des démarches administratives, le renforcement de l'inclusion bancaire doit être une priorité pour ne laisser aucun citoyen en difficulté financière sur le bord de la route. C'est pour cela que nous avons proposé des mesures très concrètes en commençant par l'adaptation des offres spécifiques dans ce contexte de crise du pouvoir d'achat et d'augmentation des dépenses courantes pour l'alimentation et l'énergie notamment à ce sujet, nous rappelons que le baromètre mensuel de l'inclusion financière. Publié le 13 avril, la Banque de France a souligné une hausse de 20% des inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers depuis la le début de l'année 2023. De plus, avec près de 17% de la population qui souffrent d'électronique. Le canal numérique ne peuvent pas être la seule voie d'échanges entre les banques et ses clients. Le renforcement de l'information en agence est donc indispensable, c'est ce que nous proposons à l'article 3. Alors que la Banque Postale prend en charge près de 1,6 millions de clients jugés fragiles, soit 47% de ce public. Cette proposition de loi a également pour objet d'interpeller les autres établissements bancaires pour leur demander de renforcer leur effort pour ces pour ces publics que ce soit sur l'information ou dans les offres proposées. Seules des sanctions pécuniaires comme prévu à l'article 7 pourront contraindre les acteurs économiques du secteur à agir en faveur de ces publics. Mes chers collègues, vous le voyez, nous vous proposons un texte avec des mesures très concrètes pour répondre à de réelles préoccupations dans nos territoires ruraux et Merci cher collègue. La parole est à monsieur Pascal Savoldelli. Pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour quatre minutes. madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Accéder à la monnaie fiduciaire, autrement dit aux espèces est-il un droit que la loi doit consacrer. Ou de cette première question se pose à nous parlementaires de déterminer si la Poste devrait garantir cette mission reconnue de service public via l'installation et la maintenance des distributeurs automatiques de billets au plus proche de nos concitoyennes et nos concitoyens. Excusez-moi de penser même si la présence est pas au rendez-vous. Mais il y a quand même un barrage que la droite est érigé pour mettre en échec la garantie d'un nouveau droit. De sa consécration et de sa mise en oeuvre concrète en promouvant l'égalité territoriale. Et nous remercions nos collègues socialistes pour cette proposition de loi. Avant je veux dire que la majorité sénatoriale. Et petites opérations de démantèlement monsieur chers collègues Sautarel. La majorité de droite sénatoriale se cache derrière une statistique. Vous l'avez évoqué pour motiver son refus. 99,2% de nos concitoyennes et nos concitoyens peuvent accéder un distributeur à moins de 15 minutes. Derrière ces statistiques qui se veut implacable bien sûr se cachent des réalités territoriales très varié qui semble échapper à ceux qui prétendent les représenter. Je ne vais pas vous rappeler la différence entre une moyenne et une médiane. D'abord parce que 3,6% de la population habitent dans l'une des 12.013 communes très peu dense que compte le territoire ce sont eux à qui s'adresse cette proposition de loi, ce sont eux qui doit faire 30 minutes ou plus si leur distributeur est en panne et près d'un quart d'entre eux, 542.000 personnes qui ne jouissent pas du pouvoir de choisir leur moyens de paiement, faute de trouver un distributeur dans l'horaire de vie immédiate. Opportunément cette proposition de loi propose de mettre à contribution les bénéfices des banques. Une taxe sur les distributeurs qui ferme. Alors évidemment on a entendu une manière c'est feutré mais réel. Allez encore un impôt s'offusque certains à droite qui semble avoir d'autres idées d'ailleurs que l'impôt pour financer les services publics. Ça viendra. Attention, nous dit-elle car les banques vont retirer leurs distributeurs avant que la loi soit votée et donc vider les recettes potentielles dévolu à la Poste pour l'installation du distributeurs de billets. Autant d'arguments idéologiques faut pour certains qui crée des problèmes et à imaginaire à défaut de trouver des solutions à ce bien réelle de nos compatriotes. Si 4598 distributeurs de billets soit de vie. 77% d'entre eux ont tout bonnement disparu. Il ne faudrait pas y voir un phénomène structurel de l'action du système bancaire, pour faire disparaître les espèces. Et non sans une certaine ironie que nos concitoyens se rassure, il existerait de nombreuses solutions alternatives aux distributeurs de billets que chacune et chacun fréquente. Peut être. Vous connaissez le dispositif allait allô facteur service de livraison d'espèces à la demande par un postier, signe que l'argent physique serait vouée à disparaître, à l'instar du courrier car les Françaises et les Français s'en serait détournée, c'est faux. La numérisation des services publics a délaissé le courrier l'habitude de l'usage de l'écrit pour interagir avec l'administration, tout comme il est devenu impossible de payer autrement qu'en ligne pour fait effectuer un nombre d'achat un autre dispositif encourager aussi le cash in shop. Qui permet à des commerçants de délivrer des espèces qu'on sera paiement par carte supérieur au prix d'achat, la généralisation de cette pratique à tous les commerçants et non plus les seuls clients d'un même réseau bancaire représente une fuite en avant. Enfin franchement, est-ce que la livraison de colis dans les points relais a accru la fréquentation des commerces qui la pratiquent. On a tous vérifier que c'est non. Les gens viennent et récupèrent et ils s'en. Est-ce que le magasin de vêtements de centre-ville concurrencés par la vente en ligne connaîtra un élargissement considérable de sa clientèle grâce à ce nouveau service. Bien sûr que non. Pire, ces commerçants exposeront leur sécurité en détenant une quantité d'espèces qui n'est pas le cas des distributeurs qui à part quelques cas regrettable de voiture bélier ou quelque fraude à la carte bleue ne revêtent pas de risque majeur pour l'intégrité des personnes physiques. Sur le volet inclusion bancaire nos amendements portent une triple volonté empêcher les banques de rémunérer sur les clients financièrement difficulté sortir certaines opérations d'un objectif de rentabilité école et garantir des offres de justice sociale. Merci. Merci. La parole est à Madame Sylvie Vermeillet. Pour le groupe Union centriste pour six minutes.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, chers collègues. Au nom du groupe Union centriste, je salue l'initiative de Rémi Féraud, et des membres de son groupe qui, avec cette proposition de loi permette un nouvel examen de l'accessibilité bancaire dans notre pays. Rémi Féraud a raison de pointer. Ces quelques points qui ont déjà fait débat dans notre assemblée. Elles ne paraissent toujours pas réglé. Face à la diminution du nombre de distributeurs automatiques de billets leur inégale répartition Rémy propose notamment la création d'un fonds de garantie de la présence bancaire territoriale. Je me permets de rappeler qu'en novembre 2018, nous avions examiné une proposition de loi de notre collègue Éric Gold sur ce sujet et puis ce que j'en avais été désigné rapporteur je pense utile de rappeler quelques conclusions de l'époque, je faisais état en 2018 de 56.000 distributeurs automatiques de billets et notre rapporteur Stéphane Sautarel nous indique qu'il y en aurait 47.853 en 2021. C'est-à-dire que plus de 8000 distributeurs ont disparu en 5 ans, soit près de 15%. Alors effectivement je trouve ce chiffre bien trop élevé, voire inquiétant. Plus encore, il s'agit de connaître l'exacte répartition de ces distributeurs en 2018, nous n'ignorions par le coût d'investissement et de fonctionnement des DAB aussi nous avions souhaité connaître la cartographie de l'emplacement de ces appareils. À cet effet, un groupe de travail mandaté par la Banque de France avait été créé afin de recenser précisément l'offre d'accès aux espèces tous canaux confondus et définir les scénarii d'organisation pour garantir l'accès aux espèces cette cartographie devait nous être présenté en janvier 2019, le 27 mars 2019. Notre commission des finances s'est réunie sur le thème des moyens de paiement et à procéder notamment à l'audition de Eric là Courrèges alors directeur général des services à l'économie et du réseau de la Banque de France que je cite en ce qui concerne la cartographie. Je suis désolé de vous décevoir mais elle n'est pas terminée. Il ne s'agit pas d'une volonté de rétention d'informations, nous avons recueilli beaucoup de statistiques auprès de l'ensemble des réseaux bancaires nous pourrons vous donner un état des lieux extrêmement précis d'ici à la fin du printemps. Monsieur là Courrèges n'a, il est vrai pas précisé de quelle année. Il s'agissait mais nous n'avons chers collègues jamais été destinataire de cette carte, je le dis avec force c'est inadmissible. Comment débattre valablement aujourd'hui de la présence bancaire de son évolution. Sans cet outil indispensable. C'est un préalable que nous devons exiger et je souhaite que notre commission des finances en soit enfin destinataire. En janvier 2019, monsieur le gouverneur de la Banque de France, a déclaré un autre commission des finances. La Banque de France n'a, n'abandonnera jamais les espèces. Nous sommes au titre de nos missions monétaire garant de la liberté de choix des Français dans leurs moyens de paiement. Nous n'avons pas à favoriser les espèces plutôt que la carte ou le paiement par mobile mais nous devons faire en sorte que chacun de ces moyens de paiement, soit également accessible d'égale qualité et d'égale sécurité aussi. Il serait heureux que le Parlement et la commission des finances du Sénat qui le demandent dispose des éléments nécessaires à l'appréciation du nombre et de l'emplacement des distributeurs automatiques de billets. Il sera alors plus aisé de remédier aux besoins territoriaux. C'est pourquoi, en l'absence de documents précis mon groupe partage l'avis de notre rapporteur qui supprime les articles 1 et 2 de la proposition de loi siphon et péréquation il doit y avoir un jour ce ne peut être qu'à la condition de détenir une cartographie en temps réel. Cependant, nous mettrons en garde contre un engrenage qui pourrait s'avérer dangereux celui de rendre un fonds pérenne et indispensable. Dès lors, les établissements bancaires conditionnerait l'ouverture d'un distributeur de billets au recours du fond et cela générerait d'autres complications quel montant pour le fond comment distribuer le fond et respecter la libre concurrence entre les différentes banques, c'est un sujet que nous n'avons pas abordé et qui mériterait clairement réponse. Nous validons les améliorations pertinentes proposées par notre rapporteur concernant les articles 3 A6 car en matière d'information dans un objectif d'efficience la qualité doit aujourd'hui primer sur la quantité. De même, nous approuvons la proposition du rapporteur de supprimer l'article 7 car nous pensons que la PCR doit rester souveraine dans ses décisions, décisions qu'elle rend déjà publiques et qui sont par là même sans doute plus pénalisante que le niveau de la sanction en tant que telle. Notre groupe votera donc cette proposition de loi, telle qu'amendée par notre rapporteur dont je suis élue, le travail et espère qu'à l'occasion de futures réunions de la commission des finances, nous puissions enfin disposer de tous les éléments nécessaires à une véritable appréciation de la présence bancaire en France, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Christian Billac hein pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 4 minutes.

Madame la présidente. Monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur. Monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues. Dans la continuité de la proposition de loi mon collègue Éric Gold qui avait été adoptée par le Sénat. 1018. Je commencerai par rappeler les problèmes de désertification bancaire. Que qu'on a seulement pour nos territoires ruraux. Avec la fermeture des gens je bancaire et la disparition du distributeur billets.

Contrairement à feu qu'on voudrait nous faire croire, il existe un réel problème de désertification bancaires en France. Qui sont des messieurs que n'a pas sur ton territoire. L'exemple d'une agence ou d'un distributeur automatique de billets redonne de fermer ou reste un ramonage le fermeture. En disant le nombre je je bancaire a ainsi baissé de 10% en France. Et un milieu rural, le phénomène de désertification est encore plus marquée. Hé bien entendu ne concerne pas que l'accès aux diffuseurs de billets. Il manque aussi de médecins, on en a parlé des transports collectifs des couvertures américain téléphonique des voyantes, voire inexistantes. La disparition des commerces de proximité. Une partie de la population vit mal la disparition de service public mais aussi des services au public. Les équipements utiles au quotidien ce ressenti chez aussi celui qui conduit la colère et aux extrêmes. Je voudrais rappeler qu'il n'y a pas de citoyen de seconde le journal qu'il n'y a pas de territoire de seconde zone. D'une part les populations les plus fragiles vieillissante et moins mobiles. Sont parfois dépendante des espèces en euros. Pour le gouvernement de rachat mais aussi dépendant de leur voiture pour leurs déplacements. Faire plusieurs kilomètres pour voitures argent constitue donc le difficulté supplémentaire notamment pour les personnes âgées qu'une heure plus conduire et les personnes à mobilité réduite, qui sont les premières à victime du désengagement des 20 coiffure nos territoires. D'autre part il faut bien comprendre que nos données s'approprie moins bien les moyens de paiement modernes. Et sont moins dotés en outils numériques. Il n'est pas question de nier l'émergence de nouvelles pratiques qui se porte davantage vers les outils et modes de paiement numériques mais considérer que la dématérialisation est aujourd'hui actée hé bien vécue par l'ensemble de la population. Constitue une erreur fondamentale. Enfin nos territoires le vérifiera tous de la couverture numérique indispensable à l'utiliser un jour d'un terminal de paiement. Dans certaines zones, l'accès à Internet ou à la téléphonie fixe est entravée et le règlement par carte bancaire se révèle impossible. À l'instar de la présente, proposition de loi, la proposition de loi du RDSE. Prévoyait dans sa version initiale, la création d'un fonds destiné aux même qui a des distributeurs romantique le billet là les zones rurales. La présente, proposition de loi risque avec les amendements que nous allons examiner tout à l'heure. Ne pas répondre à toutes les problématiques. Mais les dispositions vont quand même dans le bonne femme. Et donc je voterai propositions. Comme la majorité des membres du RDS. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à madame Véronique Favreau pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes.

monsieur le ministre, monsieur le président de la commission. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Il est aujourd'hui quasiment impossible de vivre son compte bancaire. En effet, bon nombre de transactions ne peuvent être effectués que par chèque, virement au paiement par carte. Posséder un compte est un droit, ne pas en peut en posséder aurait pour conséquence de désocialisés la personne. Si seulement 1% de la population n'est pas bancarisés c'est parce qu'il existe des dispositifs comme le droit au compte ou des formules qui permettent aux plus fragiles, de bénéficier d'une offre bancaire adéquate à leur situation. Certes des carences peuvent être observés en matière d'information relatives au droit ton compte. Toutefois la formation existe et accessible. Preuve en est, du taux de bancarisation de la population de 99%. Il convient d'encourager le travail que mène actuellement la profession bancaire pour fluidifier ce dispositif. Attention la notion de fragilité multi-facettes en matière de comportement bancaire on distingue la cigale et la fourmi. Si certains clients ont des difficultés financières à cause de petits revenus. D'autres ne savent pas gérer leur argent. Cessons de ne travailler que sur les conséquences de la fragilité mais travaillons aussi sur les causes toute l'approche commerciale des banques doit reposer sur la connaissance que le conseiller bancaire a, de son client en privilégiant une approche client au détriment d'une approche produit le conseiller peut personnaliser son offre son accompagnement et aider son client a retrouvé une santé financière une dignité afin qu'il sorte de ce dispositif. Traiter la cause c'est aussi travailler sur l'éducation financière, que ce soit au niveau des scolaires mais aussi des adultes. Je suis d'avis que l'introduction d'une autorisation de découvert sans frais proportionnelle aux revenus n'est pas une mesure adéquate, elle pourrait faire courir le risque d'une spirale d'endettement et introduire un un droit du au crédit qui n'existe pas en droit français. Laissons la main aux banques pour agir en fonction de la connaissance client si 700.000 clients opté pour l'offre pour personnalité fragile en 2021 soit une hausse de 80% depuis 2019. La proposition de cette offre dépend aussi des valeurs de l'entreprise bancaire certaines ne veulent pas gérer cette clientèle peu rentable quand d'autres mettent en place des dispositifs spécifiques comme par exemple une plateforme dédiée à cette clientèle qui est a pour objectif de les rencontrer, de les informer, de les accompagner. Cette offre est et doit rester une offre transitoire et donc si ces banques a développé ce système. Nous sommes conscients que l'accès aux services bancaires est un élément fondamental pour la vie quotidienne de nos concitoyens, c'est une question de justice sociale. Ces barrières peuvent et du. On vient de le voir aux difficultés financières à un manque de connaissances mais aussi en raison de la distance géographique comme il l'a déjà été dit chacun a accès à un distributeur à moins de 15 minutes. Il est cependant nécessaire de travailler le maillage territorial et se et il ne faut surtout pas confondre le nombre de DAB implanté du nombre de points d'espèces. Mieux vaut un Dave qui fonctionnent que plusieurs qui ne sont pas utilisées, donc plus rentable ce maillage doit être aussi. Adaptée à l'évolution du comportement du consommateur qui délaissent les centre-ville au profit des centres commerciaux, en terme de maillage d'autres solutions Audab existe comme il a été dit le cache une bague le cash Back pardon et le cash in shop sont déjà prévenu par le code monétaire et financier certes l'utilisation du cash-Back reste encore faible mais celle du cash in shop se développe et devrait évoluer pour exemple le Crédit Agricole avec ses relais CA propose un service de retrait notamment dans les zones rurales pour ses clients chez des commerçants comme les boulangeries les épiceries et les boucheries là où il n'y a pas d'agence bancaire. Ce service pourrait être universaliser de manière à ce que les commerçants concernés puissent distribuer des espèces à d'autres clients que ceux des banques qui les ont mandaté c'est le sens de la réflexion actuelle de certains groupes bancaires. Enfin pour terminer le fonds de garantie de la présence bancaire alimenté par une taxation sur les sur les bénéfices sanctionneraient-ils tous les établissements. Qu'en est-il de la taxation des bénéfices des des banques en ligne. Autre initiative locale pour conserver des distributeurs. Certains établissements se sont associés pour pour gérer collectivement les distributeurs. Si certaines mesures proposées dans cette. PPL vont dans le bon sens il est nécessaire d'apporter quelques ajustements pour les rendent plus efficace et équilibré, notamment pour les personnes fragiles, c'est pourquoi le groupe républicain est favorable à provision de la loi c'est qui m'ont dit par notre collègue et rapporteur Stéphane Sautarel. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Danny Watts blé pour le groupe les indépendants pour quatre minutes. la la présidente. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Monsieur là le président de la commission des finances, mes chers collègues. Les distributeurs de billets sont voie disparition cette crainte, on l'entend partout en France et notamment dans nos campagnes. En zone rurale, elle participe du cercle vicieux de la désertification. Moins d'habitants, c'est moins de commerce et donc moins de transactions. Moins de retrait. Moins distributeur et ainsi moins de service. C'est le rôle du Sénat en tant que territoires d'apporter des solutions aux problèmes que nous constatons sur le terrain. Les espèces reste le moyen de paiement plus et des Français. En 2019. La Banque de France estimé que 59% des paiements s'effectuent en espèces qu'2,5% par carte. On comprend mieux pourquoi les Français s'inquiètent de voir disparaître les gens s'bancaires. Ou les les de billets. Depuis. La pandémie a bousculé les habitudes. Le paiement sans contact a été favorisée. À la fois par les banques et par les commerçants. Pourtant jeudi les paiements en espèces reste majoritaire. Il peut avoir des différences d'ordre générationnel ou géographique, mais les chiffres sont là. Il ne s'agit pas aujourd'hui de prendre parti pour les espèces ou pour la carte bancaire soit dit en passant la question. Est intéressante. Le gourdin a de bonnes raisons de se méfier des espèces qui sont soit difficile à contrôler. La question qui nous est posée aujourd'hui c'est de savoir s'il faut légiférer pour garantir un maillage des distributeurs dans les territoires. L'article de la pression de loi fixe un objectif clair, garantir l'accès à un distributeur de billets en moins de 15 minutes sur chaque point du territoire. Le problème c'est que l'objectif est déjà atteint dans les faits, les données de la Banque de France que j'ai cités établissent que 99% des Français ont aujourd'hui accès instruire de billets en moins de 15 minutes. L'intérêt de légiférer. Le pape ne me paraît pas réel. En revanche, la taxe qui servira à financer le service public. Distributeurs de billets que nos collègues socialistes appellent de leurs voeux. Cette taxe elle serait bien réelle et elle finirait pas renchérir le coût global des services bancaires. Si la qualité de nos services publics était proportionnelle au nombre de taxes permettant de financer. Alors la France soit championne du monde. Or ce n'est pas le cas. Nous posons de notre supprimer cette taxe. Qui pénalisera le pouvoir d'achat des Français. La proposition de loi contient d'autres mesures qui me paraissent extrêmement pertinentes, notamment pour renforcer l'information des clients. Les sanctions contre les banques qui ne respectent pas leur obligation. Nous sommes favorables à ces mesures. mais iront pas bancaire en jetant toujours plus de taxes et de contraintes. Pénaliser les banques ce n'est pas favoriser leurs clients. Il en va de même pour l'accès au crédit qui s'est durcie après la remontée des taux d'intérêt. Il faut plutôt en faciliter l'accès.

Madame la présidente, monsieur le ministre. Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous le savons, le développement économique des dernières décennies s'est accompagnée d'une utilisation des services bancaires d'une part croissante de la population et d'une dématérialisation grandissante des échanges financiers. De ce fait. Plus que jamais l'accès à un compte et aux services bancaires est-il devenu une condition nécessaire d'inclusion à la vie économique et sociale de la France. À l'instar de ce qui a été constatée à la suite de la crise de 2008. Les situations de personnes privées d'un compte notamment à la suite d'incidents de paiement pourraient se multiplier en raison de la crise économique actuelle. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. À dans un tel conteste le grand mérite de provoquer vis à plusieurs outils d'accentuer la vigilance que nous devons à nos concitoyens les plus fragiles dans le contexte de crise aiguë que nous connaissons depuis 2020. Les conséquences économiques et sociales pèsent déjà lourdement sur leur situation financière. Veiller à ce que davantage de précarisation n'en résulte dans un contexte marqué par la tentation du neurone assertion. Space qui contreviendraient à terme à la liberté de choix des moyens de paiement nous au nord dans le devoir que nous avons de protéger les ménages les plus pauvres et les plus précaires. Aujourd'hui encore, bien que 99% de la population dispose d'au moins un compte en banque. Nous devons veiller à ce que des mécanismes d'accès aux services bancaires et aux moyens de paiement puisse prévenir le basculement dans la fragilité financière et l'entrée dans la spirale du surendettement, même si depuis quelques années, les dispositifs d'accompagnement associant pouvoirs publics, banques et acteurs associatifs se sont ainsi développer. De même la question des frais bancaires doit être souligné actuellement aucune sanction pénale n'est prévue pour le cas où la banque appliquerait les frais pour incidents supérieurs au plafond est à lui par la loi. C'est ce système d'impunité reposant sur une grande complexité qui fait que le citoyen se retrouvent totalement désarmés face à ce qui lui est imposé. Or les frais bancaires qui pèse sur les citoyens constitue précisément un des obstacles à la réalisation de l'objectif d'inclusion bancaire pour lequel il a existé en commission un large consensus s'normal que les banques facturent leurs services. Il n'est pas admissible que ces frais soient totalement décorrélés du coût réel des prestations qui sont supposés rémunérées. Aussi avec mon groupe nous avons déposé des amendements visant à limiter. Dans certaines conditions le plafonnement de ces derniers, veillant à protéger des publics les plus fragiles, par un système de plafond en fonction du niveau de ressources corollaire de l'inclusion sociale l'inclusion territoriale est un dépend non moins essentiels sur lesquels il convient également de se concentrer. Nous avons entendu les propositions du rapporteur en commission sur le degré de couverture territoriale. Cela étant bien des fois les chiffres ne correspondent pas à la réalité que de nombres d'entre nous connaissons sur nos territoires les agences bancaires et bureaux de poste présents sur le territoire ne se répartissent pas de manière uniforme. C'est bien une fermeture qui peut passer inaperçu. En ville ou dans des communes périurbaines mais être catastrophe catastrophique dans les villages ruraux. Pour lesquels les 15 minutes de trajet en voiture son croyez-moi vu des conditions de circulation dans des départements comme le mien et comme bien d'autres. La réalité des chiffres et des statistiques s'opposent parfois à celle du vécu à la réalité de la désertification bancaire dans nos populations. Celles pour qui la promesse de garantir un égal accès aux services bancaires sur tout le territoire n'est pas tenu La FBF reportait que les communes dépourvues d'un distributeur étaient majoritairement des communes de petite taille est situé en zone rurale. Sur 28.664 communes non équipé d'un distributeur

Je vous remercie. Merci beaucoup. La discussion générale est Close. La commission n'ayant pas élaboré de texto, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initial. Et à l'article premier j'ai une prise de parole de monsieur Marc la Mini. Oui merci madame. La présidence. Monsieur le Ministre ce Monsieur le président de la commission. Des finances sur le rapporteur général monsieur le rapporteur. Chers collègues, je voudrais aussi saluer l'initiative. De nos collègues Rémi Féraud Jean-Claude Tissot. Et. Et au niveau de son groupe socialiste écologiste républicain de cette proposition de loi qui a le mérite, je dirais de. Poser les problèmes. De l'accessibilité bancaire et puis aussi de faire référence à l'utilité. Le rôle indispensable de la Poste. Alors concernant cet article 1. Attribution La Poste d'une mission de couverture territoriale complétant en distributeur automatique de de billets puis l'on raisonne surtout en notion d'aménagement du. Du territoire puis en rappelant aussi le pour le travail d'auditions que qui a été. Réalisé avec beaucoup de d'intervenants. il y a des chiffres qui sont intéressants. 31 12 2022 17.013 points de contact, c'est elle été rappelé par les collègues dont 7000, un bureau de poste 6915 agences postales communales et intercommunales. on peut malheureusement regretter. Je dirais. Le. L'évolution en baisse des moyens humains. Et je prends l'exemple l'objectif 99% de la population située à moins de 15 minutes en voiture d'un d'un il y a eu départements qui font exception qui sont en dessous de 90% dont les Ardennes. Dont je le, que, que je représente. Donc c'est aussi un, un argument à prendre en compte. je rappellerai le travail du du rapporteur et et qui indique que les nouvelles missions impliquerait une charge supplémentaire de la Poste c'est différents. Arguments donc je me relirai néanmoins à la position du rapporteur je vous remercie. Merci cher collègue. Alors 2 amendements identiques de suppression le 15. Blé. Merci madame la présidente. Cet article propose de créer une sorte de service public de distributeurs de billets qui seraient bien sûr à la Poste. La mise en oeuvre de cette mais émission sur réalisée par la Banque Postale, filiale de la Poste. Ce qui poserait un problème de concurrence vis-à-vis des autres banques. Ce nouveau service public aurait pour mission d'assurer la couverture territoriale complète en la France dispose qu'on nous l'avons déjà dit, d'un très bon maillage. Cette création qui avait ce public avec contrainte législatives et les taxes complémentaires qu'elle implique, ne me paraît pas justifié. Donc c'est pour ça que je demande la suppression de cet amendement. Je dis merci l'amendement 18 pour la commission, monsieur Sautarel. Tu le auras Oui merci madame la présidente, monsieur le ministre effectivement cet amendement vise à supprimer l'article 1er de la proposition de loi qui confie à La Poste une mission de couverture territoriale complète tant en ce qui concerne les implantations que l'entretien et l'approvisionnement des DAB. Donc le déjà évoqué dans dans dans discussion générale. Il est évident que comme les auteurs de la proposition de loi. J'estime que, malgré le développement de moyens de paiement dématérialisé, l'accès aux espèces doit être garantie et il importe en effet de laisser à chacun le choix de son moyen de de paiement par ailleurs les espèces constituent pour les ménages les moins aisés, un outil indispensable à la gestion de leur budget. Toutefois, cet article ne saurait être adoptée et ce pour 3 raisons principales que je vais rappeler brièvement. Tout d'abord le dispositif proposé pourrait entraîner un désengagement territoriale des banques, ce qui alourdirait la charge de la Poste et le rapport sénatorial de mars 2021 sur l'avenir des missions de service public de La Poste avait expressément exclu la possibilité de cette nouvelle obligation légale de service public. Ensuite, ça a déjà largement été dit l'objectif d'accessibilité Audab. dans par cet article est largement satisfait avec les 99 2 %, même si effectivement c'est une moyenne et en tant qu'élu d'un département rural. Je sais qu'il faut aussi se méfier des moyennes. Toutefois, il y a pas non plus de différenciation territoriale qui soient apportées dans la rédaction de l'article enfin le dispositif se concentre sur le sujet de la présence territoriale des DAB, alors qu'il y a aujourd'hui, ça a été là aussi rappelé d'autres moyens d'accéder aux espèces et et à ce titre-là je je voudrais solliciter. L'avis du gouvernement sur le fait que la modification. Du droit européen permette de pouvoir universaliser l'accès au au casting choc qui est un moyen effectivement de retraits de liquide dans les commerces sans mouvement. Commercial, contrairement au cashback qui a été évoqué tout à l'heure et qui permettrait si on était sur une universalité. De l'offre sans doute d'un. Améliorer l'accès. Donc voilà la raison pour laquelle la commission propose par cet amendement la suppression de l'article premier, je vous remercie. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame le présente même avis que le. Rapporteur et et sur la question qu'ils soulèvent c'est le gens du du cash il chope il y a bien des travaux engagés pour s'assurer qu'il est bien une interopérabilité entre les banques et que ça puisse bien fonctionner. Merci. Alors je vais donner la parole à Monsieur Féraud pour explications de vote et je préviens l'assemblée que nous aurons un scrutin public. Merci madame la présidente. D'intervention pour dire que je regrette évidemment amendements de suppression de l'article 1er de l'article de parce que les 2 vont ensemble. J'entends bien que. Notre proposition qui implique à la fois une réglementation supplémentaire et une taxe supplémentaire ne vous enchante pas néanmoins, et pas seulement sur les rangs de la gauche, plusieurs collègues ont témoigné de la réalité de la désertification bancaire un certain nombre de territoires ruraux et. Plus importante d'ailleurs que les chiffres ne semble le dire mais nous avons des chiffres très partielles et ensuite surtout du risque que cette désertification bancaire soit un phénomène qui soit devant voir peut-être que notre proposition n'est pas parfaite mais elle avait le mérite d'elle a le mérite d'exister et par ailleurs de prévoir un financement qui ne fassent pas qu'à la fin, ce soit la Poste qu'il en soit pour ses frais ou bien le contribuable par une dotation pour une nouvelle mission de service public mais que ce soit bien une responsabilité collective, prise en charge par l'ensemble du secteur bancaire nous aurons créé un débat sur cette question, je suis sûr qu'il reviendra et qu'il faudra que nous soyons vigilants et que nous trouvions aussi des solutions face à cet enjeu auquel le cacher une chope ne peut pas répondre au seul. Merci. Donc j'ai été saisi d'une demande de scrutin public donc par le groupe Les Républicains sur les amendements identiques, 15 et 18 et dont le 18 et celui de la commission l'avis du gouvernement est favorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Alors résultat du scrutin. Nombre de votants 343 exprimés, 342 pour 238 contre 104, les amendements sont donc. Adopté et l'article 1er supprimé. À l'article de deux amendements identiques de suppression le 16 monsieur What blé. L'article 2 vise à créer un fonds de garantie pour la présence bancaire éditorial dont les recettes seraient générés par une taxe sur les bénéfices des banques. Se font prendre la forme d'intéressement plus national à caractère administratif chargé de garantir l'accès à un distributeur. En moins de 15 minutes sur chaque point de territoire l'accès des services bancaires le monde pas

Merci l'amendement 19 de la commission. Monsieur le rapporteur. Oui madame la présidente. Effectivement, cet amendement vise à supprimer l'article 2 qui prévoit la création du du fonds de garantie de la présence territoriale bancaire chargé de garantir un accès en moins de 15 minutes à un distributeur automatique de billets se font appuierai financièrement le groupe La Poste, pour qu'il puisse assumer sa mission de couverture territoriale prévue à l'article 1 pour financer ces dépenses 3 types de recettes sont prévues sur les bénéfices des établissements bancaires une contribution versée par les établissements bancaires au moment de la fermeture d'un DAB et les contributions volontaires des collectivités territoriales dans le cas d'une contractualisation. La création de ce fonds paraît peu utile. Il est en effet chargé de garantir l'accès à une dame en moins de 15 minutes. Cet objectif-là et aujourd'hui déjà garanti et par ailleurs le mécanisme de financement du Fonds. Inéquitable et porteur de difficultés avec l'introduction d'une nouvelle taxe, dont le taux n'est pas fixé et qui semble contestable en ce qu'elle concernerait pas les néobanques et risquerait de conduire à un renchérissement des services bancaires. De plus elle frapperait les banques de façon indifférenciée, quelle que soit l'endroit de fermeture comme je l'ai signalé tout à l'heure. Pour toutes ces raisons, donc, il vous est proposé. Cet amendement visant à supprimer l'article. En cohérence avec la suppression de l'article 1er, je vous remercie. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre favorable. Alors je suis saisi aussi pour le vote d'un scrutin public hein. Merci demande du groupe le les républicains donc pour les amendements, 16 et 19 et le 19 et celui de la commission. Hein pardon. Je ne vous avez pas vu. Mais si si bien sûr que c'est grave. C'est pas grave du tout madame la présidente. C'est une explication de vote d'ailleurs qui aurait pu valoir sur l'aussi la, la suppression de l'article. Le premier, moi je trouve que Rémi Féraud, l'a bien dit pour cette proposition socialiste franchement mettent un fonds qui garantit la présence territoriale bancaire aurait mérité plutôt la sagesse qu'un esprit de sanctions et de suppression. tout était pas réglé mais la sagesse aurait pu faire que s'acheminait positivement. C'est évident que les bénéfices des banques n'était pas déterminé donc c'était un une difficilement applicable et nous avions, nous, notre groupe proposer un amendement qui supprimait la contribution des collectivités territoriales au financement de l'an, l'implantation de l'entretien des distributeurs de billets et pour une raison simple, c'est quand même aux banques de financer service. Et et, excusez-moi de le dire ici. Mais écoutez, si les Françaises et les Françaises nous écoute. 150% de hausse des bénéfices nets par exemple de BNP Paribas pour le seul 1er trimestre, annoncé ce matin. 4 4 milliards d'euros en 3 mois. Croyez pas qu'il y a de l'argent pour installer des distributeurs franchement. Voilà donc je voulais vous dire ça et et ça a été dit aussi par notre collègue tout à l'heure vers midi et c'est on, on va s'habituer on va banaliser la disparition des DAB. Voilà, c'est ça qui va se passer dans l'accès aux espèces à l'a chuté de 8,77% entre 2018 et 2021, et en fin de compte en résiste en réagissant pas en soutenant cette proposition de loi qu'on le veuille ou non, on est en train de banaliser et normaliser la disparation des distributeurs d'accès d'espèces à une partie de nos concitoyennes et concitoyens. Voilà c'est pour ça que vote. Contre ces 2 hommes. Merci, merci monsieur le rapporteur général. Juste quelques mots de en réaction à la prise de parole de notre collègue Pascal Savoldelli. Je pense qu'il faut, il faut dire les choses jusqu'au bout. qui est de moins de. Deux lieux de retraits d'espèces, notamment de distributeurs automatiques de billets. Alors pour dire la vérité. Ça veut pas dire. Que on ne va pas optimisé. Je m'explique, quand on est en milieu urbain. Souvent il y avait pléthore d'offres. Dans un périmètre très restreint. Alors je suis désolé mais quand les banques disent que ça coûte cher. Il y a quand même un problème du côté des banques. Ou que ce soit l'installation l'entretien, l'alimentation coûte. Globalement, Globalement, sur une moyenne le mépris. Donc là je, je ne vous rejoins pas ce qu'il faut en fait, c'est avoir un maillage équilibré. Avec alors des des distribuera automatique de billets, mais également des nouvelles formes. Il y a 4 de distribution et de retraits d'espèces. Je crois que c'est ça qu'on doit avoir et, quelque part de faire avec et l'accès aux espèces. 0 zones blanche sur le territoire national. Et pour ça, j'aurai l'occasion de le redire. Je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut avoir une cartographie en temps réel des évolutions. Il est normal que les choses évoluent, là où il y a des populations nouvelles et puis qui est éventuellement donc des accès nouveau là où on réorganise parce que il y a éventuellement des moyens nouveaux qui peuvent remplir peu ou prou. Quel que soit le moyen distribution la même fonction. Ben moi je peux l'entendre. Donc le fait de simplement retenir le chiffre brut d'une baisse ne veut ne signifie pas forcément que le niveau de service. S'est réduit. En tous les cas sensiblement. Merci madame Vermeillet.

Et je pense que vraiment on. On a des moyens pour pouvoir l'exigeait. Et c'est pas possible qu'on l'obtienne pas alors qu'on nous l'avait promis pour. Début 2019, donc je pense que la moindre des choses c'est qu'on obtienne cette cartographie pour savoir et puis surtout je crois que ça a pas été dit au travers des. Des discussions des uns et des autres. Là où il peut manquer d'étape de façon assez. Sensible, c'est peut-être pas forcément dans le monde rural aujourd'hui c'est la périphérie des zones urbaines. C'est là a priori que les banques ferme. Des DAB. C'est une zone qui devient sensible et puis il y a les communes touristiques, dont parfois la population va être multiplié par 10. Lors des vacances et là il peut y avoir un manque d'accès aux espèces. On est, on, on peut. Voilà à penser que il y a ces besoins dans ces endroits là, mais on n'a pas de certitude parce qu'on n'a pas de cartographie et moi j'estime que, avant de pouvoir voter la création création d'un fonds, il faut savoir précisément de quoi on parle. Merci. Alors je vais donc mettre aux voix, j'ai été saisi. Donc d'une demande de scrutin public. Par le groupe Les Républicains sur les amendements identiques, 16 et 19. L'amendement 19 étant celui de la commission. Je vous rappelle que l'avis du gouvernement est favorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

le scrutin est clos. résultat du scrutin. Nombre de votants, 343 342 pour 238 contre 104. Les amendements ont été adoptés et l'article 2 et donc supprimée. À l'article 3, j'ai une prise de parole de monsieur Alain Cadec. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous traitons aujourd'hui de la proposition de loi visant à renforcer l'accessibilité et l'inclusion bancaire le chapitre II évoque l'accessibilité sociale bancaire. Dans ce chapitre, j'ai déposé un amendement visant à renforcer les droits des demandeurs de crédit et à assurer une transparence dans les décisions de refus de crédit des banques. Je souhaite en effet que les établissements de crédit et agences bancaires. Soient tenus de fournir une explication écrite aux demandeurs de crédit en cas de refus de sa demande. Cette explication aiderait les clients à mieux comprendre leur situation financière et à améliorer leur dossier de crédit pour l'avenir. Malheureusement mon amendement a été déclarée irrecevable. Au titre de l'article 45. Pourtant, quel serait alors le texte adapté afin de défendre les personnes cherchant à obtenir un crédit pour finaliser un projet et qui finalement ne l'obtiennent pas sans connaître. Les motifs du refus. Pour ne pas être touché par l'article 45. La solution serait peut-être que je dépose une PPL. En tous les cas je voulais faire cette remarque, parce que j'y tenais beaucoup et je voulais remercier les 55 collègue. De sensibilités diverses dont certains d'entre eux sont des membres éminents de notre assemblée et de la commission des finances, qui ont cosigné cet amendement. Qui par ailleurs me semble de bon sens. Voilà, je voulais faire cette petite remarque parce que, je regrette qu'il ait été retoqué par l'article 45. Merci beaucoup madame la présidente. monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente. Je voulais simplement prendre un instant la parole après l'intervention de notre collègue Alain Cadec effectivement sur Iran recevabilité de de d'un amendement qui avaient pu déposer parce que ça me fait l'occasion de, de préciser qu'en fait la portée. De ce texte de cette PPL de de de nos collègues touchent les publics fragiles et donc tous les les les amendements qui concernait l'ensemble des Français. Sans me prononcer sur le bien-fondé ou la pertinence de ce qu'il pouvait défendre

monsieur le rapporteur. Vous gardez la parole pour défendre votre amendement le 20. Oui merci madame la présidente, effectivement, l'article 3 de la présente PPL vise à modifier le contenu de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement, de telle sorte que les informations relatives au droit au compte et à l'offre spécifique fasse l'objet d'un affichage dans les agences bancaires. Cet article vise à améliorer l'information du public sur les dispositifs à destination des personnes fragiles et donc je l'ai déjà dit dans la discussion générale, on ne peut que. Poursuivre et partager cet objectif dès lors le présent amendement propose de modifier cet article sans en altérer l'esprit et même en pour en allant plus loin encore dans la réflexion engagée par les auteurs, je crois, de la proposition de loi, d'une part il dispose que la charte précise la nature des actions de formation et de sensibilisation entreprise par les établissements de crédit auprès des associations qui accompagnent les personnes fragiles et par ailleurs. Il propose également. Il prévoit que la charte définit les informations que les établissements de crédit devront porter à la connaissance de la clientèle et du public En prolongeant les propositions des auteurs. La banque seraient tenus de fournir, outre les informations sur le droit au compte et l'offre spécifique. Des informations relatives à la procédure de traitement du surendettement au micro-crédit et à l'exercice du droit d'accès aux fichiers gérés par la Banque de France, la charte préciserez les conditions de diffusion de ces informations, parmi lesquels pourra figurer l'affichage Anne agence mais pas seulement. Voilà donc cet amendement vise tout en respectant l'objet poursuivi par les auteurs à renforcer et amplifier. Le souci d'information auprès de l'ensemble des publics. Merci. Avis favorable du gouvernement. Merci. Monsieur Féraud. Merci madame la présidente, je voudrais remercier le rapporteur pour son amendement il poursuit exactement le même but que celui de notre article peut être avec plus de subtilité et de pertinence que nous, donc nous le voterons bien volontiers. Merci cher collègue. Alors j'ai été saisi d'un scrutin public sur la. Ah il est retiré. D'accord il est retiré. Donc je mets aux voix l'amendement de la commission qui a reçu un avis favorable du gouvernement. Donc il est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est donc adopté je mets aux voix l'article 3 qui est pourri. Ah oui y a j'ai pas suivi hein donc. L'article 3 modifier est ainsi adopté. Après l'article 3 l'amendement numéro 11 monsieur Savoldelli. Oui merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à ne pas rajouter de la misère à la misère. Nous souhaitons notre groupe interdire la perception de frais d'incident les fameuses commissions d'intervention pour les 4 un million de personnes en situation de fragilité financière et qui sont en nombre en augmentation de 300.000 entre 2020 et 2021. Il s'agit des allocataires du RSA des APL de l'allocation adulte handicapé et des étudiants boursiers. Ces frais sont liés à un compte non suffisamment approvisionné. Pour faire face à une dépense et frappe de plein fouet nos concitoyennes et concitoyens qui ont oublié une facture qui doivent s'acquitter d'une dette fiscale qui sont ça vous fera peut-être plaisir dans le rouge, plus tôt que prévu. Et si, depuis le 1er janvier 2014, les commissions d'intervention sont plafonnés à 8 euros par opération et 80 euros par mois en principe 25 euros par mois pour les clients fragiles et maximum 20 euros par mois et 200 euros par an pour les personnes qui ont souscrit une offre spécifique clients fragiles. C'est un 1er pas mais on peut constater quand même une forme d'indécence à bénéficier d'une offre spécifique clients fragiles. Pour bénéficier de frais un peu moindre. En gros ce plafonnement se veut pas se valoir de solde de tout compte. Je vous donne un exemple pour une personne seule allocataires du RSA, le plafond des incidents bancaires représentent 3,34% de ses ressources mensuelles pour avoir mis pour avoir commis une seule faute ne pas être aisée et pour ne pas être à découvert. Et quand je dis pour les plus précaires, les étudiants, les gens qui ont des allocations. Je pense que ça doit être 0 frais bancaires incidents. Et que les banques ne crient pas. Au secours, quand ils ont 6 milliards de bénéfice Net sur les 6 premiers mois de 2022. Ils peuvent ne pas être alimenté par ses petits épargnants qui aurait. Fauté. Une seule fois. Donc voilà c'est un élément pour de justice sociale. Voilà pour les plus fragiles, les plus isolées. Merci, merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Oui madame la présidente. Le le l'amendement défendu par notre collègue propose effectivement la suppression des commissions d'intervention pour les personnes fragiles et les bénéficiaires de certains minima sociaux. Il nous apparaît que cette exonération totale des commissions d'intervention paraît excessive. Puisque dans les commissions, la nature de ces commissions sont hybride il y a certes les frais d'incident dont notre collègue a fait a fait a fait part mais il y a aussi des services rendus en contre des contreparties de services rendus. C'est pourquoi il convient de de préférer un plafonnement. Plutôt qu'une exonération totale et à ce titre là je vous renverrais, au aux amendements de la commission aux articles 4 et aux articles 6 qui propose d'aller plus loin dans ce plafonnement en. Diminuant en fait tout en proposant de diminuer le niveau et la charge pour les publics les plus fragiles. Par ailleurs, la liste des critères retenus à sans lien Direct avec l'objectif. Poursuivi, je ne vais pas les rappeler ici, et enfin pour ses pour ces dispositions est un effet il faudrait que les banques sachent que leurs clients sont bénéficiaires d'aides sociales et accès aux données confidentielles qui ne leur sont pas aujourd'hui accessibles et et donc elles auraient du mal à ce titre-là à les retenir. C'est la raison pour laquelle je vous propose, chers collègues, soit un retrait ou faute de quoi un avis défavorable. Pour votre amendement. Merci. Merci l'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Merci madame la présidente. Même avis que. Le rapporteur retrait ou défavorables. Merci. Alors je vais mettre aux voix l'amendement numéro 11 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient donc pas adopté. À l'article 4 l'amendement. Du gouvernement, monsieur le ministre. Merci madame la présidente. Donc l'amendement proposé par le gouvernement. La protection des des consommateurs notamment des des plus vulnérables constitue, vous le savez, une préoccupation majeure du du gouvernement. du gouvernement. Le dispositif de plafonnement actuel s'il peut être encore amélioré à l'Avantage de concilier efficacité dans son ciblage et simplicité dans sa mise en oeuvre ainsi le dernier rapport de l'Observatoire de l'inclusion bancaire publié en juin 2022 fait notamment état d'une baisse importante des frais facturés aux clients. Moins 10% sur un an. Sur la totalité des frais, moins 17% sur les frais des incidents. Par ailleurs, le rapport 2022 de l'Observatoire des tarifs bancaires indique c'est sur les principaux frais appliquer à l'ensemble de la clientèle huit tarifs. Sur 1400 stable et un tarif est en baisse. À l'inverse, la mise en place d'une proportionnalité aux revenus dans le plafonnement des commissions commissions d'intervention contribuerait à complexifier fortement le dispositif existant au détriment de sa simplicité de son objectif d'équité en réduisant la notion de fragilité au seul critère de revenus certains publics aujourd'hui protégés pourraient être demain moins bien couverts aussi. Ce dispositif serait très difficile à mettre en oeuvre par les établissements bancaires, compte tenu des informations à mobiliser au risque de mal couvrait couvrir pardon certains publics fragiles. Le gouvernement propose donc de conserver le régime législatif actuel et la flexibilité réglementaire associé permettant de paramétrer les différents plafonds de frais. Je vous remercie. Merci. Monsieur Sautter est pour. La commission avis. Merci la présidente. Je vais donner un avis personnel sur cet amendement, puisqu'il est arrivé tardivement et donc nous n'avons pas pu l'examiner en cet amendement qui vise à supprimer l'article IV qui introduit un plafonnement des commissions d'intervention en fonction du revenu. Si je peux partager les préoccupations du gouvernement quant à la complexité de l'article IV mais son ambition sociale me paraît devoir être. En effet, si les commissions d'intervention sont aujourd'hui le font aujourd'hui l'objet de plafond spécifique pour les personnes financièrement fragiles. Ceux-ci sont fixés à 20 euros par mois c'est certes assez peu mais pour des personnes qui ne perçoivent et ne créditent leur compte que de somme tout à fait modeste. Cela peut devenir beaucoup c'est pourquoi je présenterai un amendement dans les minutes qui suivent, de réécriture proposant sous plafond pour ceux des bénéficiaires de l'offre spécifique ou du droit au compte qui présente une situation financière particulièrement délicate. C'est pourquoi je demande le retrait de cet amendement au profit de l'amendement 21 de la commission, ou à défaut un avis défavorable. Merci Monsieur Féraud pour explication de vote. je regrette que le gouvernement présente un un amendement de suppression d'autant que de toute façon l'avis du gouvernement est défavorable sur l'ensemble du texte. Je voudrais dire que ça n'est pas parce que la situation en matière de frais bancaires et moins mauvaise, un peu moins mauvaise depuis. 3 ou 4 ans grâce à des améliorations de la réglementation que c'est le conte de fées que nous a décrit le ministre-Barrot qui était. Au banc du gouvernement juste avant dans son intervention tout à l'heure. Non, ça n'est pas un conte de fées. Et je crois que le gouvernement devrait écouter les banques comme il le fait bien sûr mais devrait aussi écouter les représentants des consommateurs et les associations qui accompagnent les personnes les plus fragiles parce que nous sommes loin d'une situation idéale. Il y a encore beaucoup de progrès à accomplir et l'article IV dans notre version comme dans celles amendé par le rapporteur à la mérite de permettre d'améliorer une situation qui aujourd'hui mais absolument pas la situation idéale que décrit le gouvernement. Merci monsieur Bachelet. Madame le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Juste un sujet de méthode. Monsieur le Ministre. Ah vous êtes trop occupé en ce moment que vous n'avez pas vu arriver ce texte, c'est que vous êtes obligé de déposer cet amendement quelques instants avant son examen. Quelle est votre conception du travail du gouvernement sur les textes d'initiative parlementaire. C'est un vrai problème, Monsieur le Ministre. Je sais bien que c'est pas votre texte particulièrement donc mais vous êtes le représentant du gouvernement. Ici je veux dire. Par défaut. Mais ce n'est pas normal. Vous comprenez bien que ça n'a aucun sens. Vous auriez peut-être pu améliorer trouver mais là bon c'est assez brutal, on supprime. On n'a pas vraiment grand chose à dire, il y a un sujet. Il est posé. Par les auteurs de la PPL il est amélioré. Par le texte de la Commission et du rapporteur. Mais vous n'avez pas de propositions. Bon ben. Passez muscade. Non. Non vous ne travaillez pas ces sujets là. C'est vrai vous avez trop de textes vous n'arrêtait pas d'en déposer sur le bureau du Sénat et nous sommes débordés texte du gouvernement, donc je comprends que vous y été débordé. Non ce n'est pas sérieux et c'est un vrai sujet pour de nombreux français. Merci monsieur Savoldelli. Oui merci merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes, mes, mes chers collègues. Ça m'évitera de parler après notre groupe soutiendra les 2 amendements. Parce que faut quand même qu'on apporte des réponses aux Françaises et aux Français. Alors moi je me félicite qu'il ait quelques avancées mais enfin. Tout va bien, tout va bien. 46% des Français sont à découvert au moins une fois par an pour un coût annuel moyen de 232 euros. Chaque mois il y a 8 millions de Français qui doivent s'acquitter de frais d'incident. Avec un chiffre d'affaires pour le secteur bancaire qui avoisine les 6, 5 milliards d'euros. Donc vous voyez quand je regarde ça. J'ai, il faut essayer de prendre ce qu'on peut prendre comme avancé. C'est pour ça que notre groupe avait déposé des amendements. Certains ont été frappés de recevabilité mais qu'en même temps ça fait avancer un petit peu de la justice sociale. on les votes. C'est pour ça qu'on votera les deux amendements qui précède dont celui de la commission présentée par Monsieur Sautarel. Oui, mais merci. Alors je vais mettre aux voix l'amendement 26 du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est donc pas adopté 2 amendements. De rédaction global en discussion commune. L'amendement quatre La ma présidente chers collègues cet amendement poursuit 2 objectifs. Il vise tout d'abord encadré explicitement l'ensemble des commissions indifféremment de leur appellation. En effet, certains établissements bancaires ont développé des tautologie interne permettant d'échapper au plafonnement. Il est donc nécessaire d'inscrire dans la loi que toutes les commissions sont plafonnées. Dans un second temps, cet amendement directement au niveau législatif des plafonds pour l'ensemble des citoyens. Et pour ceux en situation de fragilité financière les plafonds actuels sont trop élevés, il est donc proposé de diviser par 2, les coûts pour l'ensemble des clients. S'agissant des plus précaires les limites correspondant au quart des montant fixé pour l'ensemble des clients. Ces limites sont donc exprimés par mois et par an et par opération. Merci l'amendement 21 de la commission sur le rapporteur. Oui madame la présidente le cet amendement. le plafonnement pardon des commissions d'intervention bancaire concerne l'ensemble de de la clientèle toutefois des plafonds spécifiques, on l'a rappelé sont applicables aux personnes bénéficiant du droit au compte ou de l'offre spécifique pour mieux les protéger. Partant du constat que pour nos concitoyens les plus modestes. 20 euros par mois et les frais bancaires peut s'avérer un montant élevé l'article IV de la présente, proposition de loi prévoit qu'en ce qui concerne les commissions d'intervention des plafonds spécifiques soient désormais proportionnel aux revenus des personnes. Un tel dispositif sera à la fois peu lisible et et très difficile à à mettre en oeuvre et afin de mieux protéger les clients dont les ressources sont particulièrement faibles. Le présent amendement propose donc de substituer à l'article 4 initial. Un dispositif de sous plafond réservé à ceux des bénéficiaires de l'offre spécifique et du droit au compte, dont la situation financière et la plus délicate, les plafonds spécifiques seraient ainsi réduit de moitié. Lorsque le flux créditeurs mensuelle calculée selon une moyenne semestrielle est inférieur à un seuil fixé par arrêté. Je précise que cette, ce dispositif est immédiatement opérationnel puisque certaines banques par exemple, la Banque Postale utilisent déjà l'indicateur du flux créditeurs mensuel pour déterminer le niveau de fragilité financière de leurs clients. Telle est l'objet de cet amendement. Merci monsieur le rapporteur. Votre avis donc sur l'amendement Oui madame la présidente. Donc sur l'amendement IV. Qui. Sur lequel je me je donnerai un avis défavorable. En demandant à son auteur de bien vouloir se rallier à l'amendement 21 de la commission pour 3 raisons, d'abord parce que son dispositif vise les commissions d'intervention, alors que son objet vise les frais d'incident. Ensuite parce que si le Sénat souhaitait plafonner les frais d'incident pour l'ensemble des Français il courait le risque de méconnaître la liberté tarifaire des établissements de crédit et partant la liberté d'entreprendre. Enfin par qui concerne spécifiquement le plafonnement des frais d'incident applicable aux bénéficiaires du droit au contre et de l'offre spécifique. L'amendement de la commission est à la fois plus plus large puisqu'il concerne également les frais de gestion et plus opérationnel. C'est la raison pour lesquelles donc j'invite l'ensemble de mes collègues qu'il souhaite plafonner les frais bancaires avec efficacité mais sans. Excès comme nous avons pu en débattre en commission à voter l'amendement 21 de la commission, je vous remercie. Merci. L'avis du gouvernement sur ces deux amendements. Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, dans la mesure où nous étions favorables à un retrait de cet article nous sommes défavorables à ces deux amendements. Merci. Monsieur,

Assez plafonnement pour les ménages très modestes mais il y a aussi. Tous ces ménages de travailleurs pauvres qui sont exclus du dispositif qui se lève le matin pour aller travailler,

le compte est à découvert. Je suis encore rejeté, il aurait fallu chaque de France à l'euro et la Banque leur met 50 euros de frais. Je trouve ça inadmissible. Alors moi ce qui me gêne un peu, c'est qu'on va plafonné pour les plus fragiles et il faut plafonner pour les plus fragiles. Mais il y a aussi les fragiles qui ne sont pas très fragile mais qui travaille dur, qui a valu une flashmob leur pouvoir d'achat Béchir. Il me semble qu'les oublie un peu. Merci Monsieur paru juste ce que vous retirez votre amendement. Oui je le retire puisqu'il est satisfait par le 21. Merci. Donc j'ai vais mets aux voix l'amendement 21 de la commission qui a reçu un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui ça. Tiens il est donc adopté l'article 4 est ainsi rédigé et voté. À l'article 5 que le l'amendement 17. Monsieur Wade blé. Oui cet article vise à créer une autorisation de découvert sans frais proportionné aux revenus des clients bénéficiant d'une offre spécifique. Cette permission ce pourrait s'avérer contre-productive et dans la mesure où l'offre spécifique doit des les publics les plus précaires à mieux gérer leur budget. C'est pourquoi s'amendement vise à supprimer cet article. Merci l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur.

me semble néanmoins que l'adoption de cet amendement empêcherait la discussion de l'amendement de la commission de réécriture de l'article 5, qui supprime également le droit au crédit au profit d'une clarification du droit existant et donc ça sera une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Même avis. Merci je mets donc aux voix l'amendement 17 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient donc pas s'adopté. En si nous savons un amendement et un sous-amendement alors le 22 monsieur le rapporteur. Au terme de l'article L. 312 1 tiré 3 du code monétaire et financier. Les personnes identifiées comme fragiles se voient proposer de souscrire une offre spécifique qui vise à prévenir la survenance d'incidents et le cas échéant à limiter les frais d'incident qui leur sont facturés le contenu minimal de cette offre spécifique défini par le législateur est précisé par le pouvoir réglementaire ne comporte pas d'autorisation de découvert. Cependant la souscription de l'offre spécifique ne fait pas Anne elle même obstacle à l'ouverture au maintien d'une autorisation de découvert. Si la situation du client fragile concernés le permet. Or l'objet de l'article 5 de la présente, proposition de loi et d'inscrire une autorisation de découvert sans frais proportionné aux revenus des personnes concernées dans le contenu minimal de l'offre spécifique, cette proposition ne saurait être retenue, d'une part parce qu'elle reviendrait à créer un véritable droit au crédit gratuit, je l'ai indiqué tout à l'heure et d'autre part parce qu'elle offre. Parce que l'offre spécifique vise spécifiquement les publics fragiles dans lesquelles l'accumulation de découvert pourraient rapidement aboutir à une aggravation de leur fragilité. Toutefois, il apparaît utile que le législateur mentionne explicitement la possibilité de bénéficier d'une autorisation de découvert. Même en ayant souscrit l'offre spécifique. Si la situation du client concerné le permet. Les bénéficiaires de l'offre spécifique pensant souvent que ce n'est pas le cas donc. Telle est l'objet de cet amendement, c'est d'inscrire de manière explicite. Dans la loi cette possibilité du maintien. De du. Le truc. Merci. Le sous-amendement 27 monsieur Alors ce sous-amendement complète l'amendement de monsieur le rapporteur, en encadrant de manière stricte par le Conseil d'État. Les critères pris en compte par les établissements bancaires pour déterminer si un client est en situation de fragilité financière en effet depuis 2013 la reconnaissance de qualité de fragilité financière est fondée sur des critères dont l'appréciation est en partie laissée aux banques que cette mesure permettrait ainsi d'assurer un traitement égal à tous les citoyens.

Que nous avons eus en commission des finances, donc pour aboutir à ce à ce sous-amendement de notre propre amendement et et en conséquence la commission a considéré que cette proposition constituait un bon compromis entre l'objectif d'harmonisation des critères retenus par les banques et une certaine flexibilité dans la détermination de de de ses caractéristiques. Et donc elle vous propose de retenir ce sous-amendement avec un avis donc favorable de la commission. Et si l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre sur l'amendement et le sous-amendement. nous nous étions favorables à. À l'amendement de de monsieur le rapporteur. Mais s'il les a ajouté le le sous-amendement, nous y sommes défavorables. Merci. Alors Monsieur Féraud. Merci. Pour notre part nous sommes favorables au sous-amendement dans le cadre de l'amendement. Et alors que le gouvernement ne soit pas favorable au sous-amendement. Quel aveu par rapport à une volonté de réglementer mais aussi d'avoir des critères qui soient beaucoup plus uniforme et objectifs entre les différentes banques et les différents clients néanmoins nous. Je regrette cet amendement parce que. Franchement. La souscription de l'offre spécifique ne peut seul faire obstacle à l'ouverture au maintien d'une autorisation de découvert. Je pense que la banque trouvera bien un autre argument. Dans les faits ça ne changera rien. Je ne crois pas que notre proposition soit. Relève du droit au crédit. Elle relève. Véritablement de presque de la vie pratique, concrète et les cas dont parlait Christian Billac tout à l'heure, c'est-à-dire d'éviter que quelqu'un qui a fait un chèque de 60 euros le 12 soit. Quand le chèque est encaissé le 22 né son compte débiteur et le compte rejetée en ayant justement une autorisation de découvert minime qui permettent d'éviter des incidents et derrière d'éviter des frais liés aux incidents donc pour notre part, nous voterons contre l'amendement du rapporteur. Merci. Alors je vais mettre aux voix, donc le sous-, amendement 27, qui a reçu un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui pour.

Qui est contre qui s'abstient. Il est donc. Adopté l'article 5 est ainsi rédigé article 6. Amendement 25 du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente. Si le gouvernement a déposé des amendements. Ce matin, c'est que nous attendions l'ensemble des des amendements et certains ont été déposées ce matin. Et et les amendements du gouvernement était déposés dans la demi-heure qui suivait le dépôt des derniers amendements. Y compris ceux du rapporteur Monsieur le Sénateur, pour revenir à à l'amendement du du gouvernement la protection des des consommateurs notamment des des plus vulnérables constitue une préoccupation. Majeure du du gouvernement. Le dispositif de plafonnement actuel s'il peut. C'est. Pardon. Monsieur le Ministre, la parole. C'est le c'est le même texte que tout à l'heure. Pardon. Excusez-moi, le dispositif de plafonnement actuel s'il peut être encore amélioré à l'Avantage de concilier efficacité dans son ciblage et simplicité dans sa mise en oeuvre ainsi le dernier rapport de l'Observatoire de l'inclusion bancaire publié en 2022. Fait notamment état d'une baisse importante des frais facturés aux clients fragiles par rapport par ailleurs le rapport de 2022 de l'Observatoire des tarifs bancaires. Indique sur les principaux frais appliquer à l'ensemble de la clientèle 8 tarifs. Sur 14 sont stables et un tarif est en baisse. À l'inverse, la mesure, telle qu'envisagée par l'article 6 de la proposition de la loi aboutirait à ce que tous les frais appliqués par les banques aux bénéficiaires de l'offre spécifique et de la procédure de droit au compte soit limité à un tiers du montant mentionné sur la plaquette tarifaire plus plafonné par mois et par opération à géométrie variable selon les revenus du client. Une telle mesure irait à l'encontre de l'objectif de meilleure protection des clients les plus fragiles en effet les grilles tarifaires étant très variables suivant les banques et leur clientèle plafonner les tarifs des publics fragiles au tiers des tarifs généraux pourraient conduire à des situations de plafonnement extrêmement variable d'une banque à l'autre. Par ailleurs cette mesure associe à un plafonnement modulée en fonction des revenus rendrait très complexe et peu lisible. La mise en oeuvre de ce nouveau régime d'encadrement au risque de moins bien protégés des publics aujourd'hui déjà couvert. Le gouvernement propose donc de conserver le régime législatif actuel et la flexibilité bancaire associés permettant de paramétrer les différents plafonds de frais. Je vous remercie. ça va être un avis personnel sans sans faire de commentaires sur les dépôts des des des amendements. En revanche, ça sera un avis, une demande de retrait au profit de l'amendement 23 de la commission, ou à défaut un avis défavorable en effet le dispositif qui est proposée à l'article cite est certes très ambitieux peut être trop et il faudra le modifier pour éviter les effets de bord mais pour autant sa logique est la bonne, il convient d'éviter une compensation ou du moins à risque de compensation par les banques du plafonnement, introduit à l'article IV par une hausse sur les autres frais donc comme par parallélisme des formes. Je je propose là aussi un. Un avis défavorable à l'amendement du gouvernement, de façon à ce que l'amendement 23. De la commission qui vient modifier l'article 6 et limite son compte tenu un plafond par opération. J'aurai l'occasion de le présenter dans un instant répondent à cet objectif de manière il nous semble plus proportionnée et plus opérante donc un avis défavorable. Une demande de retrait ou un avis défavorable. Merci monsieur Bachar. Monsieur le Ministre. Honnêtement. Dire que vous attendiez le dernier moment pour proposer un amendement de suppression d'articles. Non mais ça n'existe pas ça. Monsieur le Ministre pas vous n'avez pas assez d'expérience parlementaire, je le crains. Ces arguments bah si je suis obligé de vous le dire. Bah si. Bah non. Historiquement. Le gouvernement, il pose les amendements les examinent en commission il attend pas le texte de la commission. Ça c'est effectivement les réformes. Constitutionnelles qui ont eu lieu depuis quelques dizaines d'années. Désolé de vous le dire. Donc, non ce n'est pas les principes, vous n'avez pas travaillé pour faire l'amendement de suppression ce n'est pas du travail, le travail ça aurait été de pour faire une proposition alternative et là on aurait pu comprend il n'y a pas de travail je suis désolé vous dit tout va bien. Et donc il n'y a pas besoin de cet article et a pas besoin de cette loi et donc on le met à la dernière minute. Vous l'auriez mis normalement en disant on ne veut pas de ce texte on l'examiné, on a eu un examen normal au Parlement, je suis désolé vous méprisez une fois de plus. La procédure parlementaire. Merci. Alors je mets aux voix donc l'amendement 25 du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission. Qui ont qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient mais donc pas adopté l'amendement 23 de la commission. Monsieur le rapporteur. Oui madame la présidente, donc j'ai déjà évoqué en partie l'objet de de de 16. Cet amendement. Je ne vais pas revenir sur la proposition initiale. Qui propose que pour les bénéficiaires du droit au compte ou de l'offre spécifique que l'ensemble des frais de gestion et des frais d'incident soit limité à un tiers des tarifs appliqués. Un tel dispositif nous semble à la fois peu lisible et difficile à mettre en oeuvre ce dispositif apparaît au demeurant contestable sur le fond en effet une limitation des frais par mois apparaît contestable au regard des mécanismes existants qui ne prévoit que que des plafonds par opération, en particulier pour les frais de gestion. Qui correspondent à des services rendus. J'ai déjà eu l'occasion de le dire en conséquence par cet article, ou les auteurs souhaité éviter que les banques ne compense une baisse de certains frais résultant du plafonnement, par une hausse des frais non plafonné. On en partage les objectifs en conséquence le présent amendement de la commission propose, outre quelques modifications d'ordre logistique, l'instauration d'un principe de plafonnement par opération des principaux frais bancaires qu'il s'agisse de frais de gestion ou d'incidents réservé aux bénéficiaires de l'offre spécifique et du droit au compte. Merci l'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Comme je l'indiquais dans dans notre amendement. Le cadre actuel permet d'atteindre les objectifs qui sont proposés dans ces dans ces amendements à la fois une offre spécifique de frais de tenue de compte comme les frais d'incidents sont déjà plafonnées et et cette offre spécifique peut se concilier avec le droit au compte, donc compte tenu de de de ces éléments nous sommes défavorables à cet amendement. Merci Monsieur Féraud. Merci madame la présidente. L'amendement du rapporteur permet d'aller dans le même sens que notre proposition peut être de manière là aussi plus pertinente. Mais je remarque que notre proposition n'avait pas besoin de passer par un décret du gouvernement la proposition du rapporteur nécessite de passer par un décret du gouvernement. On voit dans ce débat le volontarisme du gouvernement en la matière donc. Voilà, si cette. Proposition Proposition de loi a été adoptée avec l'article. L'amendement du rapporteur. J'espère que le gouvernement le mettrai en oeuvre avec plus de volontarisme qu'il n'en a montré dans ce débat. Merci. Alors je mets aux voix donc l'amendement 23 de la commission qui a reçu un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour. Ces contrats qui s'abstient. Il est donc adopté, je me vois l'article 6 qui est pour. Contre qui s'abstient. Il est donc adopté. Après l'article 6 Monsieur Paris pour l'amendement six. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, la prolifération ne frais facturés pour différents types de procédures et d'incidents pèse lourdement sur les contribuables et la protection des plus modestes demeure limité. C'est pourquoi cet amendement vise à plafonner les frais bancaires en divisant par deux les frais pour rejet de chèque ainsi que pour tout autre incident de paiement pour l'ensemble des clients. Il met en place des plafonds spécifiques pour les clients, placés en situation de fragilité financière avec des limites correspondant au quart des montants fixés pour l'ensemble des autres clients. Merci l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Il s'agira d'une demande de retrait ou d'un avis défavorable à cet amendement qui diminue les plafonds applicables aux frais de rejet de chèque et aux frais de rejets de prélèvements et de virements. D'une part pour tous les Français et d'autre part pour les personnes en situation de fragilité. en ce qui concerne l'ensemble des Français les frais concernés sont déjà plafonné. Par décret. Et et et on la portée du texte ne concerne pas l'ensemble des Français. J'ai eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure en ce qui concerne les personnes fragiles. Le présent amendement nous semble redondant avec l'amendement. Que j'ai proposé à l'article 6 et. Qui était me semble-t-il préférable pour 2 raisons, d'abord plus ambitieux puisqu'il concerne l'ensemble des frais bancaires et pas seulement les frais de rejet de chèques ou de prélèvements de virements et parce qu'il me semblait mieux cibler non sur l'ensemble des personnes fragiles mais spécifiquement sur celle qui bénéficient du droit au compte, ou qui ont fait le choix de souscrire l'offre spécifique. Donc une demande de retrait ou un avis défavorable. Si l'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Même avis que monsieur le rapporteur. Merci. Est-ce que vous retirez monsieur Paretti non. Donc je mets aux voix l'amendement six qui a reçu donc un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour.

Nous débattions il y a quelques temps dans cet hémicycle d'un texte visant selon les auteurs à renforcer la protection des épargnants. Celui-ci porte l'ambition de l'inclusion bancaire thème très important. Pourtant aucune disposition de ces deux textes ne concernent les livrets d'épargne réglementée. Pourtant en 87 millions de livrets de ce type Livret A LDDS livré l'épargne populaire sont ouverts pour un encours total de 486 milliards d'euros. Voyons ce que nous dit la la Cour des comptes sur ce sujet je cite. L'épargne réglementée constitue une particularité française qui a peu d'équivalent en Europe et qui s'explique par l'histoire financière et par l'importance des dispositifs réglementaires visant à encourager et protéger l'épargne des ménages et l'offre à ces derniers des produits simples bénéficiant de la part de l'état d'une garantie sur le capital et d'une rémunération évolue évolue en fonction de l'inflation. Pour le système financier. Elle constitue une ressource stable et contribue à transformer les dépôts des épargnants en emplois d'intérêt général de long de citation. Cet amendement près propose élargir aux bénéficiaires du livret d'épargne populaire et, et de rendre sa présentation obligatoire aux épargnants qui sont éligibles. Il est emblématique de ce qui est un produit d'épargne protecteur rémunérateur car indexés sur l'inflation sécurisant par des dépôts garantis liquide et proposant une fiscalité également avantageuse. Alors que les clients les plus aisés et bénéficient de diverses. Remises commerciales et des supports défiscaliser les clients les plus modestes subissent eux la double peine, plus de frais et une épargne moins rémunératrice pourtant comme pour les aides sociales le non recours au livret d'épargne populaire et massif. L'Observatoire de l'épargne réglementée a établi dans son rapport annuel publié en juin 2019 que seuls 21% des individus éligible détiennent à L E P alors que parmi les personnes éligibles non-détentrice de LEP la moitié détient un livret A, d'où le sens de cet amendement. Si l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Oui merci madame la présidente. Cet amendement. Vise en effet à systématiser la proposition de l'ouverture d'un livret d'épargne populaire aux clients en situation de difficulté financière qui satisfont les conditions de revenu fiscal de référence monsieur Bocquet, la la rappeler, cet amendement avait déjà été déposée par le groupe communiste dans le cadre de l'examen de la PPL, protection des épargnants et la commission s'était prononcé en faveur du retrait de de l'amendement en effet. On rappelle que selon l'article L. 221 15, l'ouverture d'un livret d'épargne populaire est réservé aux épargnants dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un certain seuil, aujourd'hui c'est le contribuable qui fait la démarche de demander l'ouverture de se livrer en revanche pour déterminer l'éligibilité au. D'une personne comme le prévoit le présent amendement l'établissement de crédit, devraient avoir accès à son revenu fiscal de référence qui soulève les difficultés et pose notamment la question de la confidentialité des informations. Il me semble que c'est plutôt à l'administration fiscale d'informer le contribuable de son éligibilité à l'épargne populaire ainsi chaque année la DGFIP délivre une information qui gagnerait peut-être même sans doute à être mieux. Par exemple en figurant sur l'avis d'imposition peut-être Monsieur le Ministre pour nous éclairer sur cette évolution là, donc en clair, il nous semble que c'est plutôt. Au-delà de la démarche de l'épargnant à l'administration fiscale. D'informer les bénéficiaires de leur éligibilité en conséquence de quoi il vous est proposé soit en retrait ou à défaut un avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Même avis que monsieur le rapporteur. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 14. Qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient mais donc pas adopté. L'amendement six madame Vermeillet. Merci madame la présidente. Cet amendement de Michel Canevet vise à protéger les personnes en situation de fragilité, eu égard notamment au montant de leurs ressources en appliquant des taux d'intérêts débiteurs ne pouvant dépasser le taux d'usure. Il s'agit d'éviter des solutions coûteuses pour des personnes qui font face aux aléas de la vie et qui connaissent déjà bien souvent des difficultés financières. Compte tenu des contraintes d'encadrement du recours au crédit. Merci. Merci. L'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Cet amendement, nous semble d'ores et déjà satisfait. En effet, le taux d'usure se défini au terme de l'article L. 314 6 du code de la consommation comme le taux d'intérêt maximal légal par définition les intérêts débiteurs du lorsqu'un compte se trouve à découvert sont donc obligatoirement inférieur au taux de l'usure, parce que je partage la Commission partage néanmoins l'objectif de mieux encadrer les intérêts débiteurs et vous le savez, le taux d'usure et parfois fixé relativement haut en particulier sur les prêts dont le montant est faible. Cela peut paraître excessif pour des clients fragiles en conséquence l'amendement à l'article 6 présenté par la Commission prévoit justement un plafonnement de nombreux frais bancaires qui répondent aux mêmes objectifs et au nombre desquels figurent les intérêts débiteurs pour protéger davantage nos concitoyens les plus fragiles, a donc une demande de retrait parce que satisfaits ou à défaut un avis défavorable. Merci. L'avis du gouvernement. Même avis. Merci madame Vermeillet. Je partage l'avis du rapporteur je retire l'amendement. Alors à l'article 7 l'amendement 24 de la commission. Monsieur le rapporteur. Le présent amendement comme je l'avais indiqué, dans la discussion générale vise à supprimer l'article 7 qui prévoit d'obliger la commission des sanctions de la CPR a adopté une sanction pécuniaires à l'encontre des établissements de crédit qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière de droit au compte, ou qui n'appliqueraient pas la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement en effet l'objectif visé par cet article est en grande partie satisfaits puisque la commission des sanctions de l'ACPR dispose déjà en matière de droit au compte de respect de la charte d'inclusion. D'un pouvoir de sanction, y compris pécuniaires toutefois la modification introduite. En prévoyant donc que la commission des sanctions est tenu de prononcer une sanction nous semble excessive. Conformément au principe de proportionnalité et de gradation des sanctions. La commission des sanctions de la CPR doit pouvoir rester souveraine dans le choix de la mesure la plus adaptée à la situation. Je rappelle également. Que la publication des décisions sous forme nominative déjà pratiqué par l'ACPR. Paraît avoir davantage d'impact encore qu'une sanction pécuniaire pour les établissements de crédit et qu'elle a été dans les années qui viennent se passer activé au moins à 3 reprises. Dans au au à l'encontre de d'établissements bancaires qui n'avait pas respecté la charte. La proposition de la Commission et donc à travers cet article de supprimer l'article 7. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur Ministre. Même avis de suppression de cet article 7. Vous êtes pas favorable. Merci. Alors donc je mets aux voix l'amendement de la commission qui a reçu un avis favorable du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est donc adopté l'article 7 est supprimé après l'article. Me suis par Engie pour l'amendement la la présidente chers collègues cet amendement souhaite apporter quelques modifications au droit au compte. Afin d'accompagner les clients les plus précaires. Ainsi, il prévoit une procédure d'ouverture de compte en 2 temps. Tout d'abord, les banques ne pourront demander que des documents strictement nécessaire entendu comme des. Les informations requises par la Banque de France. Puis, une fois le compte ouvert, il sera toujours loisible de demander des informations complémentaires pour respecter leurs obligations. Si l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Oui là aussi nous avons eu un, un débat en commission et je remercie monsieur Paretti d'avoir modifié son son amendement. Et, et en conséquence, l'avis de la commission sera favorable après les rectifications apportées cet amendement cherche à trouver un juste équilibre entre les obligations contradictoires qui pèse sur les établissements de crédit en matière de droit au compte d'une part et en matière de connaissance de leur clientèle. D'autre part, d'une part, lorsqu'un établissement de crédit est désigné par la Banque de France pour ouvrir un compte au titre du droit au compte. Il doit bien sûr le faire dans les meilleurs délais. D'autre part pour satisfaire à ses obligations de vigilance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ce même établissement de crédit doit parfois requérir de nombreuses pièces justificatives. Ce qui peut retarder effectivement l'ouverture d'un compte. La Cour des comptes avait relevé une réticence croissante des établissements de crédit depuis 2018 à satisfaire à la procédure du Dac au nom de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les documents complémentaires demandées par Bank doivent en effet être transmis avant l'ouverture du compte, le présent amendement permet de décaler la transmission de ces documents complémentaires après l'ouverture du compte, afin de permettre son ouverture dans des délais plus courts mais toujours avant la première opération sur le compte. Il répond ainsi à une problématique bien identifié, tout en conservant un réel garde-fous. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable à cet amendement ainsi rectifié. Merci. Il avait du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, la réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme imposé un ensemble d'obligations aux établissements de crédit lors de l'entrée en relation avec un client certaines modulations dans la mise en oeuvre de ces mesures de vérification sont prévues par le droit européen c'est modulation qui peuvent notamment conduire au différé de la vérification de l'identité du client ne peuvent cependant qu'être justifié par le degré de risque de la clientèle. Toutefois l'amendement vise à aménager la procédure du droit au compte, afin de l'inscrire dans une situation de faible risque de LCB Tiret FT c'est cet aménagement n'est donc absolument pas conforme à l'esprit du droit européen ni à l'esprit des recommandations du Groupe d'action financière, par ailleurs, la loi numéro 2020. Un tiret 1774 du 24 décembre 2021. Vidant visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle. Dis toi loi Rixain et il est désormais possible à toute personne de mobiliser la procédure même si cette personne dispose déjà d'un compte joint. Cette évolution bénéficie en particulier à toute personne victime de violence conjugale et potentiellement co-titulaires d'un compte avec son conjoint maltraitant lui permettant de saisir directement la Banque de France pour activer un droit au compte. Dans une perspective d'émancipation. Par conséquent nous sommes défavorables à cet amendement.

de violence conjugale, c'était dans le le les premiers éléments de l'amendement, mais ça a été retiré puisque satisfait comme vous venez de le rappeler, Monsieur le Ministre. Donc c'est plus l'objet de de l'amendement qui est présenté. Nous sommes tout à fait conscience que cet amendement même rectifier ne donne peut-être pas encore pleinement satisfaction d'un point de vue technique. Pour autant, il nous semble, qui va dans le bon sens et a le mérite d'engager une discussion, notamment pour ce public fragile qui seraient rassurés par une telle mesure je fais confiance à la délibération parlementaire et à la navette entre le Sénat et l'Assemblée pour encore l'améliorer et lui permettre d'être tout à fait opérant. C'est pourquoi je maintiens, un avis favorable sur cet amendement. Merci donc je mets aux voix l'amendement qui a reçu un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui. Pour. Qui est contraint qui s'abstient. Il est donc adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Donc Monsieur Féraud. Merci madame la présidente pour une explication de vote sur l'ensemble de la proposition de loi si c'est bien si c'est bien le moment avant que nous passions vote évidemment nous regrettons que les articles 1 et 2 sur. L'accessibilité bancaire territoriale été. Entièrement supprimée au moins. Aurons-nous lancer le débat je suis sûre qu'il rebondira ici même. Dans l'avenir, je pense que un certain nombre d'interventions montrent que la réflexion a besoin d'avancer sur cette question. Ensuite pour dire que nous voterons favorablement au texte issu de nos débats, parce que même si ces articles 1 et 2 ont été supprimés. Ce qu'il reste du texte en matière d'inclusion bancaire et ah non négligeable. Je veux remercier le rapporteur de son travail. Je pense que l'adoption de cette proposition de loi, j'espère qu'elle pourra ensuite poursuivre son chemin parlementaire montre qu'il y a besoin de mieux protéger les Français en situation de fragilité face à l'ensemble des frais bancaires que la réglementation existe que les pratiques se sont certes améliorés mais bien trop peu, bien trop lentement qu'il reste encore beaucoup trop d'illisibilité des frais bancaires dans notre pays que cette illisibilité d'ailleurs a tendance à encore s'accroître et que par ailleurs le fait que nos concitoyens les plus modestes participe autant au 25 milliards d'euros dans leur ensemble des frais de gestion et des frais bancaires dans notre pays. Ça n'est pas acceptable, c'est une redistribution à l'envers. Et cette une difficulté supplémentaire pour ceux qui sont déjà en difficulté donc j'espère que cette proposition de loi permettra de faire avancer la législation en la matière et une fois encore merci au rapporteur de son travail. Merci monsieur le rapporteur général. Oui madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, quelques mots effectivement également d'explication de vote moi aussi pour saluer le travail collectif en commission et dans l'assemblée et remercié peut-être plus particulièrement le rapporteur Stéphane Sautarel qui. A eu un temps de travail très court mais dont je je crois chacun apprécie à la fois la qualité d'écoute, de dialogue et la recherche de points de convergences sur une proposition de loi dont le thème. Est éminemment important je dirais peut-être plus. Encore Encore en s'étant, je le disais tout à l'heure lors de la séance des questions au gouvernement de tension sociale. La question de l'accessibilité de l'inclusion bancaire, je veux faire de remarque particulière sur l'accessibilité. Je veux vous informer que j'ai demandé à priori nous obtiendrons rapidement de la Banque de France a porté à connaissance national avec des cartes départementales sur les points d'accès à la fois au distributeurs mais pas seulement évidemment ce que l'on souhaite, c'est d'avoir ce que une toile d'araignée qui nous permet, qui nous permettent en tous les cas, de bien travailler pour être dans la stratégie du zéro zones blanche en terme d'accessibilité aux espèces et sur le sujet de l'inclusion bancaire. Je pense que le travail que nous avons à nouveau conduit ensemble ici permet d'avancer cet important et Monsieur le Ministre, je crois que vous, ça a été dit. Je pense qu'en tous les cas vous partagez. Les orientations même si vous avez, malheureusement je crois parfois rendu des avis défavorables et maintenant je pense que il appartient aussi au gouvernement. De s'emparer de de ce dossier de ce texte pour le faire prospérer. Ce serait d'abord une reconnaissance supplémentaire et je crois que le Parlement. On a besoin de l'utilité des travaux dans les semaines d'initiative parlementaire, dans les 2 assemblées donc la balle est dans votre camp, je compte évidemment sur le gouvernement pour faire prospérer ce texte. Merci monsieur Savoldelli. Merci madame la présidente. C'est aussi une explication de vote. Sur la loi initiale déposée. Nous avions un vote très favorable. Avec des arguments et avec des amendements dont certains ont été comme d'autres d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure il y recevable. Moi je vais vous dire, je pense que la question du fonds de garantie nous aidait à ce que vient de dire aussi le rapporteur général qu'on ait la vraie cartographie. Et qu'on mette à plat la réalité de ce que vivent les Français. Vous savez ce que c'est, on a des. On va à un guichet, vous avez une gratuité si c'est pas votre banque de plusieurs tirages et après vous payer des frais. Si le DAB n'est pas liée à votre banque de dépôt. Donc il y a rien qui est gratuit dans cette histoire après. Moi je vous le dis, je pense que c'était c'était initiative vraiment intéressante et il y a eu un débat, moi je. Nous nous trouvons intéressant. On aurait souhaité que le gouvernement encourage ce débat parlementaire franchement avec des amendements avec des enrichissements voilà ça me paraissait juste. Je pense qu'on aurait dû retenir d'autres idées, ça a été dit par Biya tout à l'heure, c'est dit. Il a raison, il y a des salariés pauvres aurait été pas mal d'élever l'accès à l'épargne populaire. Voilà, vous voyez, il y avait plusieurs dispositions qu'on aurait pu mettre en place. Qui n'ont pas été retenus. Nous avions aussi souhaité que les collectivités territoriales soient pas une nouvelle fois mis à contribution ne l'avait dit d'ailleurs à nos collègues socialistes on n'est pas que les collectivités, on pense que les banques peuvent le faire, je le redis la hein vraiment hein. Je vous dis ça pour qu'on, qu'on ne mette pas du désordre puisqu'il n'y en a dans la société. Mais quand il y a 6, 5 milliards de frais d'incident ramassés par les banques. Excusez-moi, ils peuvent participer à l'effort de l'accessibilité et de la collusion bancaire. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce projet de loi. Merci. Merci. Alors je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer l'accessibilité et l'inclusion bancaire. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est donc adopté alors je vais suspendre la séance pour quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour. La séance est suspendue.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle à discussion de la proposition de loi visant à résorber la précarité énergétique présentée par Monsieur Rémy Cardon mesdames Viviane Artigalas, Catherine Conconne, Annie Le Houerou et plusieurs de leurs collègues. C'est une demande du groupe socialiste, écologiste et républicain dans la discussion générale. La parole est à monsieur Rémy Cardon, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre. Madame la rapporteure, mes chers collègues. Antoine de Saint-Exupéry, nous disait nous héritons pas de la terre de nos parents nous empruntons à nos enfants. Et dans quel état. Allons nous rendre la Terre à nos enfants. La science est unanime, les effets du changement du changement climatique se font de plus en plus pressants de plus en plus dramatique. De plus en plus irréversible. Nous sommes conscients des dangers. Nous savons qu'il reste peu de temps pour inverser la situation et Inde et endiguer les conséquences désastreuses d'un réchauffement global. Oui, mes chers collègues. Est plus que temps d'agir. Cette proposition de loi. Il y en a vécu des habitants de mon département et du vôtre. Ou encore des retours d'expérience des associations qui sont fortement mobilisés. Elle se veut être une première réponse aux dysfonctionnements et aux fringues qu'ont constaté sur le terrain. Évidemment. Elle n'a pas la prétention de résoudre tous les problèmes de la politique de rénovation énergétique. Mais elle permet de traduire un corpus de mesures applicables immédiatement et qui nous permettrait d'avancer concrètement. Et je souhaite exprimer le regret de mon groupe, sur le sur le rejet de ce texte en commission sans avoir même tenté ni proposé de l'amender. Il y aura donc aucun signal positif envoyé ce jour par au Sénat par le Sénat à des milliers de Français qui souffrent de la précarité énergétique et été comme et été comme hiver. Oui. Les travaux de la commission d'enquête sur le la rénovation thermique sont nécessaires et je salue d'ailleurs. Mes collègues du groupe geste de leur initiative et des propositions qui ne manqueront pas de faire dans les prochains mois. Mais mais là n'empêche pas l'autre. L'urgence ne nous permet plus de rester figé dans l'immobilisme d'objectifs toujours plus ambitieux sans mettre les moyens pour les atteindre. L'exemple du Grenelle de l'environnement et parlant. Si les objectifs de rénovation énergétique prévu en en 2008 avait été tenu. La France économiserait déjà l'équivalent de ses importations de gaz russe et des millions de gens seraient sortie de la précarité énergétique. Logement correspond. Au secteur le plus consommateur d'énergie, avec le transport et représenterait plus de 18% des émissions de gaz à effet de serre en France, il correspond d'ailleurs au 1er poste des dépenses des ménages pourtant. Les efforts pour adapter nos logements aux nouveaux défis du siècle, reste insuffisant. L'été les épisodes caniculaires s'enchaînent et se de plus en plus fréquent. Cela induit pour les foyers les plus chanceux disposant d'une climatisation. Une consommation d'énergie accrue pour refroidir les logements pour les autres. Et températures grimpent très vite à l'intérieur, faute d'isolation efficiente l'hiver. Les 6 millions passoires thermiques du pays ne permettent pas à leurs occupants de vivre dignement. Qui puiser dans un contexte en plus d'envolée des prix de l'énergie, les foyers les plus fragiles sont confrontés à un choix cornélien. Se priver ou s'endetter pour se chauffer. Et que dire des maladies induites bronchites à répétition asthme. Nous sommes donc confrontés à plusieurs enjeux majeurs, d'abord un enjeu social. En diminuant les dépenses énergétiques des ménages et en améliorant leur confort de vie ensuite un enjeu de santé publique. Et enfin un enjeu environnemental en permettant à la France de respecter ses engagements climatiques dans le cadre des accords de Paris. Alors oui des avancées sont intervenues ces dernières années mais les résultats ne sont pas à la hauteur et beaucoup reste à faire d'ailleurs. Selon la Cour des comptes sur les 700.000 subventions MaPrimeRénov débloquer en 2021 le nombre de logements sortis du statut passoires thermiques initialement annoncé à 80.000 par le gouvernement finalement a été ramenée à 2500. À ce rythme là il faudra plus de 2000 ans pour rénover les 6 millions, pas sûr thermique du pays vous le savez à l'urgence climatique c'est c'est ajouter avec une inflation délirante. L'urgence économique et sociale. D'ailleurs, la Fondation Abbé Pierre nous le rappeler encore hier lors d'une table ronde, que tous les indicateurs de rénovation globale était en baisse en 2022. Je peux vous dire, mes chers collègues que nous partageons un certain nombre de constats issus des remontées de terrain des auditions que nous avons menée conjointement, ici même au Sénat, mais trop peu de personnes s'engage dans une dans un parcours de rénovation globale et performant Les raisons de la non-massification des rénovations globales et performante sont multiples. Et pourtant. Les moyens ont été engagés. Plus de 3,4 milliards d'euros ont été distribués par l'année en 2022 et les mais les freins sont encore trop nombreux.

988 euros et 1267 euros par personne. Mes chers collègues. Combien faudra-t-il de rapport alarmant pour s'attaquer à la précarité énergétique et au mal-logement des plus modestes. Notre proposition ne vise pas à créer de nouveaux dispositifs de nouvelles normes. Elle vise simplement à réaffecter les moyens dont nous disposons au bon endroit et à cibler prioritairement les personnes qui aujourd'hui ne vivent pas dans la dignité. Comme nous le disent de nombreux rapports. Ainsi, nous pourrions éradiquer les passeurs thermiques en 2030 plutôt qu'en cas en 4020. Mes chers collègues. Il y a une urgence à changer de cap et à revoir le pilotage de la politique de rénovation énergétique. un d'ailleurs dans un contexte, je l'ai dit où les tarifs de l'énergie sont toujours plus élevés. Il y a urgence également car les logements les plus énergivores vont disparaître du marché de la location faute de rénovation. La crise du logement ne frappera pas que les grandes villes, les ménages qui s'imposent les plus grandes restrictions habite parfois dans nos communes rurales. Et les bourgs de moins de 20.000 habitants. En cumulant interdiction progressive de la location des passoires thermiques et les effets d'Usain nos communes rurales. Pourraient être. À voir se multiplier des éléphants blancs d'un d'un nouveau type et de devenir des musées à ciel ouvert de l'habitat d'antan. Vous l'aurez compris, il est urgent d'agir. Et ce, sans forcément attendre la nouvelle feuille de route du gouvernement. Alors oui, la révision de la. De la stratégie française sur l'énergie et le climat doit être l'occasion de clarifier, Monsieur le Ministre, dans les prochains mois les priorités d'actions de notre pays d'établir une stratégie de rénovation des logements et de lutte contre la précarité énergétique plus performante et plus ambitieuse. encore plus de temps car le terrain. C'est en tout cas sur le terrain les retombées. On voit que ça ne fonctionne pas bien. J'ai ainsi en tête ce couple de retraités dans mon département de la Somme qui a engagé des travaux de rénovation globale dans son logement. À l'heure où je m'adresse à vous. Les travaux sont terminés depuis plusieurs mois. Malheureusement ce couple n'a toujours pas reçu sa subvention de MaPrimeRénov'. Ils ont dû ils ont dû contracter un prêt à taux de 15% pour pouvoir avancer les travaux et surtout pour être en capacité de continuer à se nourrir. Je pense également à cette personne qui après avoir été constamment démarchés par des commerciaux a fini par accepter son que son logement soit rénové dans l'espoir de voir ses factures baisser. Que ne fut pas son désarroi quand elle s'est rendue compte. Que les travaux a été avait été bâclé que la société qui avait opéré ne donnait plus de nouvelles et que ses factures n'avait pas diminué. J'ai également une pensée à toutes celles et ceux qui ont renoncé à effectuer des travaux chez eux parce que les démarches étaient trop compliqué à tous ces mères aussi qui n'osent pas rénover logements communaux par la complexité des dispositifs. Pour toutes ces personnes. Cette proposition de loi entend recentrer l'effort budgétaire du pays sur les passoires thermiques. Alors avec l'article hein. Nous voulons donc. Un meilleur fléchage des aides publiques vers les travaux de rénovation plus performante. Nous voulons tout simplement aussi un mécanisme qui permet un reste à charge zéro pour les plus précaires. Sans ce reste à charge zéro. Les objectifs de rénovation se mettront en de manière inégalitaire. Et ne seront jamais atteints. De toute évidence la mention du reste à charge minimale obtenue par le Sénat lors de. L'examen de la, de, du projet de loi climat résilience est aujourd'hui sans effet avec un reste à charge parfois qui peut atteindre 40% pour les plus modestes. Avec l'article de nous souhaitons favoriser le aller vers. Le aller vers vers les personnes en situation de précarité partout sur le territoire, leur assurer un accompagnement gratuit qui se traduit par un montage à la fois technique et financier du projet et qui se poursuit d'ailleurs jusqu'à la fin de leurs travaux. L'article 3 lui vise à s'adapter aux contraintes des propriétaires occupants en leur permettant de s'engager dans un parcours de rénovation plus incitative. Enfin, l'article 4. Prévoit une adaptation des normes dans les territoires d'outre-mer pour mieux tenir compte des spécificités territoriales. Voilà les propositions que nous défendons pour résorber la précarité énergétique. Voilà comment nous entendons replacer la question sociale dans la transition écologique pour en finir avec la logique objectif trop ambitieux. Rétropédalage permanent. L'heure n'est plus aux rapports alarmants. L'heure n'est plus au plan de sobriété cosmétiques et autres bouclier tarifaire qui n'apporte que des solutions temporaires. L'et de passer des paroles aux actes. Hé oui pour l'apaisement. Il faut des actes. Ayons le courage de le faire ce soir, notre objectif avec cette proposition de loi et d'envoyer des signaux positifs aux citoyens qui aujourd'hui ne perçoit toujours pas dans leur quotidien, les effets concrets de la transition énergétique. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Dominique Estrosi Sassone, rapporteur de la commission des affaires économiques pour 10 minutes. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, mes chers collègues, la commission des affaires économiques vous propose dans sa majorité de rejeter le texte. J'ai conscience que sur un tel sujet, la lutte contre la précarité énergétique. Cette position peut surprendre. Je voudrais cependant vous en expliquer les motifs sachant que nous aurions préféré un renvoi en commission qui n'a pas été acceptée par l'auteur de la proposition de loi, ni par son groupe choix que nous respectons. Pour autant, monsieur l'auteur nous n'avons aucunement empêché d'amender le texte. J'insisterai en 1er lieu sur le fait que nous partageons sans hésitation les constats et les objectifs de lutte contre la précarité énergétique. Mais pour des raisons de temporalité et de fond. Nous pensons que des mesures qu'elle propose 100 pour certaines contre-productive et pour d'autres satisfaite par le droit existant. Je veux tout d'abord insisté sur la nécessité d'une accélération de la rénovation des logements et des passoires thermiques pour permettre la sortie de la précarité énergétique. Le rapport de l'Observatoire national de la précarité énergétique qui a été publié le 16 mars dernier dresse le constat alarmant d'une situation qui s'est aggravé en 2021, 11 9 % des Français ont dépensé plus de 8% de leurs revenus pour payer leur facture énergétique de leur logement et sont donc considérés comme souffrant de précarité énergétique en 2022, 863.000 ménages ont subi une intervention d'un fournisseur d'énergie en raison d'impayés, soit une hausse de 28% par rapport à 2019. La France s'était pourtant engagé à travers la loi pour la transition énergétique et la croissance verte de 2015 à rénover 500.000 logements par an, dont la moitié occupés par des ménages modestes pour disposer d'un parc basse consommation d'énergie en 2050 et réduire de 15% la précarité énergétique à l'horizon 2020. Cet engagement a d'ailleurs été réitérée à l'occasion de la loi climat et résilience, mais notre pays risque de ne pas atteindre cet objectif ambitieux. ambitieux. Selon le rapport de juin 2022 du Haut Conseil pour le climat, les émissions du bâtiment représente 18% des émissions nationales de CO2. Elles ont baissé de 0,2 millions de tonnes sur 2019 2021 alors qu'elle devrait baisser de de 3 à 4 millions de tonnes, selon la stratégie nationale bas-carbone dans la période 2022 2030. Cette trajectoire devrait se traduire par 370.000 rénovation globale et performante, puis 700.000 par an à partir de 2030. Or, selon le rapport de février 2023 de l'Observatoire de la rénovation énergétique des logements en 2019 2, 4 millions de logements ont bénéficié d'une aide pour des travaux qui ont permis 8. 6 TWh par an d'économies d'énergie. Mais il s'agit pour l'essentiel de rénovation partielle. Selon l'Agence nationale de l'habitat 66.000 rénovations globales ont été réalisées en 2022 en progression certes mais encore très loin de l'objectif visé au total 3 4 milliards d'euros de subventions ont été distribuées par l'Anah, mais l'essentiel n'a conduit qu'à changer le mode de chauffage, on peut donc dire que si la massification des aides et des gestes de rénovation a été réussie, celle des rénovations globales restent à entreprendre, à cet égard les mesures les plus contraignantes contre les passoires thermiques de la loi climat résilience commence juste à entrer en vigueur et donc à produire leurs effets. Les biens les plus énergivores et classé j'ai plus sont interdits à la location depuis le 1er janvier 2023 avant léger en 2025 Les S en 2028 et les oeufs. En 2034, de même l'obligation de réaliser un audit énergétique pour les bien classés G et F est entré en vigueur le premier avril seulement de cette année, il s'appliquera aux bien eux en 2025 et au des, en 2034. Les conséquences de ce calendrier exigeant qui avait d'ailleurs suscité notre inquiétude dès 2021 sont d'ailleurs particulièrement lourde et complexe pour les propriétaires bailleurs pour les vendeurs et pour l'ensemble d'un secteur immobilier sous forte tension est en cours de structuration pour faire face à cet enjeu. Si comme vous l'avez compris. Je partage donc les constats et la volonté d'aller de l'avant des auteurs de la PPL, j'estime que ce texte arrive à contretemps et que les solutions proposées sont soit contre-productive soit déjà satisfaite par le droit existant. En effet, l'examen de la proposition de loi intervient en avance de phase 2 2, échéances importantes pour notre assemblée, tout d'abord à la demande du groupe écologiste solidarité et territoires. Le Sénat a lancé en janvier 2023 une commission d'enquête que je préside sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique des bâtiments. La précarité énergétique comme l'ensemble des sujets qui sont liées, font de ce fait actuellement l'objet d'un examen approfondi les conclusions et les propositions de la commission d'enquête devrait être publié fin juin. Ensuite, comme l'a récemment confirmé la Première ministre, le gouvernement doit présenter au Parlement d'ici la mi-2023. La nouvelle loi de programmation quinquennale sur l'énergie qui permettra de fixer dans la loi les objectifs de politique énergétique dont ceux afférents à la précarité énergétique. S'en suivra l'actualisation de la stratégie nationale bas-carbone et de la programmation pluriannuelle de l'énergie en découlant peut être d'ailleurs Monsieur le Ministre pourrez-vous nous donner quelques éléments sur le volet rénovation énergétique de ce futur projet de loi sur le fond, après avoir consulté plusieurs acteurs du secteur. Et suite aux auditions de la commission d'enquête, je doute de l'efficacité des mesures proposées par la proposition de loi certaines dispositions paraissent contreproductives. Je voudrais en donner 2 exemples, la proposition de loi prévoit dans son article 1er un reste à charge nul pour les plus modestes, alors que la loi prévoit déjà à la demande du Sénat sur mon initiative un reste à charge minimale certes aujourd'hui le reste à charge est trop élevé et rend difficilement envisageable le lancement d'une rénovation globale pour ces ménages mais d'une part ce n'est pas la loi qui changera cette situation liée au montant et à la structure des aides et d'autre part, la plupart des acteurs rejettent cette idée pour des raisons de respect et de dignité des personnes concernées philosophique philosophiquement je suis convaincu que chacun doit toujours contribué à la hauteur de ses moyens, même de manière très réduite pratiquement j'ai également la conviction que les ménages doivent rester des acteurs de la rénovation de leur logement, au risque sinon de retomber dans les travers des rénovations à un euro. Ensuite, l'article 3 prévoit d'accorder jusqu'à 6 ans pour la rénovation d'une la réalisation pardon d'une rénovation globale et performante. Or, tous les acteurs du logement estime que l'idéal et de la réaliser en une seule fois et au maximum en 2 ou 3 étapes dans un délai court au risque sinon d'en perdre le bénéfice d'ailleurs actuellement, la loi prévoit un délai compris entre 18 mois et 3 ans selon la situation du logement et notamment la taille de la copropriété. Il n'est pas souhaitable d'aller au-delà. Au-delà de ces 2 questions, beaucoup de dispositions de la proposition de loi soit sont aujourd'hui satisfaites par le droit existant. Je voudrais citer donc l'article 3 qui propose que l'Observatoire national de la précarité énergétique contribue à identifier localement les ménages en difficulté. Or là aussi à la demande du Sénat et sur mon initiative. La loi prévoit déjà la transmission des audits et des diagnostics de performance énergétique non seulement à l'Ademe, mais aussi à tous les acteurs de l'aide sociale, y compris aux associations de lutte contre la précarité énergétique. Par ailleurs, l'Observatoire national de la précarité énergétique a déjà un outil de géolocalisation de la précarité énergétique. J'ai type il a été utilisé par 1500 communes environ et pourrait se développer plus encore à l'avenir. Enfin l'article IV voudrais préciser les missions du Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB mais aux dires mêmes de son président que j'ai interrogé. Non seulement il dispose d'ores et déjà des compétences évoqué mais la rédaction de la proposition de loi pourrait être un obstacle à leur bonne exercice sur tout le territoire. Voilà, madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous avez là devant vous. L'ensemble des raisons qui ont conduit la commission des affaires économiques a rejeté cette proposition de loi nous en partageons les constats. Vous l'aurez compris, mais nous pensons que nous devons encore travailler sur les solutions pour très Vincent vraisemblablement être deux semaines de nature à les intégrer. D'une manière ou d'une autre dans la future loi qui viendra au Sénat à l'Automne sur la programmation de l'énergie mais aussi à partir à partir des propositions qui seront faites par la commission d'enquête sur des futures propositions de loi qui pourrait également en découler. Je vous remercie. Alors la parole est à monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement. Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires économiques. Madame la rapporteur mesdames et messieurs les sénateurs. L'examen de cette proposition de loi nous permet d'évoquer un phénomène trop souvent méconnue mais qui touche des millions de Français. Une précarité que l'on ne voit pas une précarité qui se joue derrière les portes d'un appartement ou d'une maison. Un phénomène qui se fait d'autant plus prégnant dans ce contexte d'inflation couplée à une crise climatique. Nous sommes aujourd'hui à la, à la croisée des chemins. Nous avons dû affronter une crise énergétique exceptionnel qui s'est ajoutée à une urgence climatique que nul n'ose plus aujourd'hui contestée. Cette précarité. Cela a été rappelé lors des travaux en commission a des conséquences multiples. Économique tout d'abord, pour ma part je ne crée pas d'antagonisme entre fin du mois et fin du monde. Dans ce contexte de crise il serait insupportable que certains de nos concitoyens et à choisir entre manger et se chauffer. Nous n'acceptons pas cela. Des conséquences sanitaires, ensuite comme vous l'évoquez dans l'exposé des motifs avec des logements dans lesquels on respire mal où on développe des pathologies respiratoires. J'en suis convaincu rénové s'est des vies c'est parfois même sauver des vies. Des conséquences sociales aussi. Nous savons bien l'atteinte à la vie sociale que c'est pour des occupants qui ont honte de recevoir des gens dans un appartement rongé par l'humidité, la moisissure et qui n'osent pas y élever une famille. Et enfin des conséquences environnementales évidemment. Les plus pauvres sont les plus sobres énergétiquement mais pour eux c'est une sobriété subit au détriment de leur confort de leur santé, voire de leur dignité. C'est pour cela que j'ai également annoncé il y a quelques jours la liste des 25 premiers quartiers résiliant dans le cadre de l'ANRU afin de développer l'excellence environnementale dans les opérations de renouvellement urbain. En un mot l'urgence environnementale et une urgence sociale. Voilà pour les constats. Mais en tant que ministre, bien évidemment, je ne peux pas me contenter de dire que ces constats sont inacceptables. Le plus important c'est d'agir et c'est ce que je fais, c'est ce que nous faisons, c'est ce que font les services de l'État avec les parlementaires, les collectivités et les associations. Oui, l'État agit. Avant de parler de la rénovation qui est au coeur de notre réponse de fond. Ce gouvernement a agi pour protéger tous les Français, dans le contexte actuel de prix de l'énergie très élevé. C'est l'objectif des bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité qui continueront de protéger les Français en 2023 en particulier les plus fragiles. Bruno Lemaire l'a annoncé le bouclier tarifaire sur l'électricité sera maintenu jusqu'en 2025 serait maintenu jusqu'en 2025. Le gouvernement sera présent aux côtés des ménages tant que les circonstances le nécessiteront. Nous avons agi également au coeur de la crise avec le chèque énergie exceptionnel venu compléter les boucliers pour près de 12 millions de foyers les moins aisés. Dans ce contexte particulier et malgré les dispositifs déployés. Nous devons continuer à faire preuve d'une vigilance toute particulière sur la question des impayés de loyer et de charges. Pour agir sur le fond au bénéfice de nos concitoyens nous avons massifier la rénovation thermique avec une aide plus simple plus puisse plus puissante. Rénov'. Une aide bonne pour la planète est bonne pour le pouvoir d'achat dont ont pu en bénéficier, 1,5 millions de ménages majoritairement des modestes et des très modestes. Eh oui, monsieur le sénateur. Plus de 70.000 rénovations performantes ont eu lieu les 2500 que vous avez évoqué, ce sont les familles qui ont accepté et demandé sollicité le bonus. Il y a également MaPrimeRénov sérénité qui complète le dispositif pour les ménages très modestes souhaitant engager une rénovation globale de leur logement. Notre objectif est d'aller vers plus de bouquets de travaux plus de rénovation globale et performante, en particulier dans l'habitat collectif. Toutefois derrière l'objectif il y a la réalité. Et je sais les difficultés et les contraintes que peuvent représenter les rénovations globales. Ainsi les rénovations par geste même si elles ne sont pas idéales permettent de concrétiser une première étape et d'emmener des personnes réticentes sur le chemin de la rénovation énergétique. Et ma prime Rénov'n'est pas une simple aide qui est distribué. Non l'accompagnement doit être au coeur de cette démarche. Je parlais de personnes réticentes l'accompagnement doit permettre de créer cette confiance. L'accompagnement est indispensable pour expliquer les modalités et réaliser les travaux. Rénové. Ça ne doit jamais ça ne doit plus être un parcours du combattant. C'est la mission du service public France rénovent avec ses 550 guichets qui maille l'ensemble du territoire national. L'écoute. L'expertise technique et l'attention des conseillers partout sur le territoire national font la force de ce service public. Les plus de 2250 conseillers font en sorte que l'engagement dans des travaux vertueux ne soit plus jamais des sceptiques. Ils sont avec les collectivités, les acteurs principaux de notre stratégie d'aller vers. Damien à Tarbes, en passant par Nice. Ils sont présents pour que nos concitoyens y compris des territoires ruraux ou dans des quartiers populaires puissent avoir accès à ce service public de la rénovation. Je sais la visibilité que tous les acteurs de France rénovent ainsi que les collectivités qui le cofinancent attendent. Pour y répondre. Nous venons d'annoncer avec Christophe Béchu et Agnès Pannier-Runacher, le lancement d'une concertation avec les parties prenantes de France rénovent sur l'avenir du réseau et de son financement. La prolongation du programme Sar pour une année supplémentaire va permet de sécuriser la continuité du service public en 2024, ce qui est notre priorité. Elle va permettre également de travailler sereinement à un cadre de contractualisation ciblent plus simple, plus lisible, plus efficace. Notre objectif affiché par la Première ministre dans la feuille de route du gouvernement atteindre avec les collectivités un guichet par intercommunalités d'ici à 2025. Pour massifier l'accompagnement. Il faut faire appel à tous et je pense notamment aux accompagnateurs rénovent. La plateforme d'agrément de ces acteurs clés pour le parcours de rénovation des ménages vient d'ouvrir en ce début de semaine pour prendre en compte la situation des acteurs économiques déjà actifs puis agréer de nouveaux acteurs prêts à s'engager sur ces prestations. La concertation sur l'avenir de France Rénov sera l'occasion de donner de la visibilité à ces nouveaux acteurs sur le modèle économique qui sera soutenue par la création d'un nouveau programme. National de ces deux. Notre Notre cap est clair, disposer là d'ici la fin de l'année d'un vivier d'accompagnateurs rénovent permettant de soutenir une montée en charge significative des rénovations globales en 2024 en cohérence avec les travaux de la planification écologique. Un mot aussi sur les dispositifs de la loi climat et résilience qui interdiront progressivement la mise en location des passoires énergétiques. Une loi qui répond d'ailleurs largement aux demandes de votre proposition de loi tant sur le service public de la rénovation que sur l'identification des ménages en situation de précarité énergétique, cette avancée ayant été permise par le Sénat. Sur le calendrier mis en place par la loi. J'entends les doutes et les inquiétudes de certains professionnels du secteur mais j'ai aussi entendu comme vous, d'autres personnes me dire que nous n'allions pas assez vite et je les comprends aussi. Tenir le calendrier, c'est tenir la promesse faite aux occupants de ces passoires thermiques et qui va changer concrètement leur vie. Tenir le calendrier, c'est la crédibilité de la parole publique qu'il ne faut surtout pas entamé sur un sujet aussi grave. Les mesures les plus contraignantes viennent d'entrer en vigueur. Récemment, vous le savez, depuis le 1er janvier les biens étiqueté j'ai plus sont interdits à la location et l'obligation de réaliser un audit énergétique pour la vente de maisons individuelles classé F et G est est entré en vigueur depuis le premier avril. J'ai installé le 13 avril dernier, un comité des partenaires de la rénovation du parc locatif privé. Il ne s'agit pas de créer une instance de concertation, de plus mais de créer un espace d'échange et de travail avec les acteurs impliqués au plus près du terrain pour informer, faire connaître les bonnes pratiques qui fonctionne et levée des freins très opérationnel. Là aussi, le cap est clair. Nous sommes dans le temps de l'action de la mobilisation pleine et entière de tous les leviers qui existent pour apporter des réponses concrètes aux Français qui vivent dans les logements les plus énergivores. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Même si nous partageons les constats que pose cette proposition de loi, force est de constater que beaucoup a été fait pour lutter contre cette précarité énergétique. Cela ne signifie surtout pas qu'il ne faut pas continuer d'agir. Le gouvernement et le Parlement sont au travail avec plusieurs échéances qui rendent moins pertinente, l'examen de ce texte. Je pense aux travaux de planification écologique conduit avec la pluie du secrétariat général pour la planification écologique, sous l'égide de la Première ministre dont la rénovation des bâtiments de tous les bâtiments est un chantier de 1er rang. Ces travaux permettront de donner de la visibilité à tous les acteurs et de décliner concrètement de grandes orientations que nous partageons tous. Accélérer la rénovation du parc de logements notamment l'éradication des passoires énergétiques et la sortie des énergies fossiles. Faciliter le parcours de nos concitoyens, en particulier les plus modestes. Former les filières de demain et structurer la filière. sera présenté la restitution des travaux du Conseil national de la refondation du logement il abordera bien sûr le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Enfin je pense également aux conclusions dans les prochains mois de la commission d'enquête sénatoriale que vous présidez madame la rapporteur sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique et qui viendront naturellement alimenter notre feuille de route. Ainsi. Ces travaux nous permettront d'approfondir les propositions du texte, dont de nombreuses sont en partie déjà satisfaite. Comme l'a souligné la Commission. Je tiens à saluer d'ailleurs la qualité de ses travaux et le temps consacré à l'audition des différents acteurs. Mesdames, et messieurs les sénateurs, vous le comprenez au regard du travail déjà accompli des chantiers engagés des échéances à venir. Le gouvernement ne soutiendra pas cette proposition de loi. Je veux croire à la mobilisation collective, pour réussir au plus vite l'éradication des passoires thermiques de notre parc de logements. C'est pourquoi nous ferons avec vous monter en puissance le service public de la rénovation. C'est pourquoi nous encouragerons encore davantage les rénovations globales afin que les ménages, notamment les plus précaires vivent mieux dans leur logement. Ainsi nous bâtirons une transition énergétique qui soit efficace, concrètes et populaires. Je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre, alors dans la suite de la discussion générale. La parole est à Madame, Viviane Artigalas pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour six minutes.

Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, madame le rapporteur, madame la présidente de la commission des affaires économiques, mais chers collègues ces derniers mois notre assemblée a eu à débattre de plusieurs textes, relatifs aux politiques du logement et tout récemment de la proposition de loi visant à mieux protéger les locataires bénéficiant d'une allocation de logement et vivant dans un habitat non descend. S'il n'apporte pas toujours de solutions adaptées ces textes partagent en revanche un même constat, alors que la France a pris des engagements environnementaux et sociaux visant notamment à réduire les passoires thermiques d'ici 2028 qu'la même à louer des moyens conséquents et obtenu quelques progrès 3,1 milliards d'euros ont été dépensés en 2022 pour des travaux dans 670.000 logements. Les politiques publiques demeure inefficaces face à l'ampleur de l'enjeu au contraire la précarité énergétique s'accroît renforcer en cela par un contexte de hausse des prix de l'énergie qui touche les plus vulnérables. 5,6 millions de ménages sont concernés et ce chiffre ne baisse pas, 37% des passoires thermiques sont occupés par des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté et les territoires ruraux sont particulièrement touchés par la vulnérabilité énergétique pour ce public précaire, il est impossible d'engager des travaux de rénovation globale donc performante à raison de reste à charge de 35 à 55 à 50% du monde tente des travaux ce qui n'est pas un montant minimal c'est une dépense beaucoup tout près importante que pour leurs finances. Et de ce fait les passoires thermiques demeure. En raison d'une complexité administrative réel de dysfonctionnements techniques persistants je pense naturellement à la plateforme Mac prime ne rénove et de l'importance de la fracture numérique. Les publics concernés par les aides de l'État n'y accèdent pas, faute d'un accompagnement adapté et d'un manque de coordination des différents corps de métiers de la filière, artisanat et quand ils y accèdent, les subventions mettre trop de temps à arriver. Objectif et constats sont partagés. Les moyens sont là, pourtant, rien n'avance, alors qu'il y a urgence à tenir les engagements annoncés. La France risque de passer encore une fois à côté d'un enjeu majeur pour la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, faute d'avoir pu obtenir un DPE conforme les logements les plus énergivores risque faute de rémunérer l'innovation de sortir du marché de la location. 90.000 logements du parc privé sont potentiellement concernés. Depuis le 1er janvier 2023, ce chiffre passerait à 160.000 au 1er janvier 2025. La révision de la stratégie française sur l'énergie et le climat sera discuté dans les prochains mois ce l'autre doit être l'occasion de porter des priorités d'action nouvelles. Agir pour la priorité Hertner génétique. agir pour résorber la précarité énergétique est une nécessité à la fois social et environnemental, qui demande une stratégie de rénovation des logements plus performante et plus inclusive. À travers ce texte visant à résorber la précarité énergétique que le groupe socialiste, écologiste et républicain se veut déjà force de propositions dans la perspective de loi de programmation pluriannuelle dont nous débattrons cette année c'est 4 articles structure une stratégie cohérente pour atteindre les objectifs de la loi climat et résilience et rétablir le principal le principe d'égalité et de justice sociale dans la mise en oeuvre de notre transition écologique principe que nous avions déjà défendu lors de l'examen de cette loi. Nous souhaitons ainsi prioritairement recentrer l'effort budgétaire de la France sur l'éradication des passoires thermiques mettent à ma place. Reste à charge zéro pour les personnes les plus précaires favoriser le aller vers pour toucher tous les foyers et les Gibloux aux aides à la rénovation d'énergétique et pour se faire poser le principe de l'égalité d'accès au guichet France rénove et aux accompagnement. Accompagnateur rénovent sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones de faible densité de population, dans un souci de prise en compte des réalités quotidiennes. Nous souhaitons également permettre aux propriétaires occupants sans possibilité de relogement de réaliser leurs travaux de rénovation globale en plusieurs tranches dans leur cadre d'un parcours financer accompagné et planifié. Enfin nous proposons d'encourager l'innovation dans les techniques de matériaux de rénovation afin d'améliorer la prise en compte des spécificités locales, ce qui vaut particulièrement pour les territoires d'outre-mer. Bien que nos constats sur le besoin d'accélération de la qu'rénovation énergétique des bâtiments et la lutte contre les passoires thermiques et était unanimement partagé, lors de l'examen en commission l'autre texte a été rejetée par cette même commission. Nous ce temps néanmoins rappeler qu'il y a urgence à trouver des réponses efficaces et concrètes. Nos propositions sont adaptés à la réalité quotidienne de nombreux notre de nos concitoyens. Elle se base sur des situations réelles vu et entendu et entendu dans nos circonscriptions et dans de nombreux reportages. En 2021 11,9 % des Français ont dépensé plus de 8% de leurs revenus pour payer les factures énergétiques de leur logement et sont donc considérés comme souffrant de précarité énergétique. En 2022, le nombre de ménages ayant suivi plus subi une intervention d'un fournisseur d'énergie en raison des épée d'impayés avaient augmenté de Vire, 28% en 3 ans, notre texte se veut une alerte les efforts de rénovation subissent de fortes inégalités territoriales et ce n'est pas normal. Nos concitoyens subissent une forte inégalité d'accès aux dispositifs nationaux encourageant les rénovations et ce n'est pas normal. La transition énergétique, comme bien d'autres domaines assez privilégié ces laissés pour compte et nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pour ça que je vous invite à voter cette proposition de loi, je vous remercie. Merci. La parole est à madame Marie-Noëlle Lienemann. Pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour 4 minutes. Mes chers collègues résorber la précarité énergétique devait être une priorité absolue de la nation dans cette période. Période d'inflation. En jeu de précarité. Énormes problèmes de pouvoir d'achat. Un enjeu social. Enjeu environnemental à la fois au regard de la lutte contre, effet de serre mais aussi jeu de souveraineté parce que plus nous commençons, nous dépensons d'énergie, notamment en gaz et autres, plus nous sommes fragilisés dans nos écoles nous échanges commerciaux. Donc on devrait dans cette situation mobiliser tous nos efforts et nous constatons et nous de ce point de vue nous partageons totalement le diagnostic fait par nos collègues du groupe socialiste, c'est que, en la nature même de nos efforts n'est pas à la hauteur de la tâche, ni pour les médias ni pour l'avenir. Alors que les médias avant de rentrer sur le bâti. Je voudrais dire quelques mots d'un certain nombre de décisions urgentes qui s'imposent. En effet, vous savez que la dérégulation des prix du gaz va avoir lieu au au début de l'été ça va avoir un effet catastrophique en dépit des boucliers qu'on nous annonce sur de nombreuses familles et notamment des familles précaires. Nous demandons le report de cette dérégulation. De. Et de l'abandon des tarifs réglementés. 2ème sujet majeur. Ce qui est, ce que nous avons proposé depuis des années, c'est-à-dire la revalorisation de l'APL charge. Qui n'a pas été revalorisée dont nous demandons au moins le doublement car c'est un, un moyen de solvabiliser les familles. Alors après on va nous dire que la prime énergie mais il n'est pas à la hauteur des problèmes et d'ailleurs dans certains cas, elle est même pas encore mis en oeuvre. Je voudrais soutenir la démarche des gestionnaires de pension de famille de résidences sociales de foyers de jeunes travailleurs car à ce jour il ne touche pas le la prime énergie et vous savez comme ça j'ai pas d'un bail et d'une location. C'est bien le gestionnaire qui doit toucher l'argent en l'occurrence, ces jeunes, ces personnes en faisant en pension de famille sont en difficulté majeure. on, je ne vais pas revenir tout le monde a dit sur l'ampleur des mobilisations nécessaires pour le bâti tard évidemment il s'agit pas simplement d'aider les familles. Il s'agit structurellement de résorber. Elle est pas sûr thermique et globalement de fermeté tout le parc de logements dans une qualité environnementale avec la moindre consommation énergétique. J'entends bien Monsieur le Ministre, ce qui vous nous dites quand je vous écoute. J'ai l'impression qu'il suffit de continuer comme on est et qu'on va atteint des objectifs sur ce qu'il y a pas un spécialiste. qui considère qu'avec l'état actuel de la prime Rénov'. Nous allons atteindre nos objectifs. Veut tout, une fois de plus être au tribunal pour insuffisance énergétique. Donc moi je le dis tout Net, c'est une révolution copernicienne. Nous attendons beaucoup des travaux de la commission d'enquête mais les propositions actuelles du groupe socialiste sont une première étape qui devront être complétées peut être réorientée dans certains cas le signe politique doit donner aujourd'hui ici et maintenant. Je voudrais terminer sur un problème que nous rencontrons qui les fameux accompagnateur. Prime. Notre grande crainte et qu'on ouvre, tellement les vannes de la légitimation de certain nombre d'acteurs dont certains sont privés. Pas toujours avec les compétences. Je pourrais vous donner 1002 exemples, par exemple de pompes à chaleur qui sont sous sous nous estimé quant aux volumes nécessaires et quand vous regardez le bilan de la facture des gens, elle est supérieure à ce qu'ils avaient avant avec ancienne une chaudière. Il faut que ces acteurs de d'accompagnement soient certifiés de sérieux en public et en tout cas c'est impératif car l'accompagnement doit être un prérogatives de service. Public. Merci. La parole est à madame daphné Ract-Madoux pour le groupe Union centriste pour six minutes.

Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires économiques qui s'est absenté madame la rapporteure, chers collègues. Sous l'influence conjuguée de la hausse du coût des matières premières et de l'inflation des prix de l'énergie. La précarité énergétique a éteint en 2022, un niveau inédit. Je souhaite donc remercier Rémi Cardon et nos collègues du groupe socialiste pour avoir mis sur le devant de la scène cette problématique primordial pour notre avenir collectif. Loin d'être seulement l'apanage des frimas hivernaux cette précarité touche les Français les plus modestes à toutes les saisons. Ainsi. Un Français sur 4 déclarait avoir souffert du froid. Pendant au moins une journée complète au cours de l'hiver 2021 2022, quand 59% des foyers interrogé en 2022 par l'Observatoire national de la précarité énergétique. Estimait avoir souffert d'un extrait de chaleur dans d'un excès durant la période estivale. Nous devons donc penser une rénovation énergétique globale pour l'ensemble des saisons. C'est une obligation. Si les Français ont su participer pleinement à l'effort national en matière de sobriété énergétique. La mise en place des bouclier tarifaire sur le gaz et sur l'électricité. A été une réponse conjoncturelle salvatrice pour les ménages. Je crois que nous pouvons tous le reconnaître. En parallèle, le gouvernement agit depuis plusieurs années pour lutter structurellement contre ces phénomènes de précarité énergétique. La montée en puissance des différents dispositifs comme ma prime Rénov'est à saluer, mais des dysfonctionnements persistent et il reste du travail pour faire progresser cet outil et le rendre plus opérationnelle en massifier en notamment les actions de rénovation globale des logements. En première ligne dans ce combat les copropriétés ont été dotés d'un dispositif spécifique permettant de faciliter la rénovation collective. En 2022, c'est un peu moins de 645.000 rénovations individuel du logement et seuls 26.000 copropriétés ont été rénovés grâce à ma prime Rénov'co-propriété. Dans cette perspective, le relèvement des plafonds de ce dispositif le 25 avril dernier, est un nouveau pas réalisé en direction d'une massification de la rénovation énergétique. S'il est encourageant. Le bilan de la rénovation énergétique reste néanmoins perfectible. Sur les 670.000 rénovations déjà réalisé près de 604.000 sont des rénovations mono gestes là où on compte seulement 65.000 rénovation globale, Monsieur le Ministre, nous devons faire plus. Nous serons à vos côtés pour relever ce défi. Le succès de la lutte contre la précarité énergétique passera indubitablement par une meilleure reconnaissance du rôle joué par nos collectivités pour bâtir des solutions locales et adapté aux réalités de nos territoires. À ce titre, je tiens à saluer les initiatives prises par le département de l'Essonne et notamment la prime écologique 91 cette aide forfaitaire versée sous condition permet aujourd'hui aux propriétaires de financer des travaux induisant d'importants. Gains énergétiques ce type de dispositif local. Permet de diminuer le reste à charge est de renforcer les effets de leviers en matière de financement des rénovations énergétiques, soit 2 axes identifiés par les travaux d'une commission d'enquête sénatoriale, mais ils ne sont pas les seuls. Pour agir plus efficacement localement, nous devrions également consolider généraliser le modèle des agences locales de l'énergie et du climat les Alec ces agences qui réalise gratuitement des diagnostics énergétiques objectif et indépendant afin que chacun puisse bénéficier des meilleurs audits dans le cadre de son projet de rénovation. Ce sont des institutions qui ont fait leurs preuves. Mais elles ne sont pas présentes partout. On compte aujourd'hui par exemple une Alec en région Normandie 10 en région Île-de-France et 40 sur la France entière le travail mené par les Allègre doit être mieux associés à celui réalisé par les accompagnateurs rénovent sur le terrain. Cessons d'agir en silos et bâtissons de nouvelles synergies afin de coupler plus efficacement diagnostic et rénovation énergétique. Arrivons à contretemps et ceux qui sont des solutions conjoncturelles détricotant les mesures prises mises en place par nos lois les plus récentes. Cette proposition de loi pose les bonnes questions mais formule malheureusement les mauvaises réponses, je tiens à féliciter notre rapporteur Dominique Estrosi Sassone pour l'excellence de son travail qui mettrait justement en lumière les limites de ce texte. En effet, l'illusoire reste à charge zéro porté par les auteurs du texte n'est pas la seule préoccupation, que nous devons avoir en matière de rénovation énergétique du logement. Si nous devons diminuer effectivement le reste à charge. Il nous faut également impliquer, responsabiliser les propriétaires. Enfin là où la commission d'enquête sur la rénovation énergétique même des travaux fournis dans l'optique notamment de l'examen prochain prochain de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Cette proposition de loi est une démarche arrivant à contretemps. Avec un mail Gacquerre et les membres du groupe centriste. Nous sommes conscients que la précarité énergétique est une problématique fondamentale et qu'il ne faut pas galvauder avec des demi-mesures et des fausses promesses, nous suivrons donc notre rapporteur et nous ne voterons pas pour ce texte. Je vous remercie. Merci la parole est à madame Guylaine Pentel pour le groupe du Rassemblement démocratique. Et social européen pour 4 minutes. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques. Madame la rapporteure, mes chers collègues. Le phénomène de précarité énergétique a pris une place particulièrement médiatisée dans notre espace politique, économique et sociale. En plus d'être délicate. La situation est inédite et là je multiple. Après la crise du Covid, qui a mis en évidence d'urgence à remédier à ce phénomène. L'année 2022 la accrue par son inflation élevée provoquée par la hausse des prix de l'énergie comme des matières premières et exacerbée par des hein, nationaux et internationaux que chacun connaît. L'année passée, 22% des Français ont déclaré avoir souffert du froid chez eux aussi. 69% des Français ont réduit leur consommation énergétique et ont eu des difficultés à payer leur facture. Sur la forme, le groupe RDSE rejoint la position de la Commission car il serait préférable d'atteindre des conclusions de la commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Attendu à juillet 2023, avant de légiférer. De même que la loi de programmation quinquennale sur l'énergie. Quant au fond, nous ne pouvons aborder la thématique de la précarité de la précarité énergétique sous le seul prisme de ses conséquences sociales et économiques. En effet, si elle est synonyme d'une situation financière dégradée d'un isolement social et d'une santé physique menacé sa dimension environnementale témoignent de l'urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons. La rénovation énergétique des logements est un objectif majeur pour la transition vers une économie moins carbonée. Elle n'est d'ailleurs pas qu'une obligation imposée par le changement climatique et une précarité grandissante. Elle concerne aussi la sauvegarde du Patrimoine bâti la défense de notre balance commerciale et la création d'emplois. L'action publique d'un sous-domaine doit donc être largement repenser et nécessite de trouver une articulation juste entre plusieurs principes. Le secteur du bâtiment fonctionnant avec des talons. Il faut donner aux acteurs, une vision de long terme et une politique publique stable afin qu'ils aient la capacité de préparer et d'un anticiper les changements. Afin de créer une dynamique forte. Pérenne et massive de rénovation énergétique. Il faut s'appuyer sur 2 éléments indissociables d'une part signale législatif et réglementaire orientale la réflexion et la décision du propriétaire. Et d'autre part le réflexe de performance énergétique à chaque occasion de travaux. Or cela ne peut se faire face d'une structuration de l'offre et une adaptation de la filière professionnelle. Par ailleurs le principe de réduction du besoin de consommation doit guider le projet de rénovation globale les rénovations énergétiques partiel focalisé notamment sur sagement du mode de chauffage ne peuvent pleinement satisfaire nos objectifs a matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il est nécessaire de rénover les enveloppes de manière performante et d'utiliser une énergie décarbonée. Ainsi pour une accélération efficace la fille la vision doit être globale et embrasser tous les problèmes pouvant faire obstacle à sa mise en oeuvre. Néanmoins, au-delà de la viabilité économique d'autres Fremm peuvent empêcher ces ces rénovations d'être menée à bien. Complexité des dossiers crainte des surcoûts des malfaçons difficulté de trouver des artisans dérangement causé par l'ampleur des travaux de rénovation globale. Les réponses à ces frais ne sont pas nécessairement financière mais plutôt dans la qualité des services et de l'accompagnement proposé aux ménages. En somme, le groupe RDSE souhaite s'appliquer à ce que l'ensemble de ces frais soient pris en compte à travers la loi de la programmation sur l'énergie et le climat. Nous partageons dans le constat de l'urgence mais nous reconnaissons l'inadaptation du calendrier législatif notre vote ce distribuera entre le pour et l'abstention. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à Madame, Catherine Bell Rithy pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues. C'est un constat accablant qui nous réunit ici aujourd'hui à la lumière des crises que nous traversons et qui s'enchaînent. Le poids des factures énergétiques des logements pèse lourdement sur les Français et aggrave la situation des plus modestes, dont le budget est déjà gangrénée par l'inflation depuis des mois ces dépenses sont souvent liés à la vétusté des logements et en particulier à leur isolation. Le constat dressé par le sénateur cardons et ses collègues et je le crois très largement partagé dans cet hémicycle. La rénovation des logements est actuellement insuffisante et son rythme doit être accéléré dans une logique, à la fois social, économique et environnementale. Les objectifs posés par la loi pour la transition énergétique et la croissance verte de 2015 était pourtant assez ambitieux et explicite rénover 500.000 logements par an, dont la moitié occupés par des ménages modestes pour disposer d'un parc basse consommation d'énergie en 2050 et réduire de 15% à la précarité énergétique à l'horizon Ces objectifs ont été réaffirmée à l'occasion de la loi climat et résilience en 2021 qui fixe une finalité disposer d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Inutile d'épiloguer sur la question. Cet engagement n'est pas tenu à l'heure actuelle et les quelque 66.000 rénovations globale réalisé en 2022 ne laisse guère présager une amélioration nette dans les prochaines décennies. Cependant si ce constat fait consensus. Les solutions proposées par le texte soumis à notre examen sont insuffisantes et requiert un sérieux approfondissement tout d'abord en matière législative il convient de ne pas aller trop vite en besogne, afin de conserver une certaine cohérence. Or la pertinence de ce texte est largement remise en cause par le calendrier, le Sénat qui sera amené à débattre à au moins 2 autres reprises et de manière exhaustive de cette question dans les prochaines semaines. Outre la future loi de programmation sur l'énergie et le climat présenté cet été par le gouvernement. Les conclusions de la commission d'enquête du Sénat sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique attendu pour juillet permettront en mettant en exergue l'ensemble des lacunes actuelles des dispositifs d'aide de l'État de dégager les solutions concrètes à leur apporter cette commission transpartisane. je le sais produit jusqu'à présent un travail rigoureux et complets dans ces auditions des différents acteurs du secteur et je suis persuadé que ses conclusions seront à la hauteur de l'investissement fournis par la présidente Estrosi Sassone et ses collègues dans ce contexte, il serait regrettable d'adopter des dispositions qui irait à l'encontre des travaux de la commission d'enquête, tout en étant potentiellement en décalage avec les futures propositions gouvernementales au-delà ce calendrier défavorable l'esprit du texte ne me semble pas non plus parfaitement en adéquation avec les objectifs actuels en effet loin d'être un approfondissement des lois votées précédemment sur le sujet. La PPL de monsieur. Fixe des nouveaux objectifs vertueux à atteindre sans prendre en considération le panorama des défis actuels et s'doter son texte des moyens nécessaires à leur réalisation. Cela transparaît dès l'article 1 qui cherche à conditionner l'accès aux aides à la réalisation d'une rénovation performante et global et à instituer un reste à charge nul pour les ménages les plus précaires. Concernant l'évaluation globale. La loi a déjà prévu une incitation financière accrue qui doit rester prioritaire néanmoins cette incitation doit demeurer souple et son évolution progressive pour ne pas déstabiliser le secteur et préserver les premiers succès obtenus par ma prime Rénov'. En effet, tous les ménages ne peuvent pas se permettre une rénovation globale quant. Qui elle même n'est pas toujours opportunes concernant le reste à charge. La loi prévoit déjà, à l'initiative du Sénat un reste à charge minimale qui est pour le moment, malheureusement pas appliquer la prise en charge même infime des coûts de rénovation est une question de dignité sociale cependant un reste à charge nul pour les ménages qui entreprendrait une rénovation globale aurait un coût exorbitant pour nos finances publiques. Dans ces conditions, mes chers collègues. Il me paraît impensable de voter en faveur de ce texte. La question de la karité énergétique située à l'embranchement de l'économie de la transition écologique et de la question sociale est trop importante pour être abordée de manière imparfaite et ce texte ne répond pas efficacement à 3 problématiques qui me semble. Essentielle à ce débat. Tout d'abord les modalités de financement et l'équilibre entre les aides de l'État et le nécessaire investissement personnel du ménage. Ensuite les moyens humains et matériels mis à disposition des ménages leur déploiement et l'usage qui en est fait par nos concitoyens. Enfin, l'information et la communication sur le sujet, aussi bien au niveau de la sensibilisation que de l'accompagnement de chaque étape et la de la démarche de l'initiative à la réalisation des travaux, la commission d'enquête nous donnera prochainement un premier aperçu de l'étendue du travail qu'il nous reste à accomplir en la matière,

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteur, madame la présidente de la Mission des affaires économiques. Mes chers collègues. La France a beau essayer d'atteindre objectif de réduction de gaz à effet de serre. Les émissions mondiales ne cesse de croître. Dans ces conditions, il est à craindre que le d'égarement climatique se poursuivent. Nous devons redoubler d'efforts pour mettre au point les technologies vertes de demain. Celle qui nous permettront de concilier croissance écologie. Cela ne justifie pas pour autant que nous avons renoncer à sobriété. Dans un contexte de hausse des prix de l'énergie. Tout le monde. On comprend l'intérêt. Et les partis partiellement pertinent d'investir pour réduire nos dépenses. A fortiori lorsque le disons si nous et nos émissions de gaz à effet de serre. La progression de loi que nous deux amidon entend lutter contre la paix précarité énergétique d'entropie. Nous partageons tous cette ambition, déjà mis en oeuvre par la loi. L'auteur de cette PPL propose plusieurs mesures. Il tient à ce que les fonds publics. Soient destiné à la région des ménages se concentrer sur les plus vulnérables de nos concitoyens et que ceux-ci puissent bénéficier d'arrêt ça se charge nul. L'intention est louable. Car sur le plan économique, ce sont nos ce qui concerne les plus modestes qui bénéficieraient le plus de ces rénovations. Mais les besoins sont-ils créateur de roi. Nous ne le pensons pas. Nous sommes en effet convaincu que les révélations doit être réalisé parce qu'elles sont rentables. Tant du point de vue économique qu'écologique. La rentabilité est une des conditions nécessaires et suffisantes au fonctionnement des rénovations. Dans cette logique. La question le le l'emploi l'agent public peut soulever des interrogations. Celle d'un reste à charge nul. Nous paraît encore plus emblématique et problématique dans la mesure où ce sont l'occupant et le propriétaire du bien qui récolteront les fruits de cet investissement. Il me paraît parfaitement incompréhensible, qui ne serait parti, pas du tout. À son effort et à son financement. Les travaux de le rapporteur nous a fait nous a fait apparaître que certaines des autres dispositions du texte sont satisfaites des guichets itinérants sont déjà en service de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire, sans qu'il soit de besoin d'en créer de nouveaux. Les spécif, les territoires notamment ultramarins sont déjà prises en compte. Pour le choix des méthodes et des matériaux employés à la rénovation. Pour le concitoyens et notamment parce qu'il est question d'argent public. Nous devons nous assurer de l'efficacité des dispositifs existants et de les parfaire le cas échéant. Nous sommes particulièrement attachés. Raison pour laquelle notre groupe a proposé au Sénat de mieux lutter contre. L'habitat non descend. En exhumant la PPL d'autres collègues, j'ai vu la gourde. Là aurait été a rappelé qu'une commission d'enquête sénatoriale a été lancé en janvier dernier. Elle vise précisément à faire le point sur l'ensemble des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. Ces conclusions doit être rendu prochainement avant l'été. Nous permettant et nous permettront de légiférer en connaissance de cause. Le calendrier défavorable à cette position de loi. Ce n'est pas l'élément qui motive notre vote. La rénovation énergétique est un investissement qui doit susciter selon nous les financements par sa rentabilité et non pas offrir aux propriétaires une rénovation Perrier par l'argent public. Le groupe les indépendants votera donc contre son adoption. Merci. La parole est à Monsieur Daniel Salmon pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour 4 minutes.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente des affaires économiques. Madame la rapporteure, mes chers collègues. Malgré une ambition politique sans cesse réaffirmée avec des des moyens financiers conséquents. Tous les rapports qu'ils viennent de la Cour des comptes de l'Assemblée nationale du comité d'évaluation de France, le plan France relance tous déplorent l'échec des politiques publiques en matière de rénovation énergétique des logements. De nombreux chiffres éloquents ont été rappelés, je n'y reviendrai pas. Si cette proposition de loi de notre collègue Rémi Cardon, part d'une bonne intention et d'un constat que nous partageons toutes et tous, à savoir la trop lente résorption des passoires thermiques le nombre trop faible de rénovation globale un reste à charge excessivement élevée pour les familles modestes des dispositifs d'accompagnement compliqué et trop méconnu. Ce texte nous le regrettons, est confronté à un problème de temporalité évident comme nous l'avons souligné en commission. Les travaux d'enquête. Les travaux de la commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique à l'initiative du groupe écologiste solidarité et territoires sont encore en cours. Elle a été mise en place pour faire justement la lumière sur les dysfonctionnements actuels formuler des recommandations structurantes et permettre ainsi une massification effective de l'indispensable effort national en matière de rénovation énergétique que nous appelons tous de nos voeux. Les résultats de ces travaux pourront être traduits dans une future proposition de loi ou dans la loi de programmation énergie climat annoncé a priori pour cet Automne. Pour résorber la précarité énergétique. Nous sommes convaincus de plusieurs éléments qui rejoignent en effet les objectifs de ce texte, l'accompagnement personnalisé des ménages par un référent est essentielle. Ah parcours simplifié une prise en charge financière pour des ménages modestes et nécessaire, le reste à charge actuelle étant toujours trop élevé. La formulation la formation de la filière, notamment sur les enjeux d'adaptation des normes et de l'innovation dans les techniques et matériaux de rénovation écologique et durable est un enjeu également majeur en ce sens, nous soutenons le principe de recentrer l'effort budgétaire sur les passoires thermiques pour respecter nos engagements climatiques et pour répondre à la précarité énergétique de nos concitoyens les plus modestes. Nous soutenons bien sûr l'accent mis sur les plus précaires à travers des aides via reste à charge zéro le principe d'égal accès aux guichets France rénove et aux accompagnateurs rénove et l'adaptation des normes et de l'innovation dans les techniques et matériaux de rénovation particulier selon les spécificités en outre-mer. Mais nous regrettons plusieurs points l'absence de mesures sur l'efficacité, les moyens financiers, la lisibilité des dispositifs d'ingénierie publique des agences de l'État au 1er rang desquels Lana et l'Laden tout comme de l'ingénierie territoriale notamment des agences locales de nerf de l'énergie et du climat les Alec ou encore l'absence de propositions sur le rôle et les moyens des collectivités locales pour accompagner cet effort national. Par ailleurs, les solutions proposées ne sont pas encore assez mûr ni optimale en ce sens. Nous regrettons la faible portée normative de certaines de ses propositions, je pense par exemple l'inscription dans la loi du principe d'égalité d'accès aux guichets France rénovée aux accompagnateurs cela n'entraînera pas nécessairement des changements concrets. Le guichet France rénovent est en plein déploiement et l'imperfection du dispositif actuel est largement partagée. Oui, il existe une une inégalité territoriale dans le traitement des demandes mais l'outil législatif n'est pas forcément le plus adéquat n'le plus efficace pour y remédier. En conclusion, nous voterons pour ce texte qui est un début de réponse avec des mesures que nous ne pouvons que soutenir mais il y a un questionnement sur leur efficacité. Nous considérons cette proposition de loi comme une étape participe à 100 essentielle qu'est la lutte contre la précarité énergétique. Je vous remercie. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques Madame la rapporteure. Mes chers collègues. En France, sur les 30 millions de logements, 5 millions sont considérés comme des passoires énergétiques. Or nous avons tous ici conscience de l'importance des déperditions de chaleur consécutive à un logement dont l'isolation et défectueuse. Ce constat nous place devant 2 conséquences majeures qu'il faut considérer avec la plus grande atteinte des attention. Rappelons tout d'abord qu'en raison de la piètre isolation de certains foyers quasiment 4 millions de ménages ont des difficultés à payer leur facture de chauffage. Nous ne pouvons rester insensible face à cette situation d'étranglement financier d'une partie non négligeable de la population. Nous avons déjà agi contre ce phénomène en effet ma prime Rénov'a permis de délivrer 416.000 subventions entre janvier et août 2022. Ensuite, l'existence de ces passoires énergétiques renforce ce phénomène qui représente probablement la plus grande menace de notre siècle. Je veux parler des émissions de gaz à effet de serre. En effet, le secteur du bâtiment représente à lui seul 27% des émissions de CO2. Il est donc fondamental pour notre société, de mettre en oeuvre toutes nos Todd RJ pour contrecarrer cette production qui empoisonne notre planète nous subissons déjà les premières conséquences du dérèglement climatique. L'ensemble de ces constats nous met face à nos responsabilités et nous avons joué en tant que législateur à agir pour stopper tenter de stopper rapidement l'ensemble de ces phénomènes, par conséquent, le groupe RDPI partage évidemment l'objectif de ce texte. Cependant nous émettant plusieurs réserves sur cette proposition. En effet, ce texte est étudié avant des échéances importantes qui concernent la sécurité, le sujet de la précarité énergétique. Je pense notamment à la commission d'enquête lancée par le Sénat sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique des bâtiments dont les conclusions seront publiées entre les mois de juin et juillet 2023. Mes chers collègues. Cette proposition me paraît ainsi prématuré d'un point de vue législatif puisqu'elle précède des événements qui permettrait son enrichissement. j'émettrai quelques réserves sur la pertinence de plusieurs mesures présentées s'il est fondamental d'accélérer la réduction des passoires énergétiques le conditionnement des incitations financières aux rénovations performantes et global pourrait potentiellement déstabiliser le secteur. En effet, celui-ci est fortement soutenu par les dispositifs comme ma prime Rénov'ou encore les bouquets de travaux le rôle économique serait donc réduit et pourrait fragiliser les entreprises, dépendantes des subventions proposées par l'État. De plus cette proposition représente une contradiction avec l'objectif de massification des rénovations énergétiques, nous partageons tous l'opinion que le reste à charge des rénovations et frais pour les ménages désireux d'entreprendre ce type de travaux. L'institut de l'économie pour le climat estime ce reste à charge à 35.000 euros pour la rénovation d'un pavillon. Si le reste à charge est nul. C'est une idée louable mais il est nécessaire d'impliquer les foyers financièrement, chacun doit se sentir engagés dans la rénovation de son logement une contribution pécuniaire même minime permettrait cet engagement. Enfin, le principe d'extension de la durée de la rénovation énergétique jusqu'à six ans ajouterait de la complexité au dispositif et limiterait son efficacité. En effet, il est admis qu'une rénovation globale doit être effectué dans un délai limité. C'est pour cette raison que le règlement prévoit entre 18 mois et 3. Durée des travaux suivant la situation dans laquelle se trouve le logement concerné. Mes chers collègues, même si nous partageons l'objectif du texte, celui-ci intervient avant de nombreuses échéances sur le sujet de la précarité énergétique. Plusieurs mesures sont à retravailler car elle pourrait entraîner des conséquences problématiques, notamment d'un point de vue économique pour l'ensemble de ces réformes. Le groupe RDPI ne votera pas ce texte. Merci cher collègue.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, madame la rapporteur, madame la présidente de la Commission, monsieur le sénateur Cardon, auteur de cette PPL collègue de la Somme, à qui je souhaite un bonne anniversaire. Mes chers collègues Chacun reconnaît l'urgence d'une politique de lutte contre la précarité énergétique consubstantielle à celle de la rénovation thermique des logements dans un contexte de baisse de pouvoir d'achat et de hausse de prix de l'énergie. Si le mérite des auteurs de cette PPL dans réitéré la nécessité sa consistance déclarative et sa temporalité en limite son opérationnalité son efficacité. Eu égard le travail en cours de la commission d'enquête sénatoriale sur les politiques publiques en matière de rénovation des bâtiments et la loi de programmation quinquennale sur l'environnement et le climat avec son volet stratégie nationale bas-carbone à venir au second semestre. Résorber la précarité énergétique. Passe inexorablement par la résorption de l'insu L'insalubrité des passoires thermiques. À la croisée de l'urgence sociale qui a plus souvent recours à des aides modulable et rapide et de l'impératif environnemental de lutte contre le réchauffement, qui nécessitent des actions global et durable pour tous les types de logements et tous les types de propriétaire l'idéal de conciliation de ces 2 exigences heurte à la réalité. Les contraintes financières des ménages et la difficulté engager une rénovation globale avec l'urgence de certains travaux. Si avec les constats. Je partage l'important souligné de la PPL de favoriser l'accès au dispositif et de les améliorer, je suis plus réservé quant à l'extension de la durée pour pouvoir réaliser une rénovation globale et des capacités au reste à charge nul plus que les délais, c'est la détection et l'accompagnement des plus fragiles, qui est en cause la continuité des dispositifs comme le souligne le rapport de la Cour des comptes leur simplification et surtout les moyens humains et financiers mis en adéquation avec cette nécessaire massification ainsi que la coordination de tous les acteurs dont les collectivités locales qui joue un rôle majeur en ces domaines, ce sont plus de 12 millions de personnes dans une situation de fragilité et 5 millions de passoires thermiques qui nécessitent une rénovation indispensable mais coûteuse insuffisamment engagée en effet certains usagers ne parviennent pas à finaliser la demande de versement du solde ce qui induit le recours aux prêts bancaires, à la demande ou à des prêts familiaux souvent impossibles dans l'attente du versement des aides ainsi augmente la précarité financière de ces millions de ménages aux revenus modestes, voire très modestes. Cette discussion est aussi l'occasion de vous demander, monsieur le Ministre de prendre acte du rapport de la défenseure des droits qui a alerté sur les graves dysfonctionnements de. Outil dématérialisés en ligne. Ce sont 900 réclamations enregistrées entre octobre dernier et avril dont 600 qui restent encore sans réponse auprès de l'. Les collectivités se font le relais en saisissant Lana des situations individuelles. Mais elle se heurte à l'absence d'interlocuteurs parfois au délai hors norme dans le traitement des demandes qui lui sont faites. Faute de moyens nécessaires. La rénovation énergétique des bâtiments nécessite un pilotage économique et social pour aider les plus modestes. Un besoin de mobilisation de tous les acteurs sur le territoire, la nécessité de diagnostics territoriaux et individuelles, l'exigence d'un accompagnement tout au long du processus plus que de délai c'est l'accompagnement administratif, technique et financier avec l'engagement des collectivités aux côtés de l'État, via des subventions et des régies d'avance pour garantir l'efficacité des rénovations. La réduction de la précarité sociale et sanitaire comme vous l'avez signalé, Monsieur le Ministre et de l'économie d'émissions des gaz à effet de serre. C'est en ces termes que devra être décliné une véritable loi de réseaux de résorption de la précarité et de lutte contre le réchauffement climatique dans la future loi de programmation promise par le gouvernement. Poursuivons la commission d'enquête sénatoriale son analyse et les propositions des acteurs permettent un travail de fond indispensable aux adaptations législatives. Au vivre mieux dans un bien loger les personnes mal logées, sont de plus en plus nombreuses. Rappelons que dans son rapport annuel, la Fondation Abbé Pierre estime à 300.000 le nombre de personnes sans domicile fixe en France et 30.000 de plus qu'en 2022 et plus de 4 millions de mal logés les impayés de la fac de, de factures d'électricité ont augmenté de 17% entre 2019 et 2021. La question est donc de territorialisées et d'améliorer les dispositifs mais aussi d'articuler les acteurs pour produire des changements suffisamment rapide et permettre à notre pays de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050 et résorber la précarité énergétique et sanitaire des plus fragiles. J'en appelle aussi au gouvernement à prendre toutes les précautions à l'égard des plus vulnérables soumis plus que jamais aux arnaques sur les réseaux sociaux. Lesquels, par manque d'accompagnement peuvent souscrire des contrats malveillants. Ce qui serait la noyade dans la grande précarité. La PPL a proposé apparaît donc trop peu efficientes pour que nous puissions l'adopter mais permettra sur ses bases à leurs auteurs de nourrir les débats des lois prochaine attendu sur le sujet d'ici la fin de l'année pour atteindre ses objectifs. Merci cher collègue. La discussion générale est Close. La commission n'ayant pas élaboré texte nous passons la discussion des articles de la proposition de loi initial et a avant je vais donner la parole à même la présidente de la commission. Merci beaucoup madame la présidente. Je voudrais intervenir quelques instants puisque dans le début de ces propos. L'auteur de la proposition a remis en question le process de notre commission un petit peu caricaturer la position de la rapporteure. Je voudrais donc rapporte. Indiqué de 3 éléments vous redire ici. Cher monsieur car, donc nous sommes au sénat et que nous évitons les positions un peu trop caricatural pour préférer le travail de fond en général transpartisan et collégiale. Cela n'empêche pas les différences. Évidemment. Mais ces différences après ce travail transpartisan et collégiale se fait un peu plus dans le respect et c'est la raison pour laquelle la raison principale. Nous avons souhaité attendre le travail de la commission d'enquête qui est en cours. Par respect pour les sénateurs qui travaille et qui travaille beaucoup. D'autre part. Sans être désagréable, un certain nombre de dispositifs de votre proposition de loi était déjà satisfait soit peu opérationnel soit pour certains contreproductif et c'est l'exemple du CSCV du. Voilà et c'est la raison pour laquelle nous vous avons proposé aurait permis qui vous aurait permis d'être pleinement intégrés aux futurs travaux de notre commission et c'est donc avec regret mais avec respect pour votre décision que nous avons vous avons enfin je voudrais vous dire que les amendements étaient déposés par votre groupe les amendements, soit de la rapporteure, soit des autres groupes et notamment l'avis de la rapporteure sur les autres amendements étaient soumis à votre accord dans le cadre d'une d'un gentleman agrément et donc rien ne vous empêchait d'en déposer mais comme vous connaissiez notre proposition la rapporteure n'a pas souhaité être désagréable à votre encontre. Voilà un peu les dispositions que je voulais vous rappeler, non pas pour vous être désagréable, mais pour vous dire que vos propos été un petit peu exagéré un peu caricatural de la façon dont nous travaillons dans les commissions du Sénat. Merci. Si. Alors. Je vais mettre aux voix l'article. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public. Par la commission. Donc il va être procédé. il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Nombre de votants, 343. 338 %. Contre 237. L'article 1er n'a pas été adopté. Scrutin public sur chaque article. Est ce que je peux considérer que c'est même même vote. Donc article de même votre. Article 3 même vote. Alors pour l'article IV, mes chers collègues. Voilà je vais mettre aux voix donc l'article 4, cet article n'était pas adopté, je considérerais que le vote serait le même pour l'article 5 devenue sans objet. Cet article n'était pas adopté, il n'y aurait par ailleurs plus lieu de voter sur l'ensemble de la proposition de loi dans la mesure où les Saintes quartier qui la composent auraient été supprimés. Il n'y aurait donc pas d'explication de vote sur l'ensemble. Dans ces conditions quelqu'un demande la parole pour expliquer son vote sur l'article 4 je vais juste. Vous rappeler qu'à 20h 35. Je suis obligé de lever la séance. Non mais je vais vous le donner, je rappelle simplement non mais parce que s'il y a plusieurs personnes d'accord donc je vous donne la parole monsieur Cardo. Merci madame la présidente. Peut-être rebondir un peu sur les différents propos. Notamment de la rapporteure et de la présidente de la commission des affaires économiques effectivement la question. Ça a été soulevée à plusieurs reprises. Le contretemps je m'je m'en excuse mais vous vous êtes bien placé pour le savoir en quand on fait des choix dans les groupes ça ça tombe pas forcément dans le bon calendrier. Donc normalement elle aurait pu passer au mois de décembre, novembre dans une niche par. Niche socialiste bon là elle passe. En ce moment même, je suis désolée d'avoir froissé. certains égo sur ce sujet. Tout ce que je vois en tout cas, c'est que les voyants étaient au rouge. Tout à l'heure en cul âgé sur la question de la rénovation thermique apparemment du logement mais c'est pareil. C'est complémentaire, ça va avec. Et je vois aujourd'hui qu'en fait rien d'alarmant, tout va bien sûr on continue comme ça en même temps vous avez tous les indicateurs de la rénovation globale qui sont en baisse en 2022. Sur toutes les aides confondues et ça le midi. Monsieur le Ministre ne fait pas aucun commentaire, j'aimerais bien l'entendent parler, et puis, dernière question. À monsieur le ministre et j'en profite. Sur, Il y a une mise à jour en cours parce que Madame la rapporteure a flatté effectivement le le le logiciel logiciel étant mises à jour. Apparemment le, l'Observatoire national de la précarité énergétique. Attends une validation de d'un d'un montant total de 90.000 euros de financement pour pérenniser l'outil et pour le, pour le mettre en oeuvre dans les prochains jours auprès des collectivités et des différents acteurs concernés, donc est-ce que ça va être fait

Un vote sur l'ensemble n'est donc plus nécessaire puisqu'il n'y a plus de texte en conséquence la proposition de loi n'est pas adopté. je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 21h 50 pour le débat sur le programme de stabilité et l'orientation des finances publiques. La séance est suspendue.